J'informe le Sénat que les candidatures ont été publiés pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte commun sur le projet de loi actuellement en cours d'examen. Ces candidatures seront ratifiés si la présidence a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement 97 au sein de l'article 4. C'est Monsieur Touraine, qui le présente. Oui, Monsieur le Président merci. Il s'agit là de prendre en compte la situation des petites entreprises de 11 à 20 salariés, les organisations syndicales sont invitées par l'employeur à négocier le protocole d'accord préélectoral pour l'organisation des élections des membres du CSA, mais pour ces petites entreprises entre 11 et 20 salariés, cette invitation est conditionnée au fait qu'au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de 30 jours par cette disposition, l'implantation syndicale dans les d'entreprise est rendue plus difficile, en effet, l'entrée des organisations 5 syndicale dans les PME se faisait traditionnellement à l'occasion de la négociation des protocole pré-électoraux avec ce nouveau texte organisé ce les organisations syndicales n'auront plus à être averti de l'organisation d'élections, sauf dans le cas improbable où un salarié se soit porté candidat avant toute négociation d'un protocole avec les risques que cela comporte, c'est pourquoi nous vous proposons : la suppression de cet alinéa. Merci, cher collègue, l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur. c'est bien les rigidités d'assouplir le formalisme des obligations qui pèsent sur les petites PME l'ordonnance a prévu qu'un employeur de moins de 21 soit salarié ne doit d'enclencher le processus de négociation d'un protocole d'accord pas de pré-électorales, c'est-à-dire inviter les organisations certes syndicales représentatives localement dans la branche ou au niveau national à y participer que si l'un de ses salariés, a fait état de sa volonté d'être candidat aux prochaines élections professionnelles, cette mesure n'a pas pour but d'empêcher ces élections de se tenir mais bien d'éviter un employeur qui veut avant tout se consacrer au développement de son entreprise de gaspiller du temps de gaspiller des ressources dans un processus voué à aboutir à un procès verbal de carence, il faut au contraire salué le fait que le gouvernement a sur ce point tenu compte des contraintes qui pèsent sur les plus petites entreprises et conserver cette mesure. Monsieur le président : avis défavorable pour les mêmes raisons que le but n'est pas le but est de permettre un dialogue social efficace aux entreprises mais en étant très pragmatique sur la situation réelle des entreprises aujourd'hui très fortes carences et 80 Et. Aujourd'hui beaucoup les élections s'organiser en peu en pure perte, souvent les salariés eux-mêmes ne comprennent pas, c'est ce principe d'élection formelle dans les entreprises de moins de 20 salariés et et qui n'apporte rien, finalement, donc, même du point de vue des organismes syndicales, c'était pas un sujet pourrait l'essentiel puisque de toute façon ça ne ça fait 20 ans qu'on essaye cette forme-là et ça ne fonctionne pas, donc Jean-Claude, il faut rester sur l'esprit des ordonnances, je pense que le plus important, dans un texte pour il soit efficace et sa cohérence et donc en terme de cohérence, le gouvernement rend un avis défavorable. Merci madame la ministre, il y a pas d'explication de vote. Je peux mettre au voile amendement 97 qui a reçu un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour cet amendement. qu'on rentre. Qui s'abstient, il n'est pas adoptée. L'amendement 185 de la Commission, monsieur le rapporteur. Oui c'est président Luis agit en fait de dispenser l'employeur d'avoir à organiser des élections professionnelles partielle si l'élection de membres du CSE a été annulé par le juge en raison du non-respect par les organisations syndicales de l'obligation de respecter la proportion de femmes et d'hommes d'entreprises dans leur liste c'était disposition a été introduite par le Sénat dans la loi, Rebsamen de 2015, il convient donc de la rétablir. Merci madame la ministre. Même avec le rapporteur, Monsieur le Président. Avis favorable. Donc, mais aux voix l'amendement 185 avec un double avis favorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté, l'amendement 98 présenté par Monsieur Touraine. Oui, il s'agit de la condition émise pour être électeur dans une entreprise et devenir délégué du CSA pas devenir de éligibles et électeurs, alors il est indiqué qu'il faut être dans l'entreprise pendant 12 mois consécutifs, or de plus en plus de salariés sont utilisés en CDD. dans les entreprises et il se trouve de ce fait exclues de la marche de l'entreprise, alors que l'employeur lui a tendance à considérer que ce sont des personnels qui l'emploie de façon régulière et qu'ils font un peu partie de l'entreprise, c'est la raison pour laquelle il vous est proposé de modifier l'article en disant on serrant les mots continue ou discontinue. Merci, monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission sur cet amendement 98. Oui, je vais répondre sur l'amendement pas sur ce qu'a expliqué Monsieur Touraine, qui va, qui n'est pas directement liée à l'amendement les salariés mis à la disposition d'une autre entreprise, c'est-à-dire les sous-traitants aux prestataires peuvent voter aux élections professionnelles de l'entreprise au sein desquelles ils exercent leur activité après au moins 12 mois consécutifs de présence dans la maman en 98. Contrairement à plusieurs de leurs amendements précédant les auteurs de cet amendement 98 souhaite donc que cette réforme ne se fasse pas à droit constant, puisqu'il propose que ces salariés mis à disposition soit électeurs après 12 mois de présence continu ou discontinu dans l'entreprise, or jusqu'à présent, aussi bien pour les délégués du personnel que pour les comités d'entreprise, c'était bien une durée de 12 mois continue qui était requise en quoi ces conditions serait-elle plus excessive et manipulables aujourd'hui que par le passé, je ne sais pas, surtout que les gouvernements précédents n'ont jamais cherché à modifier dans les nombreux textes qui nous ont présentés sur le dialogue social, cette clause, donc c'est un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, madame la ministre.

sur la représentation des salariés, il y a 85 pourcent de compte rendu à durée indéterminée dans les entreprises et les partenaires sociaux, je comprends, sont très attachés à ce que, ce qui représente les autres salariés les représenter valablement c'est la perception des salariés, donc s'ils ont une connaissance récente de l'entreprise, ils sont pas forcément considéré comme représentatif, en revanche, où là vous pointez un sujet qui est vrai, il y a 15 pourcent des emplois qui sont des emplois intérimaires, CDD etc, qui est donc la personne physique, elle va passer de façon temporaire dans l'entreprise, mais le fait des conditions par exemple pour les CDD est une vraie question dans l'entreprise, c'est pour ça que nous avons souhaité dans les ordonnances, maître dans les nouvelles compétences des accords de branche, la possible, c'est une négocier sur la gestion de la qualité de l'emploi et notamment des CDD, oui il faut prendre en compte le fait qu'il y a sur les entreprises 10 à 15 pourcent d'emplois temporaires pour en tenir compte dans le débat social dans la discussion sociale par content, terme de représentation des salariés avec les partenaires sociaux, nous souhaitons rester sur ce qui a toujours été le cas, la représentation par des gens qui connaissent bien l'entreprise et sont connus de leurs collègues, et donc le représente valablement pour ces raisons, je donnerai un avis défavorable. Merci madame la ministre, il y a pas d'explication de vote. Donc je mais aux voix l'amendement 98 qui a reçu un double avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour.

Oui, l'article L. 2003 2314 tiré 33 dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017 tirer 1386 limite le nombre de mandats successifs à 3 soit un maximum de 12 ans avec des mandats d'une durée de 4 ans, les mandats des élus n'ayant pas nécessaire serment une durée de 4 ans, il convient de prévoir dans la loi le principe du dîner d'une durée totale maximale de 12 ans ainsi, ce n'est pas tant le nombre de mandats que la durée totale pendant laquelle le salarié à exercer un mandat qui importe. Gère collègues avis de la Commission, monsieur le rapporteur. de la dîme de la limitation dans le temps du nombre de mandats des représentants du personnel que la loi d'habilitation a fixé à mon initiative Alexis hâtive de la Commission, à 3. Il ne s'agirait donc plus justement de fixer cette limite à 3 mandats consécutifs, mais à 12 ans or si la durée de droit commun des mandats et de 4 ans, il est possible, par accord de fixer une durée plus courte, ainsi dans une entreprise où la durée des mandats serait de 2 ans, les élus pourraient effectuer ainsi 6 mandats c'est tout à fait contraire à la loi d'habilitation et à l'esprit de cette réforme, qui plus est, cet amendement réintroduit la possibilité pour les entreprises de s'affranchir de l'application de cette limitation par accord collectif que nous avons supprimé en commission n'a commission donc vie à l'avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, Madame la ministre. Oui, monsieur le président, je suis favorable à cet amendement donc défavorable au point de vue de la commission, pourquoi vous a, vous avez approuvé dans la loi d'habilitation et est ce que nous souhaitons faire c'est une limitation dans le temps des mandats, sauf pour les délégués syndicaux. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la démarche aussi que des élus du personnel et des représentants syndicaux puissent avoir aussi une carrière dans l'entreprise, la contrepartie de ça c'est effectivement tous les efforts qui vont être faits pour la reconnaissance de leurs compétences, leur formation prise depuis son reprend un métier quel est le but c'est aussi, et c'est aussi une demande assez forte dans les entreprises que il n'y a pas encore, entre guillemets, qui ne sera pas représentée que par des professionnels à vie, excusez-moi, mais par des gens qui vivent au pied les évolutions de l'entreprise, du point de vue de leur métier, de la même façon que leurs collègues mais on ne peut pas infliger la double peine et cela, il est vrai qu'au départ on avait pensé à 3 mandats parce que la moyenne est plus élevée et ce sont les organisations syndicales qui, à juste titre, nous faisons fait valoir que dans certaines entreprises, les mandats sont de 2 ou 3 ans, pour le coup, quand on a pensé ou 3 mandats, on pensait 3 fois 4 égale 12 et donc pour nous c'est important de pouvoir rester sur une logique de 3 mandats ou 12 ans ce qui dans les 2 cas, dit à peu près la même chose de bien faire des contreparties sur la formation, la compétence, la carrière des élus car je pense que et le dialogue social et les entreprises ce ce bénéficieront gens qui s'engage à fond pendant quelques années mais qui aussi peuvent avoir une perspective le futur mais je, je trouve que être pour le coup, un petit peu formaliste. Monsieur le rapporteur, vous me le permettrait, qui n'est pas votre habitude c'est un petit peu excessif dans ce cas-là, donc ce si je sais que vous ne pouvez pas faire un retrait, mais enfin bon si l'jovialité bien et donc personnellement, je suis au nom du gouvernement tout à fait favorable à cet amendement. Merci ma ministre monsieur Bourquin pour explications de vote. Oui, je, je suis un peu surpris par ce débat, on a l'impression que les délégués syndicaux font une carrière. On croit rêver dans dans combien d'endroits, on ne trouve pas de militants syndicaux. Dans combien d'endroits, les militants syndicaux lorsqu'il s'engage, ont eu des problèmes de carrière. Sont venus parfois devant des tribunaux pour faire reconnaître ce qu'ils avaient perdu en en émoluments. Parfois des il y a eu des jugements qui redonne des dizaines de milliers d'euros. Assez militant. Et là on voudrait et lorsqu'on parlait hier des des questions notamment de CHSCT sondés militants qui ont une connaissance très fine des questions, des conditions de travail, pourquoi vouloir leur limitées dans le temps. S'ils le veulent poursuivre, on dirait qu'il y a un foisonnement de militants syndicaux qui veulent faire carrière, c'est pas ça du tout être militant syndical dans une entreprise, c'est très difficile, je l'été, hein. C'est très difficile parce que sa carrière en prend un coup, parfois son salaire en prend un coup et on parle de 20 heures par mois. On parle de 20 heures par mois, alors pourquoi cette limitation cette limitation dans les ordonnances, est une erreur et inévitablement, ça apportera un coup très dur au jour ganisation syndical, je trouve que ce débat là est complètement surréaliste, au contraire, je pense qu'on a intérêt à avoir des militants syndicaux, former des militants syndicaux qui puisse aussi dans la durée en faisant bien leur travail, continuer à l'être et à défendent des intérêts matériels et moraux des salariés, j'ai l'impression qu'on est à, à des années lumière du véritable débat si les organisations syndicales n'ont pas le poids qu'elle devrait avoir, hé bien c'est parce que il n'y a pas assez de personnes qui s'engagent dans la vie syndicale, c'est pour ça que je ne comprends pas du tout ce ce ce comment cette limitation et je comprends Patricia Schillinger qui aujourd'hui a certainement eu parce qu'il y a des grandes entreprises qui sont Vairelles et qui ont dit : c'est pas assez et que va-t-on faire voilà, on est sur un débat qui risque d'affaiblir durablement les organismes, les merci Monsieur le Président, juste quelques mots pour pour dire que Madame la ministre et vous, mon cher confrère, avait dit à peu près la même chose finalement, quand on dit faire carrière c'est pas faire carrière dans le monde syndical, je ne pense pas, c'est le risque quelque part quand on s'implique comme complètement délégué syndical dans la, le travail syndical dans l'entreprise, de perdre le lien, parce qu'on on s'occupe des autres salariés, etc, de le lien avec son travail et de le risque de de ne plus y arriver après donc la possibilité, j'ai fini la 20 heures mais c'est parfois plus content prend du temps qu'on se donnait complètement et on prend du du du recul, je trouve très intéressant de parler de 12 ans et non pas de 3 mandats grâce ou à cause de ça donc vous les les 2 propose se ressemblent. Donc si chers collègue Monsieur Grand pour explication de vote. Oui, Madame le Ministre, je me permets de vous demander ce qu'on est en train de débuter la le futur débat sur la réforme constitutionnelle parce que, effectivement, nous sommes à peu près sur les mêmes principes, c'est-à-dire, finalement, on ne touche à la liberté des élus car les délégués syndicaux sont des élus, moi je suis gaulliste et le et et la liberté syndicale, c'est dans nos gènes, hein, depuis la Libération, pas moi, je n'étais pas, rassurez-vous, donc je je me pose quand même une question sur cette affaire, je me demande si, là, on va pas trop loin, est-ce que demain on va va la réforme institutionnelle, maître des barrières aussi aux reconduction ministériel est-ce qu'on va dans le temps est-ce qu'on va aussi mettre une barrière à l'Otan des 2 secrétaires généraux des syndicats pour dont certains sont restés longtemps et qui n'entrerait pas dans le cadre est-ce que c'est plus dangereux d'avoir un emploi, secrétaire général de syndicats qui reste 15 ans ou un délégué syndical dans une entreprise qui reste pas trop longtemps est-ce que ce n'est pas la lune demande peut-être du MEDEF de plus vouloir de devoir changer un petit peu les têtes car les élections de leur conviennent pas je, peut-être qu'on s'étonne que je dise cela, à partir de ces dans la mais pour moi il y a des moments où, quelles que soient les bons, il faut savoir s'exprimer avec le coeur et et et une responsabilité qui est la nôtre et celle d'élus locaux qui connaissent parfaitement le le problème et qui demain vont connaître de graves difficultés, ne pourront pas cumuler sur un certain nombre d'années de mandat parce que Madame là aussi on touchera, vous le verrez au coeur de la démocratie, parce que dans les plus petits villages dans les plus petites communes, les élus, finalement, abandonneront ils auront peut-être raison merci. Merci, cher collègue. Madame polluants pour explication de vote. IgE adhère une certaine partie ce que vous avez dit mais je pense qu'il y a quand même une différence importante entre autres les mandats syndicaux des mandats politiques, mais en tout cas sur ce qui concerne les mandats syndicaux, effectivement, je crois que on est dans une situation où on serait plutôt en en situation d'encourager l'engagement syndical et l'engagement au service des, des, des, des autres personnels dans les entreprises, et moi je m'inquiète beaucoup de l'après, parce que quand même quand on est élu dans un CE dans un CHSCT quand on représente le personnel, on a des droits, on est un peu salarié protégé, même pas qu'un peu. Et moi, je crains que, à à, quand on arrive au bout du mandat auquel on ne pourra plus se représenter, hé bien il y a un certain nombre de pression qui puisse s'exercer et que la liberté syndicale là soit entravée aussi je je suis relativement inquiet par rapport à cela et je je vous demande, Madame la Ministre, quelles garanties pouvez-vous apporter pour que cumulent enfin de ce cumul dans le temps ne viennent pas la fragiliser les représentants syndicaux, surtout lorsqu'ils arrivent au bout de ce type de du nombre d'années, c'est une question très importante, à mon sens. Merci, cher collègue Monsieur Touraine presque question de vote. j'ai bien entendu Monsieur Grant et je partage la quasi-totalité de son propos, sauf, sauf une partie. Qui laisse entendre et parce que c'est pas la première fois, non plus que la remarque a été faite consiste à dire : il y a pas de raison que pour les délégués syndicaux, il y a pas une limitation du nombre de mandats, puisqu'on nous impose à nous, élus politiques d'être limité, moi je voudrais pas que l'amertume qui est la nôtre qui transparaît dans ses propos, nous fasse subir à d'autres ce que nous regrettons, je trouve que ça nous ça nous grandirait pas et ce ne serait pas très nord, donc c'est c'est pas une raison, me semble-t-il, a invoqué pour justifier de la limitation des mandats 2ème observation j'bien entendu aussi que vous laissez entendre dans votre grande bonté que la limitation des mandats, c'est plutôt pour eux, c'est plutôt pour préserver les délégués syndicaux pour qu'ils ne se retrouvent pas en situation difficile, à la fin de leur mandat, laissez-moi douter un petit peu et surtout laissez-moi penser qu'ils ont, ils ont suffisamment de responsabilités pour décider de leur sort et savoir s'il doit se représenter ou pas pour autant. La dans les ordonnances, on prévoit la limitation des mandats, et on n'indique pas le temps. Et donc, madame la ministre, vous avez raison de préciser que les les accords de branche peuvent indiquer décidé que les mandats de du Roy, entre 2 ans et 4 en or 3 mandats : 2 ans ces 6 ans ça ne laisse pas le temps. De l'expérience a n'est-ce pas le temps de la compétence, ça ne laisse pas le temps de la maîtrise des dossiers, le patron, il aura la maîtrise des dossiers parce qu'il sera présent et sera tout le temps là nous avons voté à des amendements qui demandait où nous l'avons dit qui demandait qu'il n'y avait pas cette limitation, mais je vais voter l'amendement de Madame Schillinger pour éviter le pire. Merci, cher collègue Monsieur pour explication de vote. Merci Monsieur le Président, Madame la ministre, chers collègues, moi je partage un certain nombre de remarques qui ont été faites ici. Je crois que cet amendement, je ne dis. Parlons ici du cadre de vie de l'entreprise, une entreprise, c'est une direction c'est des salariés, c'est des savoir-faire et des machines-outils, c'est tout ça à l'entreprise et on peut se poser la question de savoir pourquoi tant de salariés ne s'engage pas dans le syndicalisme. C'est une vraie question : pourquoi. Parce que beaucoup, ils subissent la répression syndicale. être syndiqué dans un groupe par exemple de la grande distribution, parce que j'en ai rencontré beaucoup, notamment de jeunes femmes s'engager dans la grande distribution, c'est se voir demain imposer des horaires qui ne pourrait pas être conforme avec un code de vie familiale, c'est parfois être. Mon collègue Martial l'a dit, c'est voir des avancements de carrière stoppée Net, combien de cas comme cela. Moi je crois que être syndiqué, aujourd'hui c'est le héros, je le dis comme ça, parce que s'engager pour son entreprise pour ses collègues parfois dans cette ambiance de répression syndicale, il faut avoir du cran aujourd'hui pour se syndiquer, souvent dans des entreprises, souvent de PME, des petites et moyennes entreprises où parfois il y a pas de syndicats, et je crois que avec cet amendement on va pas résoudre le problème, et ensuite on va pas favoriser le syndicalisme, on va plutôt, à mon sens le décourager et puis dernière chose mais notre collègue l'a si bien dit, je crois que c'est aux salariés eux-mêmes de décider qui peut les représenter le mieux et je partage en 6 ans, on fait du travail, mais parfois on n'a pas fini son travail pour passer le rôle, et parfois il faut 10, 15 ans, et les syndicats, les salariés sont eux-mêmes les plus intelligents pour parfois passer le rôle, et donc on ne votera pas cet amendement qui, à mon sens va décourager le syndicalisme plus que l'encourager. Merci, cher collègue Monsieur Bachere pour explication de vote. Oui, monsieur le président, moi j'ai d'accord avec le président de la Commission sur l'île sur sa position, il veut paraît assez logique conditions on a choisi de limiter à 3 fois. C'est ce que la loi prévoit donc. Certes, certains mandats sont 2 ans. Il est bon, peut-être, d'inciter les branches comme il a été dit par certains collègues à passer à 4 ans, à ce moment-là pour gagner en compétences. Mais la modeste expérience qui est la mienne, dans les entreprises consiste plutôt à avoir, j'allais dire parfois un syndicalisme professionnel très professionnel et un éloignement du domaine du travail et du secteur du travail de plus en plus importants alors ce qui est important, c'est peut-être de faire des passages comme parfois pour la politique. On travaille, on prend un mandat on retravaille on change et ça permet de revenir à des réalités parce que, dans nombre d'entreprises, il faut le dire très clairement, les syndicats aujourd'hui et je réponds à mon collègue gay juste juste avant moi, sont totalement déconnectés du monde du travail, alors ils sont peut-être très compétent en terme de droit du travail et c'est heureux, mais alors ils sont totalement déconnectés du de du domaine du travail et donc ça crée de la désaffection vis-à-vis des syndicats et donc c'est parce que je veux avoir des syndicats forts parce que je veux avoir des entreprises où les employées connaissent le travail que je soutiens la position de mon collègue, président et rapporteur. Merci collègue Monsieur Chassaing pour explication de vote.

personnel ira peut-être vers plus de syndicats, c'est ce qu'on peut espérer bon en ce qui concerne cet amendement pour le le nombre de mandats si vous voulez effectivement le le nombre d'années de mandat est de 12 ans ça me paraît pas quelque chose d'assez important je, moi je, je voterai cet amendement. C'est cher collègue Madame Cohen pas, explications de vote. Oui, je vais être très bref parce que beaucoup d'arguments ont été ont été développés mais je m'étonne parce que depuis hier, on parle de dialogue social et en même temps Madame la ministre dit depuis le début qu'elle fait confiance aux partenaires sociaux. Et tout à coup on veut imposer dans la loi, hé bien une règle concernant les délégués syndicaux, c'est-à-dire celles et ceux qui défendent les salariés, alors faut savoir c'est quoi le dialogue social et favori, ce qui, dans une entreprise. Et là encore, pardonnez-moi de, de souligner et de ne pas partager du tout comme l'ensemble de mon groupe que finalement donc ces ordonnances ça va toujours dans le même sens savait toujours pencher la balance du côté des 2 directions et en faveur des salariés, des salariés qui vont défendent leur outil de travail, les conditions de travail et là on va encore rajouter une règle qui valide brimés et je pense que ce que je défends la dans l'hémicycle et on l'a bien vu notre collègue et est sorti mais ce qu'il a ce qu'il a dit en en en en justifiant d'ailleurs les les arguments qu'il donnait en disant qu'il était un gaulliste et qu'il avait une haute conception de la démocratie etc, même très nombreuses et nombreux à le partager donc cet cet amendement on va dire adoucir un peu les choses, donc nous au niveau de notre groupe, on ne va pas voter contre, mais on va s'abstenir parce que là, si vous voulez, c'est quand même terrible que dans l'hémicycle on soit conduit à dire finalement on va faire ça parce que c'est moins pire. pire. Chers collègues, Madame la ministre. Juste une précision pour que avant de Woitier souhaitions sur de parler tous exactement la même chose : d'abord, les délégués syndicaux ne sont pas concernés par cet article, les délégués syndicaux, il n'y a pas de limitation dans le temps des mandats des délégués syndicaux, donc ça c'était ni dans le telles et ordonnances ni dans l'amendement de la commission dont on parle d'elle d'autres élus du personnel sachant que les délégués syndicaux peuvent être élus ou désignés comme vous le savez, donc, donc il ne s'agit pas des délégués syndicaux 2ème sujet la question c'est, et est pas dans habitué, je l'avais dit et je le redis, la question, une des questions que nous 10 organisations syndicales sur la difficulté d'engagement, donc en tant qu'élu sous les différentes formes, c'est que beaucoup de de jeunes ou moins jeunes se disent une fois que j'ai pris un engagement, je peux pas revenir en arrière, je risque effectivement d'être pénalisés dans ma carrière, dans ma rémunération, ce qui, dans un certain nombre de cas, il au moins un minimum ça ralentit je peux et puis je suis pas sûr j'arriverai, on nous demande de me projeter dans la longue durée, voilà, donc je crois que là il y a un sujet quand même qui est que la longue durée est antinomique avec la capacité de continuer une carrière non pas d'élus mais de reprendre son métier et le faire progresser, alors ce qu'on fait là-dessus, ce qu'on veut faire, c'est la mission que j'ai confiée à Dominique Simonpoli et GIAT effectivement aller beaucoup plus loin sur la valorisation des compétences, moi ça me fera beaucoup dans les entreprises, l'expérience été voilà quoi, été élu du personnel qui était ouvrier, employé, ont développé des compétences assez extraordinaire d'organisation de management de conviction de négociations parce qu'on développe des compétences qu'on a un mandat qui se sont engagés pour les autres et pour la collectivité et puis finalement quand ils arrêtent leur mandat, on leur propose finalement de revenir à la case départ, ça ce n'est pas correct et c'est dissuasif de l'engagement sur ce mandats donc sur ce sujet-là, qui n'est pas l'objet de l'amendement, mais je le dis parce que c'est un une cohérence d'ensemble, c'est très important qu'on avance sur ces sujets de d'avenir professionnel

au départ, il est vrai dans l'ordonnance, je le reconnais, nous avions prévu 3 mandats et nous avions sous-estimé le fait qu'il y avait beaucoup de mandats qui était moins de 4 ans effectivement, là ça peut revenir à limiter à 6 ans et là, ça nous paraît vraiment excessif car le temps développer ne pour le coup, d'incompétence, autant ça peut être un piège pour une carrière de faire toute sa carrière, je parle pas des délégués syndicaux donc élu du personnel toute sa vie professionnelle, autant il est clair que limitée à 6 ans nous paraît excessif, donc nous avons, c'est ce que propose amendement c'est d'aller jusqu'à 12 ans, la commission de le souhaite pas, mais vu la discussion, je pense que sur beaucoup de bancs, vous allez voter l'amendement parce que je pense que certains avec conviction et d'autres en disant que c'est moins pire. Mais en tout cas si je vais même être être faites ce que vous voulez mais vous êtes chez vous et rapporteur alors ce qu'on a prévu d'néanmoins. Je le redis, parce que ça, ça a pas été dit dans la discussion, en-dessous de 50 salariés il y a pas de limitation, parce que là il y a un problème de trouver les par dans des plus grandes entreprises au contraire que les mandats puisse tourner soit pas toujours les mêmes va aider à développer cette culture de négociation, cette culture de la représentation sur un un nombre de salariés plus important et puis par ailleurs, nous avons prévu, et ça, la Commission veut le supprimer que par accord majoritaire dans l'entreprise en plus aller de au-delà de cette limite de 3 mandats et 12 ans donc c'est aussi dans le l'amendement que propose rapporteur qui me paraît trop restrictif du développement syndical. Si Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur une attention très court. oui, oui, oui Monsieur le Président, moi je voulais juste ajouter d'abord j'ai j'ai des sentiments très quand même que dans l'ensemble des discussions qui ont eu lieu la plupart d'entre nous sommes d'accord pour dire que celui qui doit limiter le nombre de mandats dans le temps, un élu, c'est celui qui vote ou qui ne votent pas pour lui mais pas obligatoirement le gouvernement ou la loi, c'est le 1er point le 2ème point l'amendement, il est présenté par Madame chien parle évidemment de cette durée, donc on a suffisamment parlé mon type omis de dire aussi la madame la ministre vient de redire que par accord d'entreprise, les entreprises peuvent s'affranchir de cette limitation à 3 les a donc à ce moment là c'est même plus la peine de le dans la loi, donc je je confirme mon avis défavorable. Très bien, alors je vais mettre aux voix, je leur l'amendement 159 qui a reçu un avis défavorable de la commission, un avis favorable du gouvernement qui est pour. Levez bien la main parce que.

Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adoptée. L'amendement 186 de la Commission, monsieur rapporteur. Monsieur président c'est amendements rédactionnels qui vise à réaffirmer l'obligation introduite en commission de former l'ensemble des élus de ces ce aux questions de santé, sécurité et pas uniquement les membres de la commission dédiée. Merci madame la ministre. Monsieur le président, c'est une effectivement une suggestion et un vote de la commission que je trouve intéressant parce qu'il est cohérent avec ce que j'ai évoquée hier, quand nous avons eu un débat très intéressant sur la santé au travail quand je disait que la santé, la sécurité, les conditions de travail doit être l'affaire de tous et pas simplement de la commission spécialisée même si ont un rôle utile de d'approfondissement, ça va dans ce sens-là et ça serait c'est assez cohérent, je trouve, avec notre idée que pour faire de la prévention faut que tout le monde soit à bord sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail, ce qui demande un minimum de formation sera peut-être pas une formation aussi poussée que pour les membres de commissions et que tous les membres du CSE est une formation ces sujets me paraît une bonne initiative, judo, gouvernement, donc un avis favorable. Merci madame la Lamy. Donc jamais au voilà amendement 186 avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour.

ce qu'on observe dans ses ordonnances et que, par petites touches, on fragilise quand on les supprime, pas pour les entreprises plus petites, soit les, les, les, les instances représentatives du personnel, en les fusionnant en enlevant un certain nombre de prérogatives, soit en fragilisant les élus comme on vient de le voir lors du précédent débat et là autre petite touche puisque il est prévu que l'employeur n'a plus de non-maximum de collaborateurs pour assister avec lui aux réunions de l'instance mais il peut, il peut s'entourer de gens avec lui parce que, il dirige l'entreprise a pas forcément connaissance de tout dans le détail, etc, mais quand on est salarié, représentant du personnel dans des instances où on doit essayer de convaincre, mais essayer de participer et essayer de construire mais aussi s'opposer. Si on a en face de soi un nombre très important, important de gens qui entoure l'employeur pour des salariés qui n'ont pas forcément l'habitude de s'exprimer en public, ce sont autant de choses qui rendent l'expression des salariés plus difficile, c'est la raison pour laquelle on avait auparavant un nombre limité de collaborateurs, autour de l'employeur que nous proposons donc de rétablir, afin de permettre à à ce que l'expression des. Salariée dans ces instances puissent être pleine puisse être entière quand on se retrouve avec son responsable Direct, hé bien c'est peut-être plus difficile de s'exprimer, le le le. Sens de cette proposition, qui je crois va dans le sens d'une de de rendre ces instances constructive et qui va donc dans le dialogue social, et qui essaye de limiter cette fragmentation par petites touches, cette fragilisation du pouvoir et des capacités d'agir des représentants de du personnel. Merci, cher collègue, monsieur le rapporteur de l'avis de la commission. Merci Monsieur le Président, en fait, la l'amendement de notre collègue à abaisser de 3 à 2 le nombre de collaborateurs qui peuvent assister l'employeur qui préside c'est je pense que les les compétences de nouvelles instances sont bien plus étendues que celles du comité d'entreprise et notamment donc on l'a dit tout à l'heure, on l'a vu dans l'amendement président en matière de santé en matière de sécurité au travail qui relevait jusqu'à présent du CHSCT est donc logique sur ce point en particulier de faire évoluer le droit est de permettre à l'employeur de disposer d'un collaborateur spécialisé sur ces questions, donc nous sommes défavorables, nous pensons qu'il vaut mieux rester à 3. Merci madame la ministre. je pense qu'on peut débat des 2 la portance c'est que, de part et d'autre, les personnes qu'il faut pour discuter et donc je me remettrait à la sagesse du Sénat. Merci, même taille pour explications de vote. Oui, pour préciser qu'il n'est aucunement question de limiter à 2 personnes qui souhaitent toutes les mêmes à chaque point de l'ordre du jour de l'instance, il est tout à fait possible et cela se fait que lors d'un sujet particulier l'employeur demande à aux préventeur de risques professionnels de devenir quand il s'agit d'un sujet à ce qui a trait à la finance, de l'entreprise, on fait venir voilà donc 2 ça permet à l'employeur d'être correctement entouré ne de ne pas fragiliser la voix des des salariés. Merci donc je mais au voilà Mandement 139 qui a reçu un avis défavorable de la Commission invite sagesse du gouvernement qui est pour.

Testament, l'ancien président, qui vise à préciser la nature des engagements pris par l'employeur dans le règlement intérieur du CSE et les conditions dans lesquelles il peut dénoncer sur la base de la jurisprudence de la Cour de cassation. Merci mon ami. Oui, Monsieur le Président, le gouvernement est favorable à cet amendement qui consiste à codifier une jurisprudence établie de la Cour de cassation, c'est quand même plus sympa pour les employeurs, comme le syndicat de salariés il il s'agit des obligations un peu ailleurs, le code du travail, faut déjà il y accéder, on va essayer de le rendre plus lisible par le code numérique mais alors il faut pas regarder tous les accords, les arrêts de la Cour de cassation, donc je pense que l'appartement ou la jurisprudence établie qu'elle correspond à une pratique qui convient au législateur mieux de codifier. Merci donc je mais aux voix l'amendement 193 de la commission avec un avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté. L'amendement 140 Madame taillé pour Merci Monsieur le Président Madame la Mini, cet amendement a pour objet de rétablir la présence de représentants aux fonctions spécifiques en matière de santé et de sécurité dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés qu'est-ce qui peut légitimer le fait, alors que dans ces que ces entreprises plus petites, il n'y a pas d'instance spécifique au moins de commissions spécifique avec une spécialisation des représentants on sait tous, et ça a été dit développé hier parfois tard mais que que que que c'est que ces représentants spécifiques, il y avait des connaissances des connaissances à la fois techniques à la fois humaines aussi des situations de travail dans l'entreprise était indispensable pour faire vivre la prévention des risques professionnels dans l'entreprise, donc nous proposons cela afin de effectivement de dans ce que dit Madame la Ministre-ce à droit constant, la prévention des risques professionnels, on n'a rien perdu, si beaucoup de salariés vont y perdent. Merci, chers collègue monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président, voilà un amendement, donc il y a baisse de 300 à 50 salariés le seuil d'effectif à partir duquel la création d'une commission spécialisée en matière de santé, sécurité et des conditions de travail est obligatoire au sein du, c'est ce que lui confère la personnalité civile, ce qui lui permettrait notamment de rester en justice, il part cet amendement du postulat erroné,

qu'il est possible dans le créer une par accord collectif dans les entreprises de plus petite taille, je ne pense pas que l'absence de cette commission dans les entreprises de taille moyenne, empêche les membres du C. se de se spécialiser chacun sur les questions pour lesquelles ils ont une appétence particulière, il pourra s'agir de la santé au travail, ou bien des problématiques financières de l'entreprise, selon la façon dont les élus décident de s'organiser, par ailleurs, je suis opposé à la commission aussi à ce que la Commission. Dédiée soit dotée de la personnalité civile émettent elles-mêmes des avis c'est contraire à l'esprit de la réforme qui repose sur la création d'une instance unique de représentation du personnel, cela reviendrait à en recréer une seconde surtout je pense que c'est un facteur de qualité des avis émis que de permettre à l'ensemble des membres du CCE de se prononcer sur des questions de santé, de sécurité, de travail, ils ont chacun leurs expériences propres en la matière et sont à ce titre légitimes pour se prononcer sur ces questions, je pense par ailleurs, je tiens par je tiens par ailleurs rappelé que pour cette raison, la commission a rendu obligatoire la formation de l'ensemble des membres du CSE aux problématiques de santé, de sécurité et des conditions de travail et pas uniquement celles celle des membres de la commission, c'est donc un avis défavorable. Merci madame la ministre. C'est le président, un avis défavorable en cohérence avec ce que j'ai dit hier et tout à l'heure sur des sujets de santé sécurité de conditions de travail, je voudrais rajouter que ce serait complètement contradictoire de recréer une sous-commission qui qui a une personnalité morale alors que justement fusionnent pour créer une seule personnalité morale et quelle est la vue d'ensemble de l'entreprise, mais je rappelle que cette commission est déjà obligatoire pour les entreprises de moins de 300 salariés pour les établissements quoi sensibles, c'est-à-dire tout ce qu'on une installation nucléaire ou classée Sévéso que l'inspecteur du travail peut imposer la création d'une telle commission lorsqu'il y a des sujets spécifiques liés à la nature de l'activité ou l'agencement l'équipement des locaux et puis surtout, vous venez de rendre obligatoire la formation pour tous les membres. Du CSE et le CS dans ses compétences doit au moins 4 fois par an consacrés entièrement consacré ses travaux sur les sujets de santé, d'hygiène et sécurité au travail, donc il est faux de dire que ce sujet ne sera plus traité ou pas assez bien traitées. Donc je pense que cette amendement n'est pas nécessaire et même contre contraire je dirais contradictoire avec ce que nous voulons faire, et donc le gouvernement, un avis défavorable. Merci madame polluants pour explication de vote. Oui, bon, je confirme qu'il est certainement contraires à l'esprit des ordonnances, cet amendement, vous dites que il reste il reste dans les entreprises dites sensibles, effectivement, mais dans beaucoup d'entreprises, il y a des situations de travail qui sont sensibles, sans pour autant relever de la réglementation Sévéso etc, par ailleurs, vous dites qu'il faut fusionner parce que il y a, il faut une vision globale pour traiter des questions de santé et de sécurité au travail mais justement il ne faut pas laisser d'autres considérations rentrer en ligne de compte quand on parle de santé et sécurité au travail dans ces instances, parce que sinon on le, on finit toujours par les négligés et les salariés n'ont qu'un corps protégeant le Silvouplay. Et ne faisons parce que quand on a des, des, des élus qui vont avoir toutes les autres considérations et d'autres appétence comme vous disiez, hé bien la panthère facile de négliger les questions de santé et de sécurité au travail, surtout lorsqu'elle ne présente pas un caractère grave un caractère dangereux imminents lorsqu'elles sont plus diffuses, alors on les oublie et c'est la raison pour laquelle ces instants spécifiques était incomparable en terme de d'efficacité, de prise en compte de prise de conscience de situations de travail qui provoquait. Des dégâts sur la santé des salariés, donc pour toutes ces raisons, bien entendu, il est essentiel, il serait essentiel de notre point de vue effectivement en contradiction avec les l'esprit des ordonnances de, de, de, de prendre en compte ces dispositions prévues dans cet amendement. Merci, cher collègue Monsieur Savary pour explication. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la ministre n'est bon là surtout pas là-dessus, c'est le principe même de l'intérêt de la loi contre rien lâcher, nous discutons avec des salariés ou des chefs d'entreprise sur le terrain, on voit bien que l'intérêt l'Avantage qu'ils ont trouvé à travers les propositions travers vos ordonnances c'est véritablement de faire en sorte qu'il est plus de souplesse, c'est ce qu'il nous dise davantage instance représentative, que ces entreprises sont sensibles au problème de santé, c'est la meilleure façon d'avoir une meilleure compétitivité pour l'entreprise de faire en sorte qu'un bn être au milieu de ses collaborateurs qui puissent épanouir à travers le travail donc plus, le problème est moindre : plus on le prend en considération à travers la souplesse à travers la volonté d'chacun quand il est grave, bien sûr, tout le monde, face à un problème grave, on va prendre des mesures, mais c'est trop tard, ce niveau de la prévention qu'il faut agir et on voit bien que, en ayant des actions de prévention volontaire le dynamisme des entreprises, elle sera plus performantes que d'autres et les salariés voudront travailler dans celles où il y a une protection de leurs droits à une protection également de des conditions de travail par rapport à celles qui n'offrent pas parallèlement ces mêmes conditions, donc je pense que c'est un un, un moment important de la loi sur lequel faut rester particulièrement ferme. Merci, cher collègue Monsieur Touraine pour explication de vote. vote. Quiconque a eu l'occasion d'ériger un un établissement d'importance dans lequel il y avait un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, c'est l'enthousiasme. L'engagement des membres de ses comités, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont été, qui, s'ils ont une mission particulière qui leur est propre et ils ont une responsabilité à l'égard de l'ensemble des salariés alors. Bien sûr qu'ils sont casse-pieds. Tout le tout directeur tout chef d'établissement, c'est bien, c'est bien que ce sont des aiguillons qu'il vous amène des problèmes que vous auriez mieux aimé ne pas voir parce que ça va induire des modifications ça va induire des dépenses supplémentaires oui mais. Combien de mots ont été ainsi éviter combien de maladies combien de handicap, combien de difficultés pour les salariés. On a pu éviter par par ses En vous écoutant, je me dis. Que nous sommes au fond, d'accord, vous êtes d'accord sur le fait que ça va réduire la dilution à l'intérieur des c'est ça va réduire la capacité d'intervention en matière de santé et de sécurité si puisque vous essayez d'apporter des palliatifs vous le le rapporteur nous dit : ah oui mais dans certaines entreprises, ils pourront le faire, donc, puisqu'ils peuvent le faire, on peut se contenter de cela, pourquoi est-ce que ça n'est pas dans le droit commun tout à l'heure, vous nous avez dit par dérogation, on peut avoir plus de 3 mandats, pourquoi ne pas le faire rentrer dans le dans le droit commun, donc il y a un aveu chez vous un aveu implicite du fait que vous savez pertinemment que

Oui, monsieur le président, même la Mini chers collègues on on n'auditionnait ce matin le numéro 2 de Lactalis et dans les interventions qui se sont, qui se sont produites il y a eu un rapport qui a été fait et il y a eu plusieurs articles dans la presse spécialisée sur le fait qu'en ayant mis par exemple Lienemann Ajman dans cette entreprise, il aurait pu avoir des problèmes concernant la sécurité alimentaire. C'est un une question à regarder de près, le parquet est saisi, on verra sur ce problème, comment ça se passera mais les délégués du personnel. Les délégués du personnel et du CHSCT avait mis en garde la direction sur ces questions. Tout à l'heure monsieur le rapporteur, disait, ben il y aura pas moins d'attention sur les questions de sécurité au travail bien sûr que si. Bien sûr que si moins de personnes, nous sommes un seul organisme. Bien sûr que si, il y aura moins d'attention alors que les questions de santé au travail, se pose avec une acuité particulière qui nous a pourquoi, bah parce que il y a un facteur qui produit des textes régulièrement les questions de haute se pose avec aussi acuité et donc on a besoin au contraire de mettre l'accent sur les questions de la santé au travail des pays scandinaves, notamment le font mieux que nous, il y a aussi, on parlait de l'Allemagne, hier, qu'il le fait avec beaucoup d'attention et en fait un élément de productivité au travail et donc je ne comprends pas très bien cette volonté de s'opposer à tout ce qui se met en place aux propositions qui sont faites, notamment sur cet amendement pour essayer de remédier et de traiter mieux la question de la santé au travail, dernière chose. J'ai peu de temps, j'ai vu qu'on proposait, on a refusé tout à l'heure, les 12 ans et surtout on veut limiter, je me suis posé la question, Madame la Ministre, vous êtes pas posé la question de limiter le temps des PDG à la direction des entreprises, mais une question comme ça, sous forme de boutade mais sachez bien que beaucoup de syndicats disparaîtront parce que ils ne pourront plus avoir de délégués qui merci, cher collège chez par la limitation des mandats. Si j'ai un collègue Madame Schillinger pour explication de vote. Oui, nous, notre groupe a naturellement soutenir Madame la ministre, elle a, elle, a bien expliqué les choses en disant que quand même des choses fausses qui ont été dites donc on peut pas tout entendre les attributions du CHU n'ont pas disparu, elles ont été transférées au CSE, qui continuera à jouer un rôle de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi qu'améliorer la que leurs conditions de travail et en plus, le texte a prévu la possibilité le même l'obligation dans les entreprises, établissements d'au moins 300 salariés de créer. Une ou plusieurs commissions entièrement conçu. Sacré aux questions de ses de santé et de sécurité, de conditions de travail, le fait est-ce devra se réunir également. Au moins. 4 fois par an, sur ces sujets de santé, de sécurité, de conditions de travail, donc moi je pense qu'on a bien expliqué, moi, je voterai contre l'amendement. Merci, cher collègue Monsieur Vatrin pour explication de vote. Oui nous voterons cet amendement de repli, parce que il est suffisamment porteur mais peut-être pas aussi ambitieux que nous le souhaiterons, mais je pense que il faut d'abord dire que la santé au travail était un n'éléments d'Eternit déterminant du niveau de santé, on est dans l'impro, dans une société où le vieillissement va prendre de plus en plus de place, bon c'est pour beaucoup sur le lieu de travail se détermine

par exemple quelqu'un qui a exercé une fonction de professions libérales et et un ouvrier à la production, dans une entreprise, donc c'est pas seulement question économique, une question sociale, c'est une question sociétale qui est posée et c'est l'intérêt de la société dans son ensemble, de prendre toutes les mesures pour prévenir le vieillissement précoce pour prévenir les invalidités pour prévenir les accidents du travail, pour prévenir les maladies professionnelles, je crois qu'il y a beaucoup à faire et au lieu de réduire les possibilités de prévention ne pense au contraire qu'il faut les augmenter en plus madame la Ministre, savait très bien que du que vous le voyez, ou non, en reportant le débat sur les questions de santé au travail bien sûr dans une commission, mais plus largement en les fondant dans le comité économique et social, vous faites défendre dépendre des questions de santé au travail, plus largement, de questions stratégiques de l'entreprise, donc ces questions d'organisation du travail, ces questions liées à l'impact par exemple des Restructuration à l'impact de suppressions d'emplois, par exemple, vont se trouver noyés dans des débats stratégiques sur le devenir de l'entreprise et donc, il nous semble que c'est quelque part diminuer la portée même des débats nécessaires sur les questions de prévention au travail, alors pourquoi je disais en introduction, c'est un amendement de repli, parce que, effectivement, si les CHSCT dans leur fonctionnement actuel n'était pas toujours satisfaisant, parce qu'il manquait de moyens, c'est parce que souvent, le médecin du travail n'était pas présent ou l'inspecteur du travail n'était pas présent, merci, merci Jean-Claude les supprimer, améliorons le système. Je suis désolé, je suis pour le respect du temps de parole de chacun et je rappelle aux orateurs que il faut respecter ce temps de parole donc surtout pour 2 minutes et demie on attend quand même de dix piqué son son vote Madame Fournier pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, écoutez, je voudrais quand même réagir sur ce qui a été dit et concernant principalement ce CSE sur lequel je ne reviendrai pas, j'aimerais quand même vous réaffirmer chers collègues qu'il serait temps de faire un peu confiance aux chefs d'entreprise, ce sont des personnes responsables, de même que les personnes qui les entourent, comme les DRH, sachons-le, de toute façon si le personnel se sent bien dans son entreprise, il va y travailler correctement, donc ça c'est une remise en question, que je souhaiterais qu'on ne fasse plus, il faut qu'on évolue et qu'on arrête d'avoir ce langage parfois un peu archaïque pour ramener simplement le positionnement au niveau des salariés que je respecte tout à fait d'un d'ailleurs, ceci étant, en terme de prévention pour les les salariés de santé, je voudrais revenir sur mes propos de la discussion générale, en fait, si l'on veut que ses salariés soient bien protégés, je préférerais faire faire appel à la professionnalisation de la médecine du travail, nous avions dit avec madame la ministre que nous attendions, dans les mois à venir, une refonte totale de cette médecine du travail, je préfère, si vous le voulez bien faire confiance à des professionnels pour la prévention de ces salariés, ceci étant, je vous dis-je, nous voterons et bien sûr contre cet amendement, merci.

ces 3 instances sont transférés avec la totalité de leurs prérogatives, pourquoi la sécurité, la santé au travail qui est très importante, pourquoi elle serait minimiser pourquoi le C. S. minimiserait la santé au travail, donc je ne crois pas du tout, donc c'est pour ça que je voterai contre cet amendement. Merci, cher collègue, donc je vais mettre au voile amendement 140 qui a reçu un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour cet amendement. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté l'amendement 142 Madame taillé polluant.

qui a pour objet de restreindre la possibilité pour l'employeur d'être assistés en réunion de collaborateurs en nombre tels qu'ils seraient ensemble aussi nombreux que les représentants titulaires avec le risque, les représentants des salariés siègent en face de leur supérieur hiérarchique, voilà, sinon, comme j'ai expliqué précédemment bah, écoutez, c'est une risque d'entrave d'auto-censure des salariés qui va immanquablement arrivé dans certaines entreprises, il n'est pas du tout question de dire que les employeurs sont méchants. Il n'est pas non plus question de stigmatiser, il faut donner des cadres pour que. La santé des salariés qui est un bien précieux, évidemment, pour les salariés eux-mêmes irremplaçable qui est effectivement nécessaire et important car meilleure santé au travail dans une entreprise, c'est une meilleure productivité soit garantie parce qu'on le sait quand même un certain nombre d'employeurs ne font pas l'effort, on le sait, et c'est bien pour ça que des CHSCT ont été crées, donc il faut pas jeter l'opprobre sur l'ensemble, mais il faut quand même reconnaître et voir la réalité en face et certains scandales sur la santé au travail, l'ont montré, certains employeurs ne font pas le minimum certains, hé bien il faut garantir pour tous : colloque les garanties soient là et que le minimum soit fait et même le plus possible, c'est la santé des Français qui est en question. la mode par cet amendement d'interdire carrément à l'employeur d'avoir des conseillers techniques lors des réunions concernant évidemment la santé, la sécurité et conditions de travail, la commission est défavorable. Madame la Ministre. Le gouvernement est défavorable à cet amendement, je rappelle aussi que les membres de la commission santé-sécurité, conditions de travail puisqu'ils seront nécessairement désigné au sein du CSE il bénéficie associé du statut de salarié protégé qui favorise et protège leur liberté d'expression pleine et entière au sein de la commission après ce sont il y a souvent des sujets techniques qui sont, qui sont discutées ce qui est déjà le cas d'ailleurs dans la. Comme dans les CHSCT toujours incertain de nos collaborateurs techniques qui sont là, ça ne change pas le la nature du débat, je crois que ce qui est important, c'est la liberté d'expression pleine et entière et le statut de salarié protégé le garantit. Merci madame la ministre, donc jamais aux voix l'amendement 141 avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est quand Qui s'abstient, il n'est pas adopté l'amendement 187 monsieur le rapporteur de la commission. Un amendement qui une coordination président avec la décision qui a été prise en commission de maintenir le caractère obligatoire de la commission des marchés dans le sait : ce n'est plus important. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le président, effectivement la la Commission souhaite corriger sur ce point-là l'ordonnance qui avait plutôt penser que le CSE pouvait s'organiser pour ces travaux, ceci dit, je comprends aussi la logique de votre amendement qui encourage à une transparence, faisant référence à des règles connues de tous, je me remets à la sagesse du Sénat. la mise. 100 87 ans que l'amendement 187 je le mais aux voix qui, avec un avis de sagesse du gouvernement c'est l'amendement de la commission qui est pour. Qui est contre.

il s'agit là de dans un souci de simplification et afin de permettre à même financements pour toutes les entreprises et donc le bénéfice de tous les salariés donc, nous vous proposons à travers cet amendement de fixer le montant de la subvention de fonctionnement versée par l'employeur au comité social et économique, quel que soit le nombre de salariés dans l'entreprise à 0,22 dans ce pays les salariés des plus petites entreprises sont souvent beaucoup moins favorisées que dans les grands, nous venons d'avoir un débat sur la prévention des risques, nous, nous proposons donc d'aligner pour le fonctionnement de du comité social économique. Merci, monsieur le rapporteur pour la commission. Oui, c'est un amendement de qui vise à porter de 0 2 à 0 22 pourcent de la masse salariale à subventions de fonctionnement du CSE versée par l'employeur dans les entreprises comptant entre 50 et 2000 à 2000 salariés, ce qui est le niveau auquel cette subvention était porté par l'ordonnance dans les entreprises d'au moins 2000 salariés il n'est pas démontré que ce niveau soit insuffisant pour permettre aux sessions de remplir ses missions, le reliquat des moyens consacrés aux activités sociales et culturelles peut par ailleurs désormais être reversé au budget de fonctionnement L accord collectif peut également prévoir un niveau plus élevé, en revanche, la commission ne semble pas, ne pense pas souhaitable de faire peser sur les entreprises de taille moyenne, une charge sur financière supplémentaire à elle a donc émis un avis défavorable. Monsieur le Président, toujours cohérence du texte, je crois qu'à la fin, il faut qu'on ait un discours clair aux entreprises comme aux salariés, c'est une les ordonnances pour le renforcement du dialogue social, ont mis l'accent sur le fait très opérationnel, dans le contexte des petites et moyennes entreprises augmenter la charge

des entreprises amène de fait expériences mais permet de constater un besoin de nombres d'expertise surtout d'ampleur d'expertise qui est beaucoup plus grand, donc là c'est, c'est la raison de cet abondement dans les grandes entreprises qui n'est pas cessé nécessaire dans les petites entreprises où les sujets sont beaucoup plus facilement après rentable. Donc c'est un avis défavorable aussi donc jamais aux voix l'amendement 155 avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour.

Oui, il s'agit de supprimer l'sur l'article IV des alinéas 40 41 44 et 45 les dispositions de ces 2 alinéas porte atteinte à la liberté du comité social économique de disposer. De ses propres fonds, si nous sommes hostiles au principe de cette fausse humilité et il est évident que dès lors qu'elle est rendue possible par les ordonnances, elle doit être complète l'interdiction de transfert est une disposition, que l'on peut qualifier de perverse puisqu'elle n'implique que le CSA pour que l'employeur prenne en charge les frais d'expertise. il aurait dû ne pas transférer d'excédent annuel du budget de fonctionnement sur les activités sociales et culturelles durant les 3 années précédentes, de plus, si l'employeur prend en charge des frais d'expertise, le CSA ne pourra opérer de transfert durant les 3 années suivantes, ce qui pourrait pénaliser le financement des activités sociales et culturelles destinées aux salariés, dans ces conditions, ne risque-t-il pas de renoncer à des expertises, madame la ministre, vous avez dit tout à l'heure qui n'était pas au port. Tadeusz surcharger le le budget des entreprises vous n'avait pas hésité malgré tout à charger le budget en lui imposant de financer 20 pourcent du coût de certaines expertises.

le même contenu de l'amendement, elle est excellemment défendu, nous pensons qu'il y a une forme de de chantage là qui est mis en en place qui est insupportable, donc nous défendons cet amendement en ce sens. sens. Cher collègue Monsieur Touraine les amendements 101 et 100. Alors pour le sang, un homme a laissé entendre en commission que la sollicitation été satisfaite, donc je le retire. Et

du droit à l'expertise, tous ceux qui ne reçoivent aucune somme mobilisables puisque leurs moyens de fonctionnement leur sont donnés en nature par leur employeur et tous ceux dont la taille trop petite Laurent impossible tout cofinancement, je prends l'exemple dans une entreprise de 100 salariés peu qualifiés au sein de laquelle le salaire brut annuel moyen est de 20000 euros et le la masse salariale brute de 2 millions d'euros donne le montant de subventions de fonctionnement sera de 4000 euros cette subvention modeste de 4000 euros vote être largement utilisé par la Documentation l'information, les déplacements, l'informatique ou encore la téléphonie et Internet en prenant l'hypothèse qu'un maximum de 10 pourcent de cette subvention puisse servir à rémunérer une expertise, cela fait un budget de 400 euros étant donné un cofinancement à hauteur de 20 pourcent cela signifie que le budget d'expertise, avec la participation de l'employeur sera de 2000 euros, un montant très faible qui montre bien que ce droit à l'expertise ne sera plus opérationnel par cet amendement, nous vous proposons une dispense de cofinancement en fonction de la taille de l'entreprise ou du montant de la masse salariale. Merci, cher collègue, l'amendement de la commission de 194 monsieur le rapporteur. Oui merci Monsieur Président l'acide amendement relatif à la simplification des modalités de recours à l'expertise par le service et des types d'experts, il supprime notamment la notion d'experts techniques qui n'avait jamais été véritablement défini et confirme que les experts seront désormais habilités par un organisme d'accréditation comme le coffre et non plus agréé par le ministère du Travail, ce qui permettra de garantir leurs compétences. Merci, monsieur le rapporteur, donc l'avis de la commission sur les 4 amendements, discussions communes, puisque le sang a été retiré. Alors le 99 c'était une il propose d'un suppression des règles encadrant l'utilisation du service par le CCE d'excédent de son budget de fonctionnement à l'Assemblée nationale, le gouvernement à compléter le disposition issues de l'ordonnance qui fixe désormais comme principe que le CSA devra participer à hauteur de 20 pourcent à la prise en charge du coût de certaines expertises orientations stratégiques d'entreprise consultations ponctuelles ponctuelles sauf PSE et risque grave dans l'établissement afin de tenir compte des situations où son budget de fonctionnement sera insuffisant pour apporter cette participation financière dans ce cas, l'employeur devra financer l'intégralité de ce coûte toutefois pour s'assurer que le CSA ne mettra pas en place une stratégie de diminution artificielle de ces moyens pour ma campagne a systématiquement à contribution cette prise en charge a été conditionné à l'absence de transfert de l'excédent du budget de fonctionnement aux activités sociales et culturelles durant les 3 années précédentes, de plus, si l'employeur est amené à financer la totalité d'une expertise à ce type de c'est ce ne pourra pas procéder à un transfert au cours des 3 années suivantes, les auteurs de cet amendement veulent supprimer cette disposition en affirmant qu'il s'agirait d'un moyen de faire diminuer le recours à l'expertise par le CSE, je pense que c'est une fois encore faire bien peu confiance aux élus du personnel, leurs missions premières reste d'émettre des avis sur les projets non pas ailleurs, avant d'assurer la gestion des activités sociales et culturelles, bien peu responsables de leur part, de favoriser l'arbre de Noël de fin d'année au détriment des expertises nécessaires aux consultations ponctuelles dont ils sont saisis, chacun son tour Monsieur 3, par ailleurs, je tiens à rappeler que la possibilité de reverser aux vous avez laissé l'excédent du budget de fonctionnement est une nouveauté introduite par l'ordonnance, il n'est donc pas ici question de revenir sur des pratiques anciennes ou de changer des habitudes bien établie, c'est donc un avis défavorable à l'amendement 33.

C'est le président oui alors d'abord je voudrais revenir au pourquoi notre débat, c'est parce que nous avons introduit dans les ordonnances, la possibilité d'une fragilité dans le sens vers les actions sociales et culturelles, pourquoi, parce qu'aujourd'hui, ont constaté que dans beaucoup de c'est ce il y avait un un budget de fonctionnement qui n'était pas entièrement utilisé, il ne pouvait pas être transféré aux activités sociales et culturelles, donc le point départ ces 2 permet de libérer ces sommes qui sont bloqués quelquefois pendant des années sur des grandes autres c'est quelquefois des millions d'euros qui sont bloqués pendant des années, on ne peut rien faire et dont les bénéficiaires ne sont pas les salariés, donc le problème départ ça a été d'adresser cette possibilité de fonds jubilent IT excédent de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles,

annulé la mesure précédente donc ce qui avait été prévu ce que vous venez par vos amendements au c'est le fait qu'il ait une limitation de sorte fauchés, c'est que il faut pas que ça Vienne supprimer cette ce cofinancement, sauf bien sûr dans les coques par ailleurs prévu aussi, c'est que dans les petites entreprises, s'il n'y a pas assez de financement pour l'expertise à ce là l'employeur. Prendra entièrement à sa charge, ce qui est l'esprit mais pas la Lettre de l'amendement 100 parce qu'on n'a pas voulu sur un seuil précis mais qui est plutôt une évaluation au cas par cas, donc en résumé ce que je dis c'est que Bordeaux ce que nous souhaitons, c'est dans les heures, dans ce confirmer ce dans la loi ratification ce principe qu'il puisse y avoir une fragilité comme un excédent de fonctionnement 2 qui ne puisse pas se faire au détriment de la codécision sur certains types d'expertise exceptionnelle que nous avons prévu, et donc c'est pour ces raisons que je serai le gouvernement sera défavorable aux amendements 99 33 et 100 qui traite du même sujet par ailleurs sur l'amendement 194 qui est, je dirais une réécriture et une amélioration des créatures, je le reconnais, pour les sur les interventions d'experts, je le gouvernement un avis favorable. Merci Monsieur Touraine peut, explications de vote. juste un petit mot. Vous dites : Madame la Ministre, au fond, nous avons été très sensibles à la situation nécessaires, ils avaient de l'argent en caisse, nous les autorisons à utiliser cet argent à utiliser une partie de l'excédent pour des d'autres activités, pas seulement des armes de Noël, mais aussi des activités culturelles, sportives, voire sociales. Mais en même temps vous nous dire oui on leur fait un cadeau, mais il va bien falloir quand même qu'il y a une contrepartie, qu'on fasse payer puisque d'une part, vous mettez à leur charge si vous mettez à leur charge 20 pourcent du coût des expertises dont il n'avait pas avant, et d'autre part vous ne pendant 3 ans s'ils n'ont pas fait d'excédent, ils auront droit à une prise en charge totale, mais s'ils ont une prise en charge totale pendant 3 ans et ne pourront pas utiliser l'excédent éventuellement dégagés pour des activités sociales ou culturelles, je trouve que c'est un moyen de pression que vous utilisez, c'est pas une générosité de votre part, trouve que. C'est pas bien. Donc, je vais mettre aux voix les amendements, discussions communes l'amendement 99 tout d'abord, qui a reçu un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour.

l'amendement 100 même vote. Même vote et sur l'amendement 194 la commission avec un avis favorable du gouvernement qui est pour.

créée par l'ordonnance 2017 Tiret 1386 du 22 septembre 2017 prévoit ceci, je cite, un accord d'entreprise ou, à défaut, un accord conclu entre l'employeur et le comité social, économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel détermine le nombre d'expertise dans le cadre des consultations sur une ou plusieurs années ainsi donc il sera non seulement possible de déterminer à l'avance le nombre d'expertise dans le cas des consultations sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise ou la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, sur une ou plusieurs années c'est article remet donc en question le droit des représentantes et des représentants du personnel à expertiser les décisions prises par la direction, alors vous me direz, est-ce que c'est aussi fondamental ce ce droit l'expert. Nous pensons que c'est un droit important et d'autant que, finalement, on le voit au fil des propositions qui sont contenues dans ces dans ces ordonnances, y compris d'un d'un certain nombre d'amendements pour parfois aller plus loin, mais pas le sont pas dans le sens de l'intérêt des des salariés, c'est une remise en cause des droits des représentantes et des représentants donc pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article. Merci, monsieur le rapporteur pour la commission. Merci Monsieur Mélenchon à Laurence Cohen que l'ordonnance permet en effet aux partenaires sociaux dans l'entreprise de s'entendre à l'avance sur les pratiques qui seront sollicités dans le cas de consultation récurrente contrairement aux consultations ponctuelles, il est en effet possible de les anticiper si leur périodicité n'a pas été modifié par accord comme l'ordonnance permet le CSA devra donc se prononcer chaque année sur les orientations stratégiques stratégiques de l'entreprise, sa situation économique et financière et sa politique sociale sur 3 cas de recours à un expert, il n'est pas déraisonnable de fixer ce nom par accord collectif des consultations ponctuelles n'étant évidemment pas concernés par ce sujet, donc c'est un avis défavorable à l'amendement. Merci madame la ministre, pour le gouvernement. Monsieur le président : avis défavorable du gouvernement également, encore une fois, il faut bien comprendre que c'est d'abord une possibilité résultant d'un accord d'entreprise ou d'un accord entre l'employeur, le CSE donc les représentants du personnel doivent consentir consomme, c'est qu'il a un intérêt à le faire, et cette négociation, en outre, comme c'est le rapporteur a rappelé ne peut se faire que pour les consultations récurrent du ce sur lequel on peut programmer l'idée c'est de programmer un rythme

imprévisible qui arrive entreprise donc je crois que ça ne permet au contraire d'associer plus en amont, d'avoir le temps de réfléchir sur les expertises qui vont être faites passer commande d'un train d'expertise programmée et cela contribuera le dialogue social, économique, construit dans la durée sans rien restreint de. Décès du recours à l'expertise ponctuelles ou en urgence autour de ces éléments nouveaux qui font l'objet des expertises ponctuelles. Merci mamie. Donc je mais aux voix l'amendement 34 avec un double avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté l'amendement 142 Madame taillé polluant. Merci, cet amendement a pour objet d'de financement des expertises concernant les projets importants défini à l'article L. en effet, la disposition risquait de priver certains c'est ceux de leur capacité à l'expertise sur des questions importantes, notamment sur des projets d'ampleur qui permettent d'anticiper et d'éviter des problèmes sur la santé au travail, ultérieurement, donc il nous semble vraiment dommage on n'logique de prévention, de fragiliser le recours à ces expertises par les les CSE voilà d'où la proposition de cet amendement. Merci, monsieur le rapporteur. Merci Monsieur président c'est ces expertises projets importants entre dans le cadre de celle qui des consultations ponctuelles du CSC doivent être prises en charge à hauteur de 20 pourcent par cette instance, elles n'ont pas un caractère d'urgence ou de danger qui justifierait leur financement complet par l'employeur, comme c'est justement le cas des expertises commandées en cas de risque grave dans l'établissement, toutefois, l'employeur prendra bien en charge l'intégralité du coût de cette expertise, dès lors que le budget du CSE ne le permet pas, et que ce dernier n'a pas au cours des 3 dernières années un éventuel excédent à ses activités sociales et culturelles en ce sens, aucun c'est ce ne devrait être privé de son droit à l'expertise, à l'exception peut-être de ce qui, à l'avenir, préféreront leurs compétences sociales sur leur compétence consultative avis défavorable de la commission. Merci Marie. Monsieur Monsieur le président, c'est un avis défavorable je crois que bon, tous les ingrédients de la réponse ont déjà été évoquée à plusieurs reprises dans le débat précédent tout je ne reviens pas dessus. Merci madame pour explications de vote. Effectivement, ces expertises ne rentre pas dans le cas de l'urgence, au sens où il y aurait un danger grave et imminent, ont cependant elle sainte, elles doivent s'intégrer, elles peuvent s'intégrer dans le cas de projets de réorganisation et quand un employeur et on comprend bien, et c'est tout à fait légitime souhaitent mener un projet de réorganisation, il a pas envie d'attendre l'année prochaine que le CSA et les moyens de le faire, donc je pense que c'est pas une question d'urgence et une question d'opportunité à le faire au moment du projet où on peut encore je dirais faire en sorte qu'ils prennent en compte davantage les questions de conditions de travail de prévention des risques professionnels, donc de le prendre au bon moment, ça c'est pour la raison de l'pour la problématique de l'urgence ensuite lorsque le budget ne permet pas, mais parfois on peut avoir un budget qui le permet, mais parce qu'on est dans le cas des CSE ou les problématiques des conditions de travail, la santé au travail ne sont plus les l'unique prérogatives, on peut avoir d'autres priorités, avec des élus qui n'étant pas spécialiste des et des conditions de travail vont préférer organiser un certain nombre d'activités socio-professionnelle etc vous préférez mettre leur budget sur la dessus, alors vous allez me dire : c'est donc ce ne sera pas suffisamment important, il y a aussi ce sera quand même suffisamment important, mais on revient toujours au risque de dilution des problématiques pourtant essentielle de la prévention des risques au profit d'autres problématiques sont très importante aussi, mais qui doivent être traités à part du CSE. Merci, cher collègue donc jamais aux voix l'amendement 142 avec un avis défavorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement qui est pour.

puis contre. Qui s'abstient, il est adopté, l'amendement 35 monsieur. Le nouvel article le 23 15 80 du code du travail prévoit désormais que plusieurs expertises ponctuelles devront être financés à 20 par le comité, social, économique, alors qu'elles aient auparavant pris en charge par le l'employeur l'expertise restera c'est vrai intégralement pris en charge si cette consultation porte sur la politique sociale et les conditions de travail et d'emploi, sur un projet de licenciement collectif pour motif économique d'au moins 10 salariés sur une période de 30 jours et enfin si elle porte sur un risque grave constatée dans l'établissement en revanche dans les autres cas, et notamment lors de consultations récurrente sur les orientations stratégiques de l'entreprise ou de consultation ponctuelles demander à telle ou telle moment il est prévu que ceux qui en font la demande y contribue à hauteur de 20 pourcent l'entreprise y participant L à hauteur de 80 pourcent alors que les syndicats sont confrontés à des employeurs qui viennent accompagnés des meilleurs experts le projet de loi réduit donc la capacité d'action, des représentants des salariés, c'est pourquoi nous demandons la suppression de cet aliment. Oui, merci Monsieur le Président, donc l'instauration d'un cofinancement à hauteur de 20 pourcent du coût des expertises demandées par le se, dans le cas de certaines consultations ponctuelles ponctuelles vise avant tout à responsabilisés mais représentant du personnel non à les priver de leur droit de faire appel à un expert de plus, cette règle ne s'appliquera pas si budget de fonctionnement du CSU je redis est insuffisant pour couvrir ce coûteux comme l'a prévu l'amendement gouvernemental adopté à l'Assemblée nationale sur ce point, l'employeur prendra alors en charge l'intégralité de la rémunération d'experts, c'est donc un avis défavorable de la commission. Merci madame la ministre. Avis défavorable, je crois que le sujet. Donc jamais aux voix l'amendement 35 avec un double avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté l'amendement de la commission de 196 monsieur rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président, en fait, cet amendement rétablit une exception à la règle selon laquelle le conseil d'entreprise négociera les accords d'entreprise, qui figurait dans l'ordonnance d'origine mais a été supprimée par l'ordonnance 6, or certains accords sont soumis à des règles de validité spécifiques notamment d'unanimité qu'il convient de préserver.

parce que c'est ça revient à détruire le conseil d'entreprise, la différence entre un comité social, économique et un conseil d'entreprise, c'est justement la capacité de négocier sur tous les sujets, le conseil d'entreprise donc il appartient ou la fonction de délégué syndical, au sens du pouvoir de négociation en complément des autres qui avait un pouvoir d'information consultation se retrouvent dans le conseil d'entreprise, c'est évidemment cette instance qui a le pouvoir de négocier sur l'ensemble de sujets qui est compétent pour négocier avec les règles, les règles de majorité habituelle, mais qui sera compétent pour négocier, donc votre amendement revient à supprimer la différence finalement entre comité social, économique et conseil d'entreprise, donc je suis un retrait parce que je pense que c'est un mauvaise compréhension entre nous.

et représentant les salariés, les franchisés, or la mise en place de telle ou telle instance, nous sommes en totale contradiction et le principe même de la fragile puisque chacun fragilisé était un entrepreneur indépendant lié par une contrat de distribution avec le franchiseur, je répète, la franchise repose sur une totale indépendance du franchiseur et du fragilisé ainsi quand on est fragile, la commission des affaires sociales avait souligné à l'époque, il n'est pas possible d'imposer à l'employeur de chercher à reclasser en cas de licenciement économique ne salarié chez un peu fragilisé avec lequel il n'entretient aucun lien juridique ou économique, ou de permettre un hypothétique et délégué syndical de réseaux de fragilise d'accéder à une entreprise dont il n'est pas salarié, c'est pourquoi nous proposons de supprimer la mise en place d'une instance de dialogue social dans les réseaux de fragiles. Merci madame la Lamure pour le 176 rectifier. Oui, merci Monsieur le Président, cet amendement propose également la suppression de la mise en place d'une instance de dialogue social dans les réseaux de franchise, car cette disposition remet en cause le statut de la franchise, le franchisé était un commerçant indépendant du franchiseur et qui encourt les mêmes risques économiques et supporte les mêmes responsabilités juridiques: qu'un entrepreneur non franchisés d'ailleurs cet article a été déclarée partiellement contraire à la Constitution, en raison de l'atteinte disproportionnée qu'il représentait à la liberté d'entreprendre. Merci, cher collègue, l'avis de la commission sera porteur. Alors sur le 171 rectifier bis je partage et la Commission partagent le point de vue des auteurs de cet amendement, cette instance est pour le moins atypique dans le mauvais sens du terme, en effet, elle crée au sein d'un réseau de franchise, un lien entre le franchiseur, les salariés de ses franchisés, alors qu'il n'existe aucun lien de subordination de ces derniers envers lui le franchiseur ne saurait être tenu pour responsable, donc des choix faits en matière d'organisation du travail par ses franchisés, la relation qu'il entretient avec eux étant de nature purement commercial, notre commission à l'initiative de Jean Manga abouti qui était alors son rapporteur avait supprimé cette disposition lors de l'examen de la loi travail et le Sénat avait partagé la position de de Jean-Marc Butty, par cohérence, donc la commission a émis un avis favorable à l'amendement de monsieur Wauquiez l'amendement 171 rectifier bis. D'accord, ils sont identiques, donc c'est les 2 amendements et un avis favorable, Madame la Ministre, l'avis du gouvernement. l'avis du gouvernement est défavorable parce que pour nous ça n'entrait pas dans le choix, le Champ de la loi d'habitation que vous nous aviez donné, c'est un sujet qu'on n'a jamais évoqué. Non, il y a même pas osé le le bordel ça c'est exact Deuxièmement, par ailleurs, c'est une disposition pour le aujourd'hui qui a bac à notre connaissance, n'a été sollicité par personne connaît est un peu virtuelle donc elle est aujourd'hui elles gênent pas l'action parce qu'elle, elle a été en mis en place nulle part, c'est pas une raison sur le fond, mais je veux dire le degré d'urgence du sujet et comme ce n'est pas dans le Champ de la loi d'habitation un avis défavorable à l'instant T, parce que je vois pas pourquoi on aujourd'hui. Merci madame la ministre, donc je mais au roi les 2 amendements identiques 171 rectifier Bisson 176 rectifier avec un avis favorable de la commission analyse défavorable du gouvernement qui est pour.

Monsieur. Merci monsieur le président, cet amendement vise à renforcer la représentation des salariés dans les conseils d'administration, celle-ci en effet très insuffisante en France car limité aux seules grandes entreprises en comparaison en Allemagne, les salariés représentent un tiers du conseil d'administration pour les entreprises entre 500 et 2 1000 salariés et la moitié des sièges dans les très grandes entreprises, il est ici proposé de s'inspirer du fameux modèle allemand en garantissant aux salariés, un tiers des sièges des conseils d'administration des entreprises, madame la ministre, vous présentez souvent la codécision comme un modèle pour l'entreprise pour pour y parvenir, il faut commencer par an de forcer la présence des salariés et de leur organisation partout y compris dans les instances décisionnaires où s'élaborent les modalités de gestion et la stratégie des entreprises, les salariés ont beaucoup de choses à dire notre amendement propose de transformer le plafond actuel en le seuil plancher cette disposition constitue réel saut qualitatif indéniable en termes de représentation des salariés dans les oncles, les organes de décision des entreprises et participerez de la bonne gestion des années qui était collectifs de long terme de l'entreprise. rendant tout obligatoire dans les plus grandes entreprises, la présence d'administrateur représentant les salariés dans les conseils lustration les entreprises pouvaient déjà de leur propre initiative en accueillir, cet amendement vise donc à à rigidifier cette possibilité en disposant que l'entreprise ne pourra plus le faire que si ses représentants composent au moins le tiers de son conseil d'administration, voilà une proposition qui est de nature à décourager les entreprises qui n'ont pas d'obligation en la matière, d'expérimenter en ce sens, si à terme elle pourrait décider d'augmenter le nombre d'administrateurs salariés elles souhaiteront sans doute mettra en place progressivement cette représentation, la commission a donc émis pour l'instant un avis défavorable. Merci madame la ministre. à la fois le droit et les mentalités évoluent au fil de temps ce qui est vrai c'est que c'est la loi travail de d'août 2015, qui a abaissé le seuil admis les seuils à partir duquel est duquel il y a des représentants, membre du conseil ne sera ration à 1000 salariés et elle se met en oeuvre depuis quelques mois parce que c'était applicable à partir de fin au 2ème semestre 2017 avec cette loi, la France c'est à notre connaissance, le 2ème, pays le plus avancé en Europe, à part l'Allemagne que vous avez hésité sur la participation, je parle pas des représentants du personnel, qui siège au CA en plus mais d'administrateurs salariés, donc c'est un débat que nous avons qui a été amorcé pendant les concertations avec les partenaires sociaux qui avaient été d'ailleurs abordée rapidement monde la loi d'habilitation aujourd'hui les questions qui sont posées sur de plusieurs ordres. Il y a le sujet. Des femmes dans l'Ecosse admiration pour les sociétés non cotées, puisque maintenant, la loi est arrivée à son terme, il y a bien 40 pourcent de femmes dans les sociétés cotées, mais ça ne la situation qui est posée, il y a la question des administrateurs salariés qui est une question à la fois quantitatives qui est une question qualitatif, car il y a des débats sur les conditions d'exercice car pour pouvoir être au conseil d'administration, il faut évidemment avoir. Une. Pour éviter tout risque de délit d'initié il y a une confidentialité des débats, ce qui fait que dans certaines organisations syndicales y a débat sur le fait que, du coup, un administrateur salarié, hé bien il n'est plus vraiment en contact, vous êtes en tout cas, elle ne peut pas donner d'informations à son organisation, donc, même au sein des organes asocial organisationnel calme il y a débat, ensuite il y a cette mise en 9 dans les entreprises au-dessus de 1000 salariés, on commence à avoir pas mal d'entreprises de taille intermédiaire patrimonial, où il y a souvent que 2, 3, 4 membres au conseil de gouvernance de comment ça va se mettent en place, ça aussi c'est nouveau et enfin. Il y a le il y a un sujet. Sur les les champs qui n'étaient pas couverts dans cette loi, puisque cette loi avait, par exemple, économie sociale et solidaire, paradoxalement, considérant qu'étant déjà dans une logique paritaire n'avait pas besoin de d'administrateurs salariés supplémentaires mais donc il y a débat là-dessus aussi, sans compter que les entreprises, j'aurais fait le tour de la question à statut remplir l'échappent à cette réglementation, tout ça pour dire que ce n'est pas une chose qu'on. Décider. sur le bien d'un abonnement, sans avoir fait le tour de la question et c'est pour ça que dans le cas de la mission que j'ai confiée avec à Nicole Notat et Jean Domecq Sénart avec Bruno. Maire Nicole Belloubet et. Tous là Hulot nous avons posé cette cette question de la gouvernance fait partie des sujets qu'ils étudieront, mais j'ai, j'ai fait juste une liste de questions, voyez que rien que la liste des questions, elle est assez grande, et donc avant d'avancer une étape loin, c'est pour ça que nous avait paru prématurée dans les Ardennes, les ordonnances sont au moment où cette loi qui s'applique maintenant au-dessus de 1000 salariés est en train de s'appliquer, on n'a pas le recul dessus mais surtout, il faut faire le tour de l'ensemble des questions avant de procéder à un niveau. L'aménagement législatif qui si oui se trouverait dans le cadre du projet pacte au printemps prochain, donc pour toutes sortes raison je pense que il est prématuré de se poser la question sous forme d'un amendement et donc le gouvernement, un avis défavorable. Kim illustre donc ce jeu mais aux voix l'amendement 38 avec un double avis défavorable à commission et du gouvernement qui est pour.

Merci Monsieur le Président, oui j'ai j'ai bien entendu la réponse de Madame la ministre, à l'instant et qui, pour partie, à mon avis va valoir en réponse aux amendements que je présente à cet instant en lui place de Madame Lienemann qui devait le faire ces amendements visent effectivement également à nous pousser est un tout petit peu plus audacieux en matière de partage du pouvoir dans la gouvernance d'entreprise, de co-détermination et de participation de des salariés à la gouvernance des entreprises, je je crois en effet que c'est une question qui, aujourd'hui, pour les salariés et centrale, qui leur permet, lorsqu'ils siègent dans les instances de gouvernance d'entreprise, d'avoir accès à des aux informations stratégiques qui sont souvent un peu éludées dans l'écurie, la consultation des comités d'entreprise et qui leur permet aussi de d'équilibrer face à la place qui est accordée aux actionnaires qui est trop souvent une place déterminée par les intérêts financiers à court terme des actionnaires, des intérêts financiers à court terme d'actionnaires ne sont pas qu'on l'cohérent avec les intérêts de l'entreprise et des intérêts à moyen terme, c'est pour ça que cette série d'amendements visent les uns et les autres à renforcer la place des salariés en n'abaissant les seuils de présence des représentants dans les entreprises de plus de 500 en permettant, en en en empêchant aux entre les entreprises en retirant aux entreprises la possibilité de déroger à l'obligation d'avoir des représentants dans les conseils, administrations

qui propose d'abaisser à 500 le seuil à partir duquel la présence, administrateur salarié est requise, seuil dans les sociétés filiales dont le siège est fixé tentait tant nationale que dans le siège social est à l'étranger, voilà donc une série d'amendements qui ont toutes pour but puisqu'il s'agit de moderniser les relations du travail, les entreprises et la gouvernance de renforcer la place des salariés dans cet organisme dans ces Merci, cher collègue, l'amendement 39 en discussion commune Monsieur Guey. Merci Monsieur le Président Madame la Mini, j'ai bien entendu votre votre réponse, bon je vois que le modèle allemand, c'est quand ça vous arrange quand il y il suffit de donner des nouveaux pouvoirs de décision dans les salariés, là, il faut attendre. Bon donc toujours sur cet amendement de 39 dans l'objectif de renforcer la présence des salariés dans les conseils d'indices rations des entreprises, nous proposons avec cette amendement de repli d'assurer une représentation minimum de 2 administrations administrateurs salariés dans les conseils d'administration, à l'exception des conseils, composée de 3 membres, cette disposition avait été adopté en séance publique le 26 mai 2016 lors de l'examen de la proposition de loi visant à encadrer les rémunérations sur proposition du groupe GDR à l'Assemblée nationale, je suis persuadé que son modèle de coups, détermination et lever des facteurs expliquant la réussite et la compétitivité de l'Allemagne, démocratiser l'entreprise, c'est donc aussi faire participer les salariés à la prise de décision en améliorant leur représentation dans les instances de gouvernance nous formions clairement un 1er pas dans la bonne direction, nous vous proposons par cohérence d'adopter à nouveau cette mesure en votant cet amendement qui permettra d'améliorer la représentation des salariés dans les conseils des grandes entreprises, je vous remercie. Merci, cher collègue, monsieur le rapporteur de l'avis de la commission sur ces 5 amendements. Donc, Monsieur le Président pour les les amendements 100, 200, 300, 400 5 ces amendements donc prône un renforcement très marquée des obligations en matière de représentation des salariés dans les conseils rations des entreprises, il convient ici de rappeler que la dernière réforme en la matière, a eu lieu en 2015, à l'initiative de la ministre, qui avant de rejoindre le gouvernement occupé d'éminentes fonctions au sein du groupe de signataires du présent amendement, il s'agit de François Rebsamen. Il avait déjà divisé par 5 de 5000 à 1000 salariés le seuil d'effectif à partir duquel entreprise et soumises à cette obligation et corriger plusieurs insuffisances de ce mécanisme de représentation, introduit en 2013 toutefois, il avait très judicieusement laissé aux entreprises concernées un délai raisonnable pour s'adapter à une telle évolution de leur gouvernance, jusqu'au terme du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice 2017, soit potentiellement jusque mi-2018 pour procéder lors d'une assemblée générale modifications statutaires nécessaires pour résumer, elles n'ont sans doute pas toutes encore recueilli des représentants des salariés dans leur conseil d'administration, D'aller bien plus loin en touchant des entreprises de taille moyenne à gouvernance familiale sans période transitoire ni même évaluation de l'impact, ou du nombre des entreprises concernées, par ailleurs, vous proposez cherche Madame Rossignol par ailleurs vous proposer la mise en place du jour au lendemain de la co-détermination de à l'allemande, dans toutes les grandes entreprises françaises, si les résultats du modèle allemand sont enviables à plus d'un titre, ils ne sont pas uniquement due aux règles de gouvernance d'entreprise, qui n'est pas possible de reproduire telle quelle dans un cadre historique, social, économique bien différent dès lors en l'absence de l'évaluation et même de mises en Oeuvres des réformes précédentes, il n'est pas de bonne politique n'est pas bonne politique de remettre l'ouvrage sur le métier, sans aucune concertation, c'est donc un avis défavorable de la commission sur les amendements 100, 200, 300, 400 5 mais un avis défavorable également sur l'amendement 39. Merci, monsieur le rapporteur, Madame la ministre. voilà comment nous abordons le sujet donc je reviens pas dessus et vous comprendrez donc mon avis est défavorable sur les amendements 100, 200, 300, 400 5 à 39 logiquement avec ce que je dis avant. Je voudrais juste revenir sur un point que je ne peux pas laisser dire, il n'est pas vrai que tous les actionnaires une vision court terme et je pense notamment dans le cas des entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, que vous voulez, visée par le dernier amendement, celles de plus de 500 salariés il y a une majorité d'entreprises patrimoniales familiale qui justement sont dans une logique de long terme, donc ça n'est en tout cas ça ne peut pas être l'argument ça veut pas dire qu'il y a pas des choses à faire dans le dialogue social ou dans le sujet, gouvernance, on pourra toujours une. Discuter le futur c'est prématuré, mais maintenant, mais on pourra toujours l'aborder, je crois que ça serait un mauvais message et incompréhensible de leur part de leur dire que c'est parce qu'elles sont une obsession court terme je pense qu'une des forces d'ailleurs de l'Allemagne, l'Italie, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises patrimoniales familiale qui résonne long terme et qui sont souvent de petites et moyennes entreprises ou de grandes, mais c'était un des sujets que traiteront aussi la mission de Nicole Notat et John Nixon se renforcer toutes les entreprises et la gouvernance dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont une vision long terme. Merci madame la ministre, oui madame au Signol précipitations de vote. Nous voterons notamment Madame la Ministre, ne faites pas semblant de ne pas avoir compris ce que j'évoquais tout à l'heure Cicor je ce que je parle des actionnaires qui ont une vision qui est une vision à court terme des entreprises, bien entendu, je ne parle pas des entreprises de caractère familial dans lequel il y a une un total homogénéité entre l'entreprise et l'actionnariat permettez-moi de dire que, une des plus une des spécificités du capitalisme financiarisé c'est que justement, les entreprises et leurs intérêts sont déterminés par des groupes d'actionnaires qui sont parfois le feu dans le classique, exemple des fonds de pension qui peut-être un peu trop utilisé, mais qui est quand même une réalité, et dans ces entreprises-là, effectivement, les actionnaires n'ont pas la préoccupation, ni de l'entreprise, ni même de la marque du savoir-faire ni des salariés, donc voilà ce que je voulais dire, je pense que vous le saviez bien. Merci, cher collègue, oui Monsieur Bonnet Arenberg pour explication de vote. Merci, moi je trouve assez cocasse, que ce soit le parti communiste qui propose la co-gestion, j'avoue que j'ai quelques réminiscences historiques et ça n'a pas toujours été le cas pour notre part dans notre groupe et dans le parti auquel j'appartiens depuis toujours, nous avons toujours souhaité effectivement que puisse prospérer dans notre pays, cette belle idée de cogestion et de co-détermination, comme on le dit Mike Beastie Mondial allemand. Problème, c'est qu'effectivement les idées n'étaient pas prêtes, que ce soit d'ailleurs parmi les syndicats que ici aussi dans nos assemblées, je me réjouis pour ma part que, effectivement, nous ayons pu voter, monsieur le rapporteur, l'a rappelé la loi Rebsamen qui a permis d'ouvrir largement puisqu'on est descendu au Seuil 2000 salariés cette possibilité, alors laissons un peu prospérer ça Tider je me je je je rejoins madame la ministre sur ce point, je crois simplement qu'il faut, je dirai, faire la publicité nécessaire pour qu'elle puisse prospérer et je souhaite que le gouvernement et vous-même, Madame la Ministre, puisse faire état effectivement des premiers résultats, notamment le succès que cette idée puisse rencontrer pour rencontrer dans les années qui viennent auprès des entreprises, on pourrait se donner peut-être un certain délai le bilan de cette, de cette idée qui me paraît non seulement généreuse mais là je suis d'accord avec vous aussi

Oui, je trouve que la la la chute de notre collègue était meilleure que l'attaque parce que, effectivement, finalement, il finit en disant : ah mais je suis d'accord avec Philippe ce que ce voilà, je le souligne, pourquoi je le souligne, parce que nous sommes en 2018 et je pense qu'il faut juger et notre collègue Vanlerenberghe normalement et bien placé, parce qu'il est membre de la commission des affaires sociales, donc il nous entend, mon collègue Dominique Vatrin et moi-même à être toujours soucieux à la fois un système qui ne nous va pas qui est le système capitaliste, je le redis, et en même temps d'essayer de construire des propositions alternatives, donc il est attentif à nos propositions et c'est un petit peu disons cavalier que d'attaquer en disant : le le Parti communiste n'a pas toujours défendu ce genre de position. Ben non, on n'a pas toujours été parfaits maintenant au lait et on voulait que ça soit dit dans les mises et donc montrer que finalement nous cheminons ex-hé bien puisque vous l'avez noté enfin de votre intervention, donc c'était un petit clin d'oeil pour continuer dans de bonnes conditions de débats. Merci, cher collègue, donc je vais mettre aux voix les amendements alors d'abord, l'amendement 102 collèges amendements ont reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement donc l'amendement 102 qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté même vote pour le 103 même vote pour le CIV même vote pour le sang

Oui, merci Monsieur le Perez, président, l'article 4 bis prévoit que les accords et conventions publiés sur la base de données publiques ne divulgue pas l'identité des négociateurs et signataires et signataires nous partageons cette volonté de rendre anonymes, ces accords accessible à toutes et tous, je crois que c'est une façon de les protéger ceux-là nous sommes d'autant plus important à un moment où nous l'avons dit à plusieurs reprises dans cet hémicycle, quelle que soit d'ailleurs les bancs être syndicaliste cela expose à des conditions parfois difficiles dans au au niveau du travail comme dans l'exercice du mandat et j'en profite donc pour insister sur le un sujet que l'article et fleurs, c'est la répression des syndicalistes dans les entreprises ce que d'ailleurs, mon collègue Fabien Gay a souligné l'avis du CESE de juillet du repéré prévenir et lutter contre les discriminations syndicales, on a démontré les conséquences, tout comme l'enquête Relations professionnelles et négociations d'entreprise, produite par la d'arrêt sont 2011, qui met en évidence que les délégués syndicaux subissent une pénalité salariale de 10 malgré la protection dont bénéficient les syndicalistes avec l'obligation de l'autorisation préalable de l'inspection du travail concernant toute demande de licenciement ou de transfert de contrat de travail, de la part de l'employeur, il demeure victime de pression d'un certain nombre de dirigeants d'entreprises, on ne peut à la fois affirmé regretter la faiblesse du syndicalisme en France et refusé d'affronter cette question des discriminations syndicales qui décourage la syndicalisation il faut le rappeler ici le principal frein à l'engagement, c'est bien la peur de perdre son emploi, la crainte des représailles et des effets négatifs sur la carrière derrière les cas de discrimination, ce sont des femmes et des hommes, des carrières brisées trop souvent hélas des drames humains, avec des effets sur la santé, sur la famille et pourquoi je ré-insiste à ce moment-là de notre débat, c'est parce que vraiment nous souhaitons avec beaucoup de gravité et de sérieux, que le gouvernement s'appuie à minima sur les préconisations de l'avis du CESE pour faire progresser le droit en matière de lutte contre les discriminations syndicales en attendant et c'est aussi très important que nous puissions souligner dans cet hémicycle, nous allons voter cet article 4 bis qui nous semble aller dans le bon sens. Et merci Madame Cohen donc l'amendement 11 rectifier bis Madame Imbert. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le président, monsieur le rapporteur, dans le cadre de la loi du 8 août 2016, le législateur a prévu la publication de tous les accords collectifs, or la sensibilité des données économiques et sociales contenues dans les accords d'intéressement de participation, les plans d'épargne entreprise inter-interentreprises ou pour la retraite collectif ainsi que les accords collectifs déterminant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou les accords de performance sociale économique s'oppose de fait à leur publication intégrale, notamment au titre de la protection du secret commercial, de ce fait, l'obligation de publication conduit les partis à mettre en oeuvre la faculté d'occultation de telle façon que la publication ne présente plus d'intérêt. à ce titre, il apparaît souhaitable d'exclus c'est texte pour concentrer l'obligation de publication sur des textes qui présente un intérêt pour la transparence de la vie économique et du dialogue social, enfin il paraît souhaitable de donner la faculté à l'employeur d'occulter des partis qui porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. Monsieur le Président, je voudrais rebondir sur 2 choses. Vous avez rappelé même quand même de le sujet de la l'anonymat des signatures de de désigner. C'est ça veut dire qu'il va effectivement dans le cadre, mais ce n'est pas la seule mesure nous avons retenu du rapport du CESE contre la lutte contre discrimination, je rappelle les fameux observatoires départementaux, je regrette beaucoup que vous ayez supprimé. Mais oui, je suis un peu têtu sur ce sujet, je sais mais. Sur le sujet, vous évoquiez Madame oui, c'est important que cette transparence qui a pour but de Crépy Tony émulation entre entreprises ne soient pas à la fin, pénalisante dans un système concurrentiel parce que on y introduit forcément lorsqu'on parle du PSE, ou de l'intéressement partie passion de certains accords des données stratégiques et confidentielles qui sont partagés avec les partenaires sociaux mais que ne pas vocation et partager avec la concurrence certains, je suis favorable, enfin le la : le gouvernement est favorable à cet amendement qui exclut les accords de paix, ce départ salariale où il y a beaucoup donné stratégique et confidentielle et qui permet d'occulter certaines parties des accords lorsqu'elles sont de nature à nuire à l'entreprise et donc, in fine, et à l'employeur et aux salariés.

En tout cas qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté, après l'article 4 bis seul amendement 56, c'est monsieur Bush Oui, merci Monsieur le Président, Madame le ministère collègues nous proposons ici avec cet amendement, de mieux encadrer les conditions de recours au travail intérimaire alors que le travail intérimaire a connu une progression de 12 pourcent en septembre dernier, la progression de l'intérim a atteint 9,2 pourcent en octobre 2017 pour le trente-cinquième mois consécutif, le développement de l'intérim concerne les transports et la logistique, mais également les services aussi, cet amendement vise-t-il à encadrer le recours un peu trop systématique aux contrats de travail intérimaire rappelons également à ce stade, que l'on recense 2 fois plus d'accidents de travail chez les intérimaires que chez les autres salariés des entreprises russes sont missionnés il est donc à nos yeux essentielles d'encadrer strictement le travail intérimaire afin de faire en sorte que l'utilisateur puisse faire appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une mission précise et limitée dans le temps et seulement pour remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail ou encore pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, je vous remercie. Merci l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur.

j'espère au printemps un peu plus tard, lorsque 2 lors du nouveau projet de loi pour l'instant, c'est un avis défavorable en attendant de pouvoir en discuter dans ce projet de loi. Madame la ministre. y a, il y a le droit et le contexte, la dynamique dans lequel nous sommes le droit, je rappelle que la loi prévoit que le recours au contrat permet temporaire ne peut pas avoir pour objet ou pour effet pouvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente d'entreprise, il faut faire respecter ce droit en même temps le le but des contrats travail temporaire et par définition de faire face à surcroît d'activité, l'absence d'un salarié dans des cas limités activement énumérés par le contrat par le code du travail et qui évidemment varie selon l'activité, mais aussi selon la période et le cycle de vie de l'entreprise, donc il est très difficile même impossible mais Dakota, je veux dire qu'il serait beaucoup trop élevés dans certains cas et et pas assez dans d'autres,

une réflexion et des propositions qui soient faites sur la régulation des contrats courts car, comme vous, je pense qu'aujourd'hui nous avons un recours aux contrats courts, c'est-à-dire intérim plus CDD certains certaines aux entreprises et parfois excessif dit certaines entreprises parce que on voit que, selon les secteurs d'activité au sein même de entre parfois pour des bonnes raisons parfois pour de bonnes, il peut y avoir des variations extrêmes et ça de conséquences, aujourd'hui nous avons 1500 85 pourcent de contrat endurer à déterminer dans les 19 millions de salariés du secteur privé, c'est assez stable, la proportion, mais comme vous le savez l'Euro le le nombre d'embauches le flux entrants est flux entrants et sortants, puisqu'il y a une majorité de propositions d'emplois qui sont faites en CDD, en intérim, il faut profiter je dirais de contexte de croissance dans lequel nous sommes sur le quai, les perspectives du coût d'emploi solide et plus robuste sont plus grandes pour avoir des mécanismes qui peuvent être, soit incitatif au contraire correctif des entreprises pour là où c'est possible, là où ça fait du sens, ne pas aller vers un excès, j'allais dire de contrats courts ça aussi une conséquence sur le coût de l'assurance chômage, parce que ces contrats courts pèse pour plus de la moitié dans le coût de l'assurance chômage, donc c'est pour ça que nous a j'ai mis la balle, si j'ose, si je dois dire dans la, dans le camp des partenaires sociaux qui doivent revenir courant février que des propositions

simplement lui dire que ce qu'on constate sur le terrain n'est pas exactement ce qu'elle nous dit : je pense que le le phénomène de l'intérim est quelque chose qui est développée de manière exagérée et il suffit d'aller dans les entreprises de production, je suis allé sur la zone KP piqûres dans mon département, Boulogne-sur-Mer, on peut aller dans des entreprises automobiles, on voit que que manière. Permanente, il y a 40 pourcent voire plus de contrats d'intérim dans ces entreprises et compris le système est d'autant plus facile à identifier comme étant organisée que les structures d'intérim les boîtes d'intérim sont présentes dans l'entreprise même pour organiser ce roulement au détriment des salariés, alors bien sûr, il y a eu des choses de tenter dans les lois précédentes, on a instauré le CD or ce que l'on entend pour ceux qui en sont concernés : le retour d'expérience et que ça n'a pas réglé leurs problèmes d'insertion dans la société, car lorsqu'il s'vont dans une banque lorsqu'ils vont chercher à logement leur dit que sur leur contrat, il y a le mot intérim donc je crois que c'est une virée question il faut véritablement que dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, des réponses soient apportées, nous en faisions une et nous reviendront probablement sur celle-ci, ou sur d'autres, en fonction du déroulement des négociations. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, bon, c'est un sujet important, je voudrais simplement appel attention sur le fait que ce sujet va être évoquée très bientôt le fait qu'il ne faut pas mettre restriction au recours aux contrats et qu'on va au travail intérimaire de manière générale, surtout lorsqu'on évoque des contraintes pour des entreprises dès lors qu'il y a on salariés limitant à 10 le projet de recourir au travail intérimaire ça apporte des contraintes absolument terribles sur les petites entreprises et je voudrais rappeler ici les difficultés que nous rappelle un certain nombre de chefs d'entreprise, de trouver les collaborateurs dont ils ont effectivement besoin, elles ont de plus en plus de difficultés, je vois dans le secteur de dans la Bretagne par exemple, le secteur de la construction navale qui a des difficultés à pouvoir prendre des commandes, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la main Oeuvres dont ils ont besoin, au travail intérimaire permet d'une part de pouvoir assurer la livraison d'un certain nombre de commandes de fournitures de marché et puis permet aussi d'identifier des collaborateurs qui a ainsi peuvent rester recrutés par les entreprises, parce qu'ils ont ensuite démontré qu'ils ont les qualités répondant aux besoins des entreprises, donc il faut être très intense, très attentif au fait de ne pas mettre de contraintes trop draconiennes qui ferait que cela aurait un effet contraire à celui recherché, c'est-à-dire qu'il y a un bon nombre de nos compatriotes qui puissent retrouver un emploi.

Alors cet amendement relève le seuil de déclenchement des nouvelles obligations des entreprises, notamment en matière des attributions du Conseil social, économique, le CSE de 50 à 75 salariés en effet les franchissements de seuil entraîne de nombreuses, de nombreuses obligations supplémentaires pesant lourdement sur la vie économique et professionnelle de l'entreprise, cette situation conduit de nombreux chefs d'entreprise à limiter la croissance de leur entreprise pour rester sous ce seuil, d'autres d'ailleurs de boulot pour d'autres sociétés à côté pour pas dépasser ce seuil, en fait, c'est autre chose : ainsi, la France compte 2,4 fois plus d'entreprises de 49 salariés que d'entreprises 2 51 salariés le dépassement de ce seuil à 75 salariés est une mesure favorable à la création d'emplois, c'est l'objet de cet amendement. d'abord rappeler que la mise en place du CSE dans toutes les entreprises employant plus de 11 salariés atténuera probablement la rigueur du passage du seuil de 50 salariés je rappelle aussi que ce passage déclenche de très nombreuses obligations qui ne sont pas elles directement au droit du travail, ce sont des plus obligation en matière environnementale, en matière fiscale et en matière sociale, donc pour l'instant, c'est un avis défavorable. Madame Amir. Oui, le l'ordonnance qui fusionne donc les 3 instances d'information consultation pour en faire le côté social, économique va déjà avoir un effet assez fort sur le seuil de 50 c'était encore plus sensible dans les entreprises de 50 ou 60 salariés une rencontre beaucoup ont fait pour le coup, c'était les mêmes personnes qui siégeait en plus et du comprenez ça a amené de surtout une complexité énorme qui est celle-là est levée par la fusion alors après le seuil de 50 salariés il amène des devoirs, il amène aussi des droits et je pense notamment au droit bénéficier aux activités sociales et culturelles qui soit très populaire en France et supprimer ce droit pour les salariés de plus de 50 salariés, dire qu'il faut quand même y réfléchir à 2 fois, parce que c'est, même si ce sont des sommes modestes dans une petite entreprise, ce quelque chose qui est très apprécié, vous posez une question qui est plus vaste que ce sujet de la représentation que la question des seuils en général et comme j'ai eu l'occasion de le dire hier la question D'où ce matin vous enfin bon bref. Comme le provoque le gazon de dire quelqu'un en a parlé, la question des seuils sociaux, fiscaux et la multiplicité des seuils. Qui rend le paysage très compliquée et la question des effets des seuils, est une question qui, sans engagement, mais en tout cas fait partie des choses qui seront étudiées dans le cas de la loi pacte portera vos collègues Bruno Le Maire, donc vous, vous aurez l'occasion probablement au printemps aussi d'y revenir. Donc je mets je vois l'amendement 3 rectifier de quater avec 2 avis défavorables de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté l'amendement 156 du gouvernement, Madame la Ministre. monsieur le président, il s'agit de prendre acte des dispositions de l'article 13 de la loi organique organique même 17 13 38 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, en effet, cette loi organique impose le recours à la loi au nom de la séparation des pouvoirs pour dessiner un député ou un sénateur dans les organismes extraparlementaire et aujourd'hui, nous n'avons pas cette base légale pour le conseil d'orientation de la participation de l'intéressement d'épargne salariale et l'actionnariat salarié, le copier alors le est important et nous allons le saisir, je vais le saisir d'ailleurs très rapidement dans les tout prochains jours sur la réforme de l'intéressement, de la partie passion d'épargne salariale, le Sénat et sera d'ailleurs éminemment représentés madame la sénatrice Pascale Gruny et monsieur le sénateur Jean-Louis Touraine qui vont donc au nom du Sénat alimenter ses travaux et ces travaux ont vocation, ils sont véreux menée avec les partenaires sociaux, elles sont menées à la fois par mon ministère et celui de Bercy continue des impacts sociaux, fiscaux et le but de cette réforme et de réfléchir à comment étendre progressivement le bénéfice de l'intéressement des partis passion à tous les salariés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et aussi Carifiesta amplifier le sens de la formule de participation qui aujourd'hui n'est pas lisible pour les salariés, donc ne fait pas oeuvre pédagogique parce que ça permet pas de mesurer quel est l'impact de l'action des salariés sur le résultat de la partie passion tellement la formule est complexe, ce qu'il s'agit donc d'améliorer la transparence là dessus, il peut y avoir d'autres objets, mais en tout cas le je vais saisir Kapisa c'est donc les nouveaux sénateurs dès que la loi a voter très rapidement parce que nous aurons un travail important dans les mois qui viennent, sur ce sujet. Madame la ministre, l'avis de la commission. La commission a émis un avis favorable à l'amendement va dire aussi que la désignation de Pascal poignée Monsieur Touraine, constituer un binôme percutant.

Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté. Nous passons à l'examen de l'article 5 avec 3 demandes de parole monsieur Vatrin. L'ordonnance visé par cet article 5 intègre un dispositif qui commence à faire parler de lui, celui de la rupture conventionnelle collective, le fait que des entreprises aussi diverses que PSA Pim qui Monoprix et d'autres encore, annonce le recours à cette procédure, indique cet outil particulier de gestion des effectifs risquent de devenir un outil de gestion ordinaire des entreprises ce qui n'est pas sans conséquence, loin s'en faut, car il faut tout de même revenir sur l'aspect le plus essentiel de ce dispositif à la savoir ça son déclenchement sans justification économique avéré, c'est-à-dire une procédure de suppression collectif d'emploi sans difficultés économiques approuvé ainsi une entreprise pouvant présenter une situation financière florissante pourra proposer un accord de ruptures conventionnelles collectives aux organisations syndicales représentatives de la même manière qu'une entreprise qui rencontreraient quelques difficultés, donc il nous semble que cette disposition pose une question plus large sur le sens même qui doit ici nous sommes que la loi n'est plus l'expression de l'intérêt général, mais un outil de mise en jeu d'un intérêt particulier, celui de l'entreprise, singulièrement du point de vue de sa rentabilité financière et de la rémunération des actionnaires, quoi qu'il serait bien, dit réfléchir tout de même, au moment même où de grands de grands groupes et non les moindres annoncent des réductions massives d'emplois, sans susciter, il faut bien le dire, beaucoup de réactions de la part du gouvernement, ne faisons pas le procès ici de toutes les entreprises ne faisons bien la difficile distinction entre les petites entreprises et ces grands groupes qui manifestent et nous sommes une certaine irresponsabilité sociale dans le contexte de notre pays, qu'il y a déjà 6 millions de demandeurs d'emploi, hé bien peut-être me rétorque vous que la rupture conventionnelle n'est pas vraiment quelque chose de nouveau par rapport à ce qui a pu exister auparavant les plans FNE des années 80 par exemple, mais il y a quand même 2 différences fondamentales : la 1ère c'est qu'il y a pas de motivations économiques apportés, la 2ème, c'est que la location et les garanties des salariés sont plus faibles, nous nous opposons à ce nouveau dispositif. Oui, merci Monsieur le Président, avec la rupture conventionnelle collective il s'il s'agit d'éviter le traumatisme de licenciement mais comme la débauche la démontrer mon collègue Dominique Vatrin, c'est au contraire un appel d'air pour licencier plus facilement en limitant soi-disant les risques de conflits sociaux depuis la publication du décret, le 27 décembre dernier PSA Ping qui Le Figaro les Inroc ou encore la Société Générale, ont annoncé les premières RCC chez PSA où 1300 postes doivent être supprimés, la direction a décidé d'augmenter les primes de départ pour les salariés franciliens, ce qui laisse présager une possible fermeture de l'usine de Saint-Ouen : J'ai Pink pas signature mais suppression de 208 postes pour les autres entreprises que j'ai cité, ça n'est pas encore effectif le gouvernement met entre les mains du patronat, on le voit bien un outil qui permet de procéder à des ruptures conventionnelles collectives de contrat de travail, nettement plus facilement que dans le cas du plan de sauvegarde de l'emploi, donc on se retrouve en quelque sorte devant un faux choix entre un plan de de départs volontaires ou bien une fermeture d'entreprise, alors vous nous dites qu'il y aurait un garde un garde-fou le contrôle BRC par la Direct qui est censé vérifier la conformité dans les 15 jours et donner son avis, c'est cet avis qui validera la rupture conventionnelle collective ne laissant plus de possibilités pour les syndicalistes d'attaquer ensuite ces ruptures conventionnelles collectives devant le juge 15 jours pour donner son avis, alors que l'émission de la Directs ont été depuis 2016 sans cesse accrue, alors que les leurs effectifs sont réduits dans le même temps, comment voulez-vous que les agents puissent véritablement contrôler la conformité d'une RCC en 15 jours, comment peut-on penser sauver l'emploi en facilitant les licenciements de manière massive, si ce n'était pas aussi dramatique, on pourrait parler de fable grotesque, j'attire votre attention, mes chers collègues, les entreprises que j'ai nommé ont annoncé dès RCC. Alors que notre haute assemblée n'a pas encore voté cette ordonnance, on voit bien ce que ça pourra donner Kant ou si nous votons cette ordonnance, c'est pourquoi nous vous demandons la suppression de cet article par notre amendement. Merci Monsieur Touraine le sens ici identique. Oui, c'est le même objet. En résumé, l'ordonnance comporte des dispositions telles que la barémisation des indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la restriction territoire national du périmètre d'appréciation des licenciements économiques, la création de la rupture conventionnelle collective permettant l'évitement du plan social et des obligations de reclassement, la généralisation du contrat de chantier CDI comme contrat à durée imprévisible pour ne parler que du plus visible c'est article est donc un élément central de la réforme du droit du travail dans le sens de la précarisation du salariat par la forme des contrats de travail et les modalités de rupture des contrats le prétexte en est que plus les contrats seront précaires plus les employeurs pourront facilement licencier et plus ils embaucheront. Votre postulat est démentie par le réel depuis plusieurs décennies à bas bruit et plus et puis plus clairement, la précarisation, se répand et le chômage ne diminue pas, s'agissant de la rupture du contrat, le patronat veut à tout prix éviter la judiciarisation à tout prix mais pas à n'importe quel coût, il est certain que la suppression de la prime de préparer de précarité afférentes aux CDD grâce au contrat de chantier pourrait représenter une affaire intéressante, il suffira d'embaucher à chaque nouveau projet de débouchés, sans formalités inutiles, le sommet est atteint avec la barémisation des dommages intérêts en cas de licenciement abusif dommage préjudice vous nous demandez de valider un déni de droit, le préjudice sera réévalué au bénéfice de l'employeur, le pouvoir du juge est réduit, surtout le principe de droit selon lequel le préjudice doit être évaluée et indemniser individuellement et totalement est liquidée en quoi tout ceci va-t-il permette le développement de l'emploi, c'est vraiment prendre prétexte de la situation actuelle pour transformer au profit exclusif des employeurs, la relation et le droit du travail. la 3ème ordonnance donc permet principalement de simplifier et de moderniser les règles du droit du travail en matière de licenciement le barème comprend de nombreuses exceptions et permettra aux juges à l'intérieur des planchers et plafonds fixés par la loi d'individualiser le montant de l'indemnité allouée un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, la définition d'un périmètre national pour apprécier les causes d'un licenciement économique met fin à une exception française en Europe, qui étaient guère justifiée d'un point de vue économique et qui nuisait à l'attractivité de notre pays, je rappelle que la rupture conventionnelle collective instaurée par cette ordonnance ne peut être utilisé que s'il y a double accord tout d'abord un accord collectif, puis un accord individuel des salariés concernés qui doivent se porter candidat auprès de l'employeur pour en bénéficier, j'ajoute que la RCC doit ensuite être validé par la directe par conséquent pour toutes ces raisons, la commission sur l'amendement 41 amendements 106 a émis un avis défavorable. Merci madame la ministre. Monsieur le président, bien évidemment, gouvernement, un avis défavorable, ça paraît évident, je vais pas revenir sur tous les points qu'a évoqué monsieur le rapporteur, un moment sur ce qu'est la rupture conventionnelle collective comme c'était un élément nouveau jeu- là aussi je souhaite être sûrs que nous avons nous ayant tous la même compréhension de quoi il s'agit, la rupture conventionnelle collective qui dont le nom et l'esprit s'appuie sur l'expérience de la rupture conventionnelle individuelle, c'est-à-dire un accord des parties n'est pas le la solution pour toutes la situation du tout. Il y a des situations notamment lorsqu'il y a pas eu anticipation pas préparation ou que le dialogue social ne permet pas aux couleurs entreprise a le dos au mur, où malheureusement on ne les entreprises, objet de recours à de recourir à un PSE avec ou pas une partie de départs volontaires, je rappelle que le PS après information consultation une décision unilatérale de l'employeur, compte tenu de difficultés économiques, là on est dans le cas de la rupture conventionnelle collective, on est dans un contexte à plusieurs égards différent : il s'agit de contexte où il y a anticipation accompagnement d'évolution de réorganisation qui va être passe dire forcément une restructuration dramatique, au contraire, le but, c'est plutôt d'être dans un contexte où on ne va pas, pas y avoir de licenciement, il y aura pas la brutalité juré du licenciement économique, en revanche, un accord des parties et trouvé pour pouvoir anticiper ou accompagner les évolutions, les réorganisations nécessaires en fonction des marchés des métiers de l'entreprise, concrètement, il y a 3 conditions, qu'ils sont qui qui sont cumulatives la 1ère condition c'est qu'il faut-il qu'il y a un accord majoritaire entre les syndicats de salariés et l'employeur, je rappelle que ce n'est pas nécessaire pour PS, le 2ème condition c'est qu'il faut que les départs soient strictement volontaire alors que dans le cas de PSE on peut avoir une partie de volontariat, une partie de licenciements, la une réelle rupture collectif ne peut concerner que des départs que des départs volontaires mais par contre il y a bien des mesures d'accompagnement de reclassements de formation de mobilité qui peuvent être qui peut de prévu, contrairement à ce que la vie un peu la presse mais je pense que c'est parce que le les choses et nouvelle et qu'elle est encore mal connu. 3ème condition c'est qu'il faut Union homologation de la Direct pour vérifier que les 2 premières conditions bien été remplies, c'est-à-dire qu'il est bien d'accord majoritaire d'une part à strict au volontariat, d'autre part et j'irai, vérifier que les conditions sont bien dans lequel les salariés ont eu la formation sont bien sont bien complètes, précises et donc je dirais on est sur un terrain sur du point de vue du volontariat des salariés comme de l'accord des syndicats. Je pense que l'actualité des dernières semaines, vous l'avez évoqué à montré déjà et je pense que ça se confirmera que ce que vous ce que ce qui est prévu dans les ordonnances et robuste, c'est-à-dire que le droit correspond à l'intention pourquoi je dis ça parce que dans le cas de

Et donc il y a eu un équilibre dans cette négociation qui fait que les syndicats et salariés sont positives sur le sujet, en revanche, dans le cas de prime qui les syndicats ont refusé

moi je connais pas le cas, donc, et dans ce cas-là, c'est assez logique, ils ont refusé, donc ils ne peuvent pas faire de ruptures conventionnelles collectives, faut bien comprendre que ce n'est pas un acte unilatéral, c'est bien avec un acte de négociations qui s'inscrit dans la logique du dialogue social et économique dont on parle en permanence pour les ordonnances qui ne couvrira pas tous les cas qui permettra, plutôt, les sujets d'anticipation, d'accompagnement et je dirais qui permettra d'éviter que un certain nombre de décisions n'étant pas prise ultérieurement, il y a des choses par compte beaucoup plus brutal et beaucoup plus pénalisante, qui se passe parce que l'entreprise est oui hé ben un plan social, ça restera toujours un traumatisme est toujours de fait brutale même bien accompagné, ça reste quelque chose qui est difficile à vivre dans l'entreprise. Donc je crois qu'il faut pas

qui va prendre en compte les réalités d'entreprises et les aspirations des salariés, je crois que, évidemment, ça fera partie dans l'évaluation des ordonnances, on suivra de très près, cet objet nouveau c'est juste dire et nous en rendre compte au Parlement. Merci donc c'est un avis défavorable Monsieur Touraine pour explications de vote. Oui, madame la ministre, votre discours est séduisant et il correspond d'ailleurs au contenu du des ordonnances parfaitement conforme et je ne contesterai pas ce que vous avez dit juste préciser, j'ai rencontré la semaine dernière, la directrice de PSA sur le site de Rennes. Ou sont en train de se mettre en oeuvre les conventions, les ruptures et son raisonnement est le même que le vote, c'est-à-dire qu'elle nous laisse entendre que c'est du volontariat, que les syndicats doivent être d'accord, bref qu'il y a une préparation. Cependant je je voudrais que. que. Soit vous m'ôtez une angoisse. Soit vous essayez de voir quelles sont les perspectives possible qu'est-ce qui se passe en réalité. PSA à Rennes, en tout cas, met en place une nouvelle chaîne qui va fonctionner complètement différent différemment de la chaîne actuelle et suppose des compétences des connaissances et une formation particulière et pour un certain nombre des salariés de PSA considère que cette formation va être trop difficile compte tenu du niveau compte tenu de l'âge des salariés et plutôt que de d'engager ses procédures de formation, il préfère proposer à ses salariés de de s'en aller avec une prime, avec un certain nombre d'accompagnement, ce que vous avez évoqué tout à l'heure et en même et recruter un certain nombre de salariés qui auront des capacités à appréhender le métier beaucoup plus vite que les autres, donc on on a une espèce de remplacement progressif par des salariés de des salariés âgés par des salariés plus jeunes, et ça risque de cet homme, parce que c'est vrai que le modèle peut intéresser des chefs d'entreprise alors que c'est tout de même du chômage qui attend ceux qui vont partir, même s'ils sont d'accord, il y a tout de même cet aspect de gens à qui on propose de s'en aller, de perte de de l'estime de soi, le sentiment qu'on n'a pas été à la hauteur, moderne, il y a un espèce oui je crois qu'il y a un aspect très pervers dans cette affaire. Merci monsieur Bourquin pour explications de vote.

les bénéfices de PSA sont au beau fixe. Après quelques années où il y a, où il y avait un risque de dissolution de cette entreprise avec l'intervention du gouvernement précédent, nous avons sauver cette entreprise et aujourd'hui avec la 3008, car 308 hé bien cette entreprise connaît vraiment une situation tout à fait florissant et c'est à ce moment-là que l'on met en place la rupture conventionnelle collective, il faut le dire, c'est un peu ce allégé. Appelons les choses par leur nom, madame la Ministre, avant quand il avait des Z'suppressions d'emplois, c'est quand il y avait pas de travail pique la entreprise connaissait des difficultés maintenant même comme ça va bien, on lit ou on se sépare de de personnel 10 ce nouveau dispositif va clairement intervenir dans la gestion systématique des emplois et des formations, des grandes entreprises et il faudra certes un accord majoritaire, comme vient de le dire, la ministre, il sera ensuite impossible. Tant pour les salariés des syndicats qui ont signé de remettre en cause. Aucune obligation de reclassements. Aucune action de formation ou de maintien de l'emploi, un chèque suffira, même si celui-ci peut-être intéressant et cette mesure qui n'était pas collective existait auparavant, combien de personnes qui ont signé une rupture conventionnelle collective. Sont à la charge des CCAS, par la suite. Parce que il ne retrouve pas de travail, voilà, mais ce qui est le plus grave dans cette affaire, Madame la Ministre. C'est que c'est la discrimination par l'âge.

des questions qui méritent d'être discutés, c'est encore à nouveau recul social collègues c'est encore un nouveau recul social. Monsieur lévriers pour explications de vote. de vote. Rapide et en quelques mots, je je crois au dialogue social, je crois aux chefs d'entreprise et aux syndicats, et je m'étonne après tous les discours que j'ai entendu tout à l'heure sur la méfiance que vous avez ce chef d'entreprise aujourd'hui, c'est sur les syndicats, vous avez des méfiance, il y a des accords qui sont signés entre différentes parties faites leur confiance et donc, bien évidemment, je voterai compte. Merci, cher collègue alors sur les l'amendement 40 mais aussi sur l'amendement 106 puisqu'il est identique, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le CRC. Je vous rappelle que l'avis de la commission a défavorable à vie du gouvernement est défavorable, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par article 56 du règlement, le scrutin sera ouvert dans quelques instants.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos, j'ai été secrétaire à procéder au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du scrutin numéro 54 sur les amendements 40 et 106 identique tenue de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs groupes politique et notifié la présidence le nombres de beau temps. Nombre de suffrages exprimés 344 pour l'adoption 93 contre 251 le Sénat n'a pas adopté. Je mais au bout, alors l'article, l'article 5 et donc adopté.

Qui s'abstient. Il est adopté, après l'article 5 l'amendement 107 Monsieur Touraine.

Contre l'article 5 sur cette cette proposition d'amendement, il faut rappeler que le rapport du 16 heures intitulé l'impact du chômage sur les personnes et leur entourage, de mai 2016 décrit parfaitement les conséquences plus psychologique et social du chômage quand même financière. Les atteintes à la confiance en soi, ses capacités de rebond, les sentiments d'exclusion et culpabilité sont édifiants : ils peuvent entraîner des préjudices irréversibles pour ces personnes et leur entourage, notamment familiales rester intégrées à l'entreprise permettrait d'éviter ce type de trop Marco Constant c'est la raison pour laquelle il est souhaitable d'engager une réflexion plus rapidement possible sur ce thème, sachant que les expériences étrangères existe, de quoi s'agit-il en clair. Ce qui est la malédiction qui pèse sur le chômeurs c'est moins l'indemnisation dont il va être l'objet parce qu'elle dure 2 ans, elle est pas si mauvaise que ça, ce qui pèse sur le chômeur, c'est le fait d'avoir été licencié d'avoir peur du regard des autres d'être incapables de retrouver l'estime de soi, et par conséquent de n'être plus salarié il faudrait arriver à distinguer le chômage du statut de chômeur, c'est la raison pour laquelle une réflexion est demandée pour essayer de voir si on ne pourrait pas moduler le préavis comme ça se fait dans un certain nombre de pays et notamment en Suède sur la la durée de formation nécessaire pour intégrer une autre entreprise de façon à ne jamais perdre le statut de salarié et ne jamais se retrouver dans une situation extrêmement de délicate. Oui merci Monsieur Président, on peut évidemment comprendre les motivations de notre collègue et on connaît tous les effets somatique et psychologique du chômage, ses effets sont majeures sur ceux qui en sont atteints, mais cet amendement pose moi j'accueille 2 problèmes sur la forme, il est dépourvu de valeur normative, il ne prévoit pas la remise d'un rapport et ne fixe pas de règles de droit alors je suspecte fort que parce connaît, sachant que la commission effluves défavorable, rapport au par le plus de de réflexion que de rapports pour ne pas d'avoir un avis défavorable immédiat sur le fond ensuite. Ce serait amendement étant en partie satisfaits par l'existence du congé de reclassement dans l'entreprise de plus de 1000 salariés qui permet de garder quand même un lien entre entreprises et salariés pour lequel un licenciement économique est envisagée et du contrat de sécurisation professionnelle dans les autres entreprises, que la 3ème, banque Venance à créer un congé de mobilité qui peuvent être proposée par accord collectif, indépendamment d'un projet de licenciement économique, en conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur la forme. Oui, ce président, je crois que cet amendement effectivement on pointe une question je pense. Sur lequel il y a déjà beaucoup d'outils mais qui est une vraie question. J'ai mieux prévenir que guérir et c'est vrai qu'il est, il est. Important que les discussions de reclassement, de formation commence pendant que le plus possible, pendant que le salarié est encore, soit par l'entreprise précédente, à la fois en termes de confiance en soi et en terme de sécurisation des du parcours, ceci dit, demande proposerais plutôt le retrait de cet amendement parce qu'en fait les partenaires sociaux peuvent déjà, d'ores et déjà s'entendent pour fixer une dire de une durée préavis différente de celle appliquée à par défaut et qui, mieux adapté à leur condition de rupture et par ailleurs il y a 3 dispositifs qui qui répond déjà à cette logique

c'est le contrat de sécurisation professionnelle qui a exactement cet objet qui peut être négociée dans les entreprises de plus de salariés, c'est le congé de reclassement qui a cette même logique où c'est possible aussi de tenir compte de la durée des et mesures d'accompagnement et de formation et puis dans la rupture conventionnelle collective effectivement, on peut aussi allonger la durée

peut faire cette adaptation, en fonction notamment de la formation notamment d'autres mesures d'accompagnement, ce que je pense c'est qu'aujourd'hui c'est peut-être pas utilisé à l'ampleur de ce que ça pourrait et qu'effectivement il y a un intérêt à faire de la publicité, si j'ose dire, de ses possibilités et pour les partenaires sociaux s'en saisisse oui au finalement on a, on a l'arsenal juridique, on n'a peut-être pas encore beaucoup cette pratique cette cette pratique de négociations mais je crois que c'est quelque chose dans le dialogue social qui pourrait encourager puisque il y aura plus de marche pour le faire, on a même ajouté un objet qui est la RCC. Madame la ministre, donc il y a de vendre de retrait Monsieur Touraine il est maintenu ou retiré. Et maintenu une explication de vote Monsieur Touraine.

Je voudrais tout de même précisé non c'est juste une piste, c'est pas la seule, mais je crois que ce qui est important, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de distinguer le chômage du statut de chômeur ne sont pas à l'abri d'une recrudescence du chômage c'est par vague, il suffira que la l'économie numérique aille beaucoup plus vite que nous le pensons qu'elle révèle un certain nombres de de surprise désagréable et nous aurons des des chômeurs qui vont se retrouver à pointer et je je me dis que les solutions existent, il y a 41 milliards d'euros qui sont distribués pour la formation de ces chômeurs

pas qu'il y a d'autres, statut que celui qu'ils ont, dès l'instant où vous le modifiez voulait pointer du doigt, vous faites une espèce de, de discrimination et ils sont, ils sont dans la difficulté, notamment sous le regard j'ai cité tout à l'heure, la Suède, mais l'existant en Autriche, ce qu'ils appellent les fondations qui sont tout à fait remarquable aussi pour, le temps de formation, on est encore salarié de l'entreprise puisque la fondation d'ailleurs ce l'enseignement est dispensé la plupart du temps dans les locaux de l'entreprise, voilà c'est juste cet appel à la réflexion, si vous ne voulez pas de mon amendement, je souhaite malgré tout que vous retenez l'idée qu'un jour il faudra bien qu'on on arrive à une solution comme celle-là, pour éviter tous les dégâts collatéraux qu'on peut connaître chez les chômeurs. jamais je voilà Mandement 107 qui n'est pas retiré, qui a donc un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour.

Décidément, je vous fais confiance. C'est c'est tout simple, c'est une c'est une une interpellation d'un chef d'entreprise qui dit ceci : moi j'ai fait des efforts pour former mes salariés, une fois qu'ils ont été formés, ils ont eu plus de valeur, par conséquent, ils ont intéressé d'autres entreprises, 16 autres entreprises en ont bénéficié ont bénéficié des compétences acquises, mais c'est moi qui est payé à la formation donc est-ce qu'il est possible d'imaginer un système dans lequel la formation qui a été financé par une entreprise soient prises en charge par l'entreprise qui va accueillir l'employé ainsi valorisé et largement plus compétent. Merci, monsieur le rapporteur. Oui c'est un avis défavorable de la commission, je voudrais juste rappeler à Monsieur Touraine, que le gouvernement a déposé fin avril, c'est bien fin avril un un projet de loi pour la réforme de la formation professionnelle et que c'est dans ce cadre qu'on aura évidemment l'occasion de rediscuter de tout ça, ça c'est un 1er pas, en outre, je suis surpris par la proposition d'obliger les salariés à rembourser à son ancien employeur, une partie de sa formation s'il quitte l'entreprise dans les 6 mois, cette obligation est trop générales et floues, elle s'appliquerait ici même en cas dissentiment et on ignore le niveau de la ce serait une rupture dans le modèle de formation que nous connaissons, qui pourrait avoir des effets pervers en additionnant certaines personnes évidemment ne suivent des formations, c'est qui, un jour devoir rembourser celle-ci donc un avis défavorable, avec possibilité d'en rediscuter dès le mois d'avril. Monsieur le rapporteur, Madame la ministre sur cette réflexion. C'est pas en jeu, je note qu'il y a l'innovation dans les types d'amendements puisque c'est ni un rapport ni du droit dur c'est à nouveau, c'est un appel à la réflexion, notamment du gouvernement. J'accepte l'invitation à réfléchir, mais pas d'dans le droit, parce que je crois que ce que l'incendie, un peu compliqué, ce qui va, par défaut, ça voudrait dire que tout ce qui n'est pas dans le droit, nous allons pas y réfléchir, ça ça limiterait un petit peu le Champ mais plus sérieusement. Sur le fond, donc c'est c'est un avis défavorable sur l'amendement

il y a une continuité des parcours de formation quelquefois le salarié qui tombe, une entreprise allant dans une autre, la question peut se poser, il y a une 2ème question qui est aujourd'hui la capacité de formation, on va le voir dans l'apprentissage, les capacités de formation des grandes entreprises sont supérieures à la capacité d'embauche, c'est souvent l'inverse pour les PME, donc il y a des questions de réflexion aussi avoir ce comment dans un écosystème qui pète géographique ou sectoriel certains entreprises notamment pour l'apprentissage, mais ça peut être le cas pour la formation continue, qui disposent de capacités de formation plus importantes peuvent et à quelles conditions les met à disposition d'entreprises qui voudraient embaucher des personnes qualifiées, mais qui n'ont pas forcément le besoin de former, donc voilà, je pense que ça, ça fait pas. Ces 2 sujets mais. Nous aurons une brève interruption entre les ordonnances, la loi sur l'avancement du dialogue social et la loi si vous revenus que nous aurons encore ça en mémoire quelques mois pour en discuter. avis défavorable de la Commission et du gouvernement, je mais aux voix l'amendement 108 qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adoptée, nous passons à l'article 6 2 amendements identiques le 41 c'est monsieur Vatrin. l'article VI modifie les règles issues de l'ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, le droit du travail, il faut dire, était déjà largement flexible, mais vous avez ici, je l'ai déjà évoqué dans mon intervention général vous voulez réduire le périmètre des licenciements économiques au territoire national plafonner les indemnités prud'homales en cas de licenciement illégal au motif de lever la peur d'embaucher des employeurs autoriser les prêts de main-d'oeuvre gratuit faciliter le recours aux CDD à l'intérim, alors même que vous l'avez dit, dans le même temps, vous constatez l'accroissement de l'utilisation des ces formes d'emploi et même même proposé d'élargir le nombre de secteurs, pour les contrats d'chantier ce n'est tout de même pas rien dans votre élan, vous êtes même peut-être allé trop loin, puisque l'Assemblée nationale, votre majorité revenue sur certaines mesures en introduisant des correctifs censés d'imiter les conséquences pour les salariés de cette libéralisation outrances du droit du travail, mais ce n'est pas, selon nous, en corrigeant des dérives potentielles par exemple du licenciement économique ou en aménagement les règles du barème impératifs du licenciement bien en introduisant priorité d'embauche pour les contrats d'change que vous avez véritablement améliorer des choses : limiter les conséquences ne suffit pas, alors qu'il nous sommes c'est la racine même du texte qu'il faut d'acte originel, c'est effectivement cette ordonnance numéro 2017 13 87 sur la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail quand on décode : que veut dire prévisibilité 6 n'est anticipée des sanctions, pour leur part l'employeur du juge des prud'hommes pour calculer à l'avance le montant des indemnités en cas d'essence Simon on parle ici 2 licenciements et on sécurise l'employeur, on parle de licenciements abusifs et on sécurise l'employeur, donc nous ne sommes pas d'accord avec cela et nous proposons de supprimer cet. Merci Jacques Oleg l'amendement 109 Monsieur Touraine. Oui, il est défendu, je vais pas reprendre les termes qui ont été utilisés, j'ajoute simplement la possibilité, dans cet article de conclure par tous moyens, c'est-à-dire sans garanties pour les salariés, un accord individuel de télétravail régulier, sans passer par un accord collectif, le danger c'est que on peut toujours arriver à convaincre un salarié ne serait-ce que par l'autorité qu'on exerce sur sur lui de d'accepter le télétravail, c'est moins facile dans un accord collectif, il s'agit là d'un moyen de contournement des institutions représentatives du personnel, qui veille lors de la négociation des accords collectifs à ce que l'ensemble des garanties légales en la matière soit assurée, mise à disposition des matériels locaux adaptés, droit à la déconnexion accidents du travail et présence régulière dans l'entreprise.

Merci la ville du gouvernement Madame Istres. Monsieur le président, comme vous l'imaginez, le gouvernement est défavorable à supprimer l'article 6 et l'ensemble des articles d'accord. Merci Monsieur Chassaing pas, explications de vote.

vouloir être dans cette rupture, Colette, le collectif, donc je pense que les personnes ne vont pas dire comme ça pour faire plaisir si c'est c'est parce que ils ont peut-être envie de faire autre chose en ce qui concerne le compte personnel de prévention et de pénibilité il y avait déjà des facteurs qui ont été retirées totalement ingérable, comme la pour les petites entreprises comme la manutention des manuels de charges des postures pénibles, c'était impossible d'être quantifiée, donc je, moi je pense que c'est une bonne chose, alors le compte personnel de prévention hé bien concernant les mêmes prérogatives que le C3 c'est-à-dire que il peut y avoir effectivement des des déformations, des départs anticipés à la retraite, voilà et effectivement des critères sont conservées, mais ces critères sont gérables, donc effectivement je voterai contre les amendements. Merci, cher collègue, donc sur ces 2 amendements 41 109 j'ai été saisi d'une demande ce scrutin public par le groupe CRCE je vous rappelle que la commission et le gouvernement ont émis un avis défavorable, il va procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin sera ouvert dans quelques instants.

Le scrutin est ouvert.

Plus personne n'a demandé à voter, le scrutin est clos invité secrétaire à procéder au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du scrutin numéro 55 sur les amendements 41 109 compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs ou politique et notifié à présidence 344 Votants 344 suffrages exprimés pour l'adoption 93 contre 251 le Sénat n'a pas adopté.

Ah oui, je place beaucoup d'espoirs sur celui-là pour avoir enfin un amendement qui puisse être accepté, mais ce qui est, l'expression par tout moyen et j'ai toujours du télétravail. Par le mot écrit tout moyen, laissant entendre que ça peut-être un accord arraché et qui n'aurait pas reçu de signatures, confirmant la volonté du salarié.

Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur. l'accord implique selon moi et selon la Commission, une trace écrite, qu'elle soit manuscrite ou informatique, donc l'amendement et selon la Comission satisfait les services du ministère du Travail considère que l'expression tous moyens renvoie à un accord écrit, je pense que la ministre confirmant la vie qu'on a fait et donc c'est une demande de retrait puisque l'amendement est satisfait, sinon aussi n'avait pas de retrait, ce serait un avis défavorable. C'est madame la Ministre même avis. Oui, je me suis je confirme que, par tous moyens dans le code du travail, c'est-à-dire par tous moyens opposable, donc il faut une preuve concrète et donc il faut toujours quelque chose d'écrit simplement s'il faut qu'on réécrive par tout moyen partout dans le code, donc je vous propose de mettre à votre disposition cette analyse juridique et veut bien dire qui sous-entend qu'il y a un accord écrit et joue l'entrée d'un voilà faites confiance à cette année juridique vous dépend pas encore, je vous

Bon, donc, le 112 n'est pas retiré Monsieur Ruquier il maintient aussi donc, alors, il y avait des demandes de retrait sinon avis défavorable, hein, de la commission du gouvernement doit jamais au les 2 amendements identiques 112 et 169 rectifier avec des avis défavorables, la commission du gouvernement qui est pour.

Qui est contre. Il n'est pas, ils ne sont pas adoptées. L'amendement 167 rectifiées Monsieur Ruquier.

face à la paire de ce danger sanitaire, les pouvoirs publics ont mis en place des mesures qui se soir malheureusement révélées insuffisante et au suscité de nombreuses critiques nous passionne, qu'il existe une alternative au problème de pollution, il s'agit du télétravail aussi ne souhaite crée un droit pour le salarié au télétravail réservé à certains postes, lorsque des mesures propres à limiter labeur et les essais de la pointe du de pollution sur la population, ont été prises par le préciser, sur proposition du rapporteur nous avons rectifié autrement devant que les conditions de mise en place du télétravail Anita de pollution faut préciser dans l'accord collectif, la charte élaborée par l'employeur, nous avons entendu les craintes d'émise par la commission sur la mise à bas donne droit au télétravail opposable à l'employeur, il était toutefois rappeler que lors des pics de pollution, la mise en place de la circulation alternée ou et relativement à respecter par les automobilistes, mais nous savons partent pertinemment le à ouvrage veiller terreau gauloise, il existe malgré tout des fautifs, qui n'ont pas la possibilité de prendre les transports en commun, ni les moyens d'acheter un véhicule propre, il faut aussi, il faut chercher la réponse d'ailleurs que dans la répression, dans ces conditions, la mise en place du 31 travail toujours. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur. l'amendement rectifier va moins loin que sa version initiale qui crée un droit du salarié, opposable à l'employeur pour passer au télétravail en cas de pic de pollution mais il évitera de désorganiser les entreprises en cas de demande, nombreuses et soudaine des salariés à passer au télétravail pendant un pays de sauvages de pollution, la nouvelle version dispose que l'accord collectif où la charte devra aborder la question du passage des salariés en cas d'épisode de ce type de pollution je connais que rien dans l'ordonnance n'interdit aujourd'hui le télétravail en cas de pollution, mais je crois qu'il est intéressant de créer un lien dans la loi entre le télétravail et pollution, en raison des enjeux de santé publique liés à la pollution de l'air, la commission donc là, mais à l'avis favorable. Merci madame la ministre.

habituellement télétravail, ça veut dire que les conditions qui sont prévus dans la charte, où l'accord d'équipements de responsabilité de fonctionnement etc ne sont pas réunies donc va pas en urgence inventer du télétravail en cas de pic de pollution, je crois que c'était le sens d'ailleurs, de ce qu'a souhaité la Commission modifiée après ceci étant, c'est vrai que les cas de recours au test travaillent sur des 2 motifs. Très variés, il y a des motifs liés. On a, on le voit dans les enquêtes, souvent c'est j'ai dire c'est pour dans le clip, vie professionnelle, vie personnelle, c'est surtout par rapport à la durée, les transports, c'est souvent là ne demande numéro un en terme de télétravail, il y a une autre demande qui est de certains métiers qui suppose une concentration et où donc passer un ou 2 jours jours chez soi et parfois plus efficace et plus émet mais hier pour les 2 parties et que d'être tout le temps en situation de travail dans tous les cas, en général, télétravail, d'ailleurs, n'est qu'une partie du temps car il convient aussi de garder le lien social, entreprises, il y a aussi aussi une demande sociale qui monte, c'est pour les aidants qui parfois peuvent doivent adapter leurs horaires en fonction des et contrainte soit par rapport à des jeunes enfants ou des personnes âgées ou des personnes handicapées, il y a enfin le travail en zone rurale qui veut recourir beaucoup plus ma seule réserve qui n'est pas une réserve sur le fond, c'est que, on va créer un début et je pense qu'après beaucoup de gens vous dire mais il faut aussi qu'on réfléchisse en cas de en cas de en cas de c'est vrai que on est sur le sujet sur lequel qui sont rarement pris en compte dans le monde du travail, le sujet de la pollution et donc, compte tenu que la nouvelle rédaction dit que c'est en particulier que ça ne fait pas un droit opposable et avec l'néanmoins les réserves que j'ai dit : avant je donnerai un avis favorable. Merci, Madame la Ministre, ne jamais au voile l'amendement 167 rectifiées, qui a reçu un un double a eu favorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté, l'amendement sur 13 Monsieur Oui, toujours sur le télétravail et les Sagi de rétablir l'obligation de l'employeur, de prendre en charge les coûts découlant du télétravail, ça manque dans le, le texte, cette obligation est prévue par l'accord national interprofessionnel sur le télétravail, du 19 juillet 2005, il s'agit de l'intégrer dans les ordonnances et ça paraît tout à fait la moindre des choses que le matériel nécessaire à l'exercice du train du télétravail sont prises en charge par l'employeur. Monsieur le Président, la Commission pense que cette question de la prise en charge des frais occasionnés par le télétravail doit rester facultatives et être traitée au cas par cas et ne pas de redevenir obligatoire car je rappelle que les alinéas 7 à 11 fixe la liste des sujets impératif dans l'accord ou la charte instituant le télétravail, l'ancienne obligation étaient probablement justifiées, à une époque où nos concitoyens étaient peu équipé en matériel informatique, la situation a changé presque tous les salariés disposent d'un matériel informatique aujourd'hui, et ils ont tous un accès quasiment illimitée à Internet,

n'interdit l'accord collectif où la charte de prévoir au cas par cas n'a participation financière de l'employeur si le télétravailleur doit faire face à des coûts particulier, ce serait une demande de retrait sinon la commission a émis un avis défavorable. Merci madame la ministre. Oui, nous avons un but commun c'est développer le télétravail, c'est pour ça d'ailleurs que nous avons mis dans les ordonnances, ce droit opposable au télétravail, qui est une première européenne,

découlant directement du télétravail pour 2 raisons : la première, dans le cas des accords qui commence à se négocier ce qu'on voit c'est que il est quelquefois très compliqué de et cette mesure de simplification de distinguer dans un abonnement Internet, quelle serait la quote-part qu'il faudrait faire abonnement internet qui est prêt exister la quote-part qui est qui correspondrait au télétravail, donc concrètement le tels que s'est exprimée, c'était très compliqué, en revanche, la jurisprudence le rappelle et le juge le rappelle régulièrement l'employeur, c'est une obligation générale doit prendre en charge en ferait les frais en charge les frais professionnels nécessaires à l'exécution du travail et concrètement ce qui se passe de plus en plus de accord c'est que plutôt que à bout de l'abonnement internet qu'il impossible de dire quel serait proportion c'est quelquefois par exemple

le dialogue social, je pense, va permettre d'avoir des accords qui seront meilleures et le tout à son il y a ce filet de sécurité, c'est que, par défaut, l'employeur, il y a tenu, mais ce n'est pas spécifique au télétravail, c'est une mesure générale appartement, il était le travail à travail s'applique. Donc, pardon pour ces raisons suggérer le retrait ou sinon je traîne avis défavorable. Merci madame la ministre, donc il est maintenu, j'ai maintenu donc je le mais on voit le 113 avec 2 avis défavorables de la Commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté

dans les conditions prévues par accord collectif, il est précisé que toute contestation de ce refus doit être formé dans un délai de 2 mois sous peine d'recevabilité il convient ainsi de sécuriser toute possibilité de contestation par un délai de contentieux. Merci l'avis de la Commission, monsieur porteur. commun, posé par l'article L 4 14 71 tirer un qui prévoit un délai de 2 ans pour attaquer devant le juge une décision d'employeurs, donc c'est une demande de retrait sinon un avis défavorable. Merci mon ami. Monsieur ami. Monsieur le président, c'est également une demande de retrait vie défavorable. D'autant plus que d'avoir le but c'est de privilégier le dialogue social et donc, et des conditions qui soient définis ensemble et puis la 2ème raison, c'est que les les conditions de recours les motifs du recours au télétravail peut évoluer dans le temps, c'est parfois aussi une situation personnelle, c'est parfois il y a une situation d'une tâche particulière dans le travail et donc

on n'est pas du tout dans les mêmes sujets que licenciement, là on est par l'accord des parties sur une manière de travailler, je crois que c'est le dialogue social qui règle la question. Et ça n'est pas une limitation dans le temps du recours à toutes contestations qui est nécessaire. Merci madame la ministre est maintenant.

Pardon. Pas de souci, monsieur le Président, donc, cet amendement, s'inscrit comme le précédent dans notre volonté de favoriser le recours au télétravail en cas de pic de pollution actuellement l'article L 1222 tiré 11 du code du travail, dispose qu'en cas de circonstances exceptionnelles, l'employeur peut imposer le recours au télétravail, considéré alors comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés, il est précisé que les circonstances exceptionnelles sont notamment des menaces d'épidémies ou des cas de force majeure, notre amendement donc vise à préciser que ces circonstances exceptionnelles peuvent également être des épisodes de pollution merci. Merci, monsieur le rapporteur. Et comme l'a dit Madame Laborde, cet amendement, s'inscrit dans le prolongement du 167 que nous vont qui a eu un avis favorable cette fois-ci sera pas pareil, la Commission considère que cette précision relève du pouvoir réglementaire, comme l'avait d'ailleurs reconnu, mais l'Amérique Lamdaoui dans l'examen de la loi travail, en outre, même dans le 6 ans s'de la loi et du décret, la pollution la Commission considère que les pics de pollution peuvent déjà être assimilés à des circonstances exceptionnelles, au sens de l'article L 12 22 tiré 11 du code du travail, madame la ministre pourra peut-être nous confirmer l'analyse que nous en faisons, on attend la commission et demi à la demande de retrait ou un avis défavorable. La Ministre. Je crois qu'il est très difficile d'imposer le télétravail, d'abord on peut pas le faire en urgence et lorsqu'il y a un pic de pollution, né en urgence, par définition, il est est prévu, pourquoi, parce que ça demande tout un aménagement, un aménagement ou on l'évoquait tout à l'heure du des conditions de travail des flux d'information, télétravail c'est pas un travail isolé chez soi, c'est un travail trahi connecté suppose une collection informatique sécurisé ça demain. de définir des conditions donc, soit dans la charte et l'accord et c'était l'objet de l'amendement, il y a quelques minutes, on a prévu que dans le cas des pics de pollution telle catégorie de personnes peuvent travailler en télétravail et à ce moment-là, ça arrive, c'est directement opérationnels, soit on n'a pas anticipé de toute façon, personne ne pourra l'obliger, ça ne marchera pas, parce que tout ça demande une préparation je crois qu'on va l'imposer peu un peu théorique, l'encourager, ce qui a été l'objet de l'amendement qui a été voté tout à l'heure, permettra de prévenir ce ce type de cas donc, le contenu de l'amendement précédent je suggère un retrait. Merci un Bordeaux, explications de vote. Pour expliquer mon retrait, c'est-à-dire que je vais bien sûr retirer cet amendement mais je précise que la lation alternée ou différé parfois pire pour les entreprises, donc c'est important de le signaler et de l'anticiper, c'est pour ça que j'ai voulu insister mais je retire cet amendement. Merci, cher collègue, alors on a 11 amendements en discussion commune, il nous reste à peu près 70 amendements à discuter, on peut faire une prolongation jusqu'à 8 heures et demie mais à condition d'accélérer un tout petit peu les prises de parole et et l'examen des amendements donc ça dépend un petit peu l'accélération ou pas,

il s'agit de supprimer d'insérer un alinéa de l'article 1223 8 élargit le Champ d'application du contrat de chantier son contrat et facteur de plus de précarité qu'un contrat à durée déterminée, puisque son terme n'est pas connu et qu'il ne donne pas lieu au versement d'une indemnité de précarité. Merci, cher collègue, le 49 c'est monsieur Savoldelli. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la ministre, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, l'employeur. Ce n'est pas tenus de reclasser les salariés dans les autres établissements et surtout pris le salarié de droit essentiel, au contrat de sécurisation professionnelle qui permet un accompagnement renforcé dans la recherche d'emploi et qui garantit au salarié de percevoir 75 pourcent de son salaire brut pendant un an, et donc les mesures d'accompagnement de de reclassements externes seront plus garantis mais vont être négociés entreprise par entreprise et là quand même, ayons un moment de lucidité, la probabilité est faible de voir un accord d'entreprise qui pourrait voir, par exemple, un congé de reclassements qui maintient entre 4 à 12 mois supplémentaires le contrat de travail pour se former. Nous pensons que le volontariat des salariés qui accepteront de bénéficier des conditions imposées par la direction n'est qu'une illusion, quand on connaît la réalité des propositions imposée par la salariée pour quitter l'entreprise, je ne dirais pas à d'autres moments mais je je suis les débats depuis tout à l'heure quand on parle d'entreprise, il faut qu'on précise y compris comment évoluer une partie des entreprises quand je vous dis la pression sur les salariés, je vous dis, financiarisation de l'économie des entreprises. Et à partir de là, voyez les pressions sur celui qui dirige l'entreprise sont des pression actionnariale. dialogue social, le dialogue social, excusez-moi du peu, quand à s'financiarisée trop l'économie il y a un moment même le patron entreprise vous parle pas des sous-traitants, comment la voyez le dialogue social, c'est une autre question par rapport au au rejointe nous impulsion et aux pressions de l'actionnariat. l'amendement 42 le défend Madame Cohen. Oui, merci Monsieur le Président, l'article 30 de l'ordonnance relative à la sécurisation des raies relation de travail prévoit des temps, le recours aux CDI de chantier à d'autres secteurs que le bâtiment, selon les modalités fixées par accord de branche étendu tout d'abord, moi je l'avais déjà souligné en son temps le CDI de chantier est quand même une contradiction renferme une contradiction parce que, à ce moment-là, à partir du moment où la durée du contrat et celle d'un chantier, il ne peut pas s'agir d'un contrat à durée indéterminée avec le CD du chantier, l'employeur n'a plus besoin d'invoquer un motif de licenciement puisque la fin du projet ou du chantier suffit à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, dans une situation de précarité permanente s'opposent similitude contester la rupture de contrat de travail, alors vous nous répondent une fois de plus que les branches négocieront les modalités de recours à cette disposition et qu'il y aura donc des garanties, mais c'est la philosophie globale que nous contestons parce que pour nous il s'agit d'un nouveau contrat de travail précaire, la Fédération française du bâtiment, premières organisations patronales du secteur ne dispose pas de chiffre sur le recours aux CDI chantier dans le dans le BTP mais estime qu'il concerne surtout des projets très gros ou très long comme la construction de lignes à grande vitesse, les dirigeants de sociétés de services en ingénierie informatique notamment se frottent les mains à l'idée de bénéficier de ce contrat ultra souple dans un domaine où ces entreprises dépêchent leurs informaticiens chez les clients pour des missions plus ou moins longue aujourd'hui l'écrasante majorité des salariés de secteur Est embauchés en CDI classique rémunérer et protéger entre chaque mission un moment appeler je crois Inter constat les employeurs rêvent donc de recourir au CDI du chantier pour ne payer les salariés que le temps facturés aux clients à des tarifs plus bas que ceux des informaticiens free-lance qui sert aujourd'hui de Main-d'oeuvre d'appoint, en réalité, le compte le contrat le CDI du chantier, c'est la fin du CDI et donc pour toutes et tous et c'est pourquoi nous demandons son après son abrogation, je vous remercie. Si chers collègues, l'amendement 48, c'est monsieur Vatrin. Oui, dans la continuité de ce que vient de nous dire, Laurence Cohen nous constatons Les secteurs principalement concernée par l'extension du CDI de chantier sont la construction navale, ou bien l'industrie cinématographique vous affirmez, Madame la Ministre, qu'avec le CD chantiers, les salariés vont sortir de la précarité, disposer d'une visibilité sur plusieurs années mais le salarié ne reçoivent ne recevra plus la prime de précarité qui était la règle pour les CDD en fin de contrat, première chose, deuxièmement, cette disposition permettra aussi de contourner les protections prévues par le droit du licenciement en effet à la fin de la mission concernés qui peut durer un mois, 2 ans ou plus, le salarié pourra être licencié mais pour motif personnel comme la fin de chantier constitue un motif valable de licenciement, l'employeur ne sera pas tenu de justifier l'arrêt de la. Colombe collaboration, il est donc inattaquables devant le juge prud'homal, quant au fond, il s'agit, selon nous, plutôt de créer ici un nouveau type de contrat de travail ultra-précaire loin de sécuriser ces travailleurs vous précarise leurs relations de travail comme leur accès au logement ou aux crédits, c'est pourquoi nous demandons l'abrogation de cette disposition. Merci, cher collègue, l'amendement de rectifier qu'inquiète Monsieur Monsieur le président, Mesdames, la miss, chers collègues, donc c'est sur l'alinéa 33 remplacer le mot fixée par et selon les modalités fixées l'objet, l'Assemblée nationale a introduit un amendement pose en principe d'une priorité de réembauche de salarié en contrat de chantier, ces contrats chantiers sont aujourd'hui organisés par les branches professionnelles et leurs conditions doivent être organisées par ces mêmes branches les ordonnances prévoient d'ailleurs que ces contrats de chantier soit gérés par les branches professionnelles, estimant qu'elles connaissent les réalités du terrain et peuvent participer à la spécificité de chaque secteur, dans la continuité de ses ordonnances, cet amendement propose donc le principe de réembauche de salariés licenciés à l'issue d'un contrat d'chantiers ou d'opérations soit et négocié par les dite branche professionnelle, telle est l'objet de cet amendement.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, mais là je le rapporteur, nous avons pu voir notre groupe que la commission des affaires sociales du Sénat a autorisé la conclusion d'un accord instituant une rupture conventionnelle collective dans les entreprises dépourvues de comité social, économique, notamment en cas de de carence de candidats aux élections professionnelles, alors que l'ordonnance prévoit la mise en place d'un don comité social économique dans les entreprises d'au moins 11 salariés, la commission propose en réalité de généraliser les ruptures conventionnelles à l'ensemble des entreprises sans distinction du nombre de salariés. Romandie. N'importe quel patron de TPE pourra licencier ses salariés sans motif économique à tout moment. Alors que la loi de 2008 à instaurer les ruptures conventionnelles individuel, donc c'est une question : quel est l'objectif de la généralisation des ruptures conventionnelles collectives et selon une enquête réalisée par la Dares s auprès de 4000 signataires de rupture conventionnelle, une majorité des ruptures 57 pourcent, on est à l'initiative du salarié mais dans plus de la moitié des cas pour des raisons conflictuelles, en clair, les salariés ne souhaitant plus rester dans l'entreprise, opte pour la rupture conventionnelle plutôt que pour une démission et vraisemblablement pour bénéficier de l'indemnise l'indemnisation chômage, de même, une autre étude indique que près de 30 pourcent des salariés se disent contraints par l'employeur a signé une rupture conventionnelle en 2008 lors de la création des ruptures conventionnelles individuel le chômage atteignait 7,4 depuis ces 2,7 millions ruptures conventionnelles qui ont été signés et le taux d'chômage a grimpé à 9,4 la rupture à l'amiable n'a donc pas permis de favoriser la création d'emplois, c'est pour ça que nous sommes pour la suppression de cet article et on verra plus tard, ça me fera gagner du temps tout à l'heure, c'est que dans la suite du prolongement je sais pas si un sénatrice ou une sénateur. étant invalidée accepterait ce qui va arriver à un salarié, ouais, ouais, ouais, un salarié, il va avoir le droit d'avoir les motifs de son licenciement après la notification de son licenciement si nous les uns ou les autres, on était motif d'invalidation je croyez-moi qu'on n'aimerait pas avoir un décalage entre ce qui motive et la notification. Merci, cher collègue, l'amendement 130 Monsieur Touraine. Oui j'adhère à ce qui vient d'être dit, il s'agit de supprimer les dispositions concernant les la rupture conventionnelle collective et j'ai souligné tout à l'heure, je me suis abondamment exprimé là-dessus, par conséquent, j'ai pas y revenir mais dire simplement que j'ai vraiment une grosse crainte sur le fait que ça devienne un outil particulièrement utilisé généralisée pour remplacer des travailleurs âgés par des travailleurs plus jeunes. Merci, cher collègue, l'amendement 165 Madame Schillinger. Le présent amendement a pour objet de préciser le contrôle exercé par la directe dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, il est à ce titre, préciser que le contrôle exercé par l'administration sur les mesures de reclassement et d'accompagnement qui sont proposés dans le cadre de la rupture conventionnelle collective doit permettre à la direction de s'assurer du caractère précis et concrets de ces mesures, ce contrôle permettra de s'assurer que l'employeur met tout en que l'employeur met tout en oeuvre pour que les salariés volontaires pour bénéficier d'une aire cesser bénéficie des moyens nécessaires à leur accompagnement et à leurs reclassements, cet amendement vise en outre à corriger des erreurs matérielles.

il s'agit de donc l'alinéa 40 et 45 supprimé, c'est des Alsemberg national en plus de la Direct introduit un contrôle d'opportunité de l'administration pour la validation d'une rupture conventionnelle collective pour rappeler que la rupture conventionnelle collective simplifie et sécurise les plans de départs volontaires, cependant, la rupture conventionnelle collective est basé sur le volontariat des partis et permet de négocier les conditions des par des salariés, le fait qu'elle ne

ce nouveau mode de rupture conventionnelle collective ou la philosophie de ces ordonnances et de faire confiance à la négociation entre l'employeur et ses salariés donc dommage de revenir sur cette nouvelle confiance et des nécessaire d'éviter toute forme de contrôle abusif de l'administratif sur la RC c'est telle objet de cet amendement. Merci, cher collègue, l'amendement 14 rectifier terre Madame Bruni. Oui, merci Monsieur le Président, même la ministre,

Merci, cher collègue, l'amendement de la commission de 191 monsieur le rapporteur. Oui Monsieur Président, il s'agit d'un d'moment de coordination juridique des règles relatives à la procédure de contestation, décision du médecin du travail. Très bien, alors restez là rester là monsieur rapporteur puisque vous avez nous donner votre avis sur les 10 précédents. Je Je vais essayer Monsieur Président, à commencer par le 114 de Monsieur Touraine, donc on a déjà rejeté à l'amendement similaire, c'est donc un avis défavorable, le recours à ces contrats dans un secteur donné est soumis à 3 conditions : un acteur de branches, un accord de branche doit être conclu son contenu obligatoire est défini à l'article L. 12 23 tiré 9 notamment pour prévoir des contreparties et des garanties aux salariés mais un arrêté d'extension doit être ensuite pris par le ministre du Travail, pour toutes ces raisons, et laissons sa chance à ce contrat et faisons confiance aux partenaires sociaux, c'est donc de la part de la Commission, un avis défavorable à l'amendement 49 sur la suppression de rupture conventionnelle collective, la commission a été évidemment opposé à cet amendement car ce nouveau dispositif permet de supprimer à froid des emplois uniquement sur une base de volontariat et sans recourir à des licenciements, la rupture conventionnelle collective, on a beaucoup parlé tout à l'heure, déjà, s'inspire de 2 dispositifs qui ont montré leur efficacité tout d'abord, la rupture conventionnelle individuelle, créée en 2008 en 2016 sur 420000 demandes d'homologation reçus par la Direct, seulement 5 pourcent n'ont pas été homologuées enfin le plan de sauvegarde un emploi réformer en 2013, dont les 2 tiers sont aujourd'hui défini par accord collectif majoritaire et un tiers seulement unilatéralement par l'employeur, c'est un avis défavorable le recours à ces contrats donc de chantier dans un secteur donné est soumis à 3 conditions : un accord de branche doit être conclu son contenu obligatoire est défini à l'article L. 12 23 9 notamment pour prévoir des contreparties et des garanties aux salariés un arrêté d'extension doit ensuite être repris par le ministre du Travail pour toutes ces raisons, laissons là aussi sa chance à ce contrat et faisons confiance aux pattes sociaux et la commission a émis un avis défavorable mais amendement 48 l'ordonnance prévoit que la rupture de contrat chantier à son terme et réputée reposer sur une cause réelle et sérieuse cette présomption n'est pas je dirais fera avec un salarié peut toujours saisir le juge en cas d'abus de pouvoir ou de détournement pouvoir par leur bailleur, l'amendement cette qualification de la rupture, préférant lui substituer un motif personnel de licenciements, la commission est opposé car la rupture du contrat de chantier à son terme normal ne repose pas sur un motif inhérents à la personne du salarié, c'est donc un avis défavorable, l'amendement 2 inquiet s'cet amendement de Monsieur Chassaing, précise que la priorité de l'embauche doit respecter les modalités prévues par l'accord de branche étendu la commission il est favorable, car elle est cohérente avec les travaux de la commission, qui vise à conditionner cette priorité de réembauche à l'existence de stipulation dans l'accord,

L'amendement 130 c'est un avis défavorable, comme on l'avait déjà expliqué au niveau de l'amendement 49 l'amendement 165 de Madame Schillinger.

de l'administration sur le volet consacré aux mesures de reclassement et d'accompagnement, l'amendement prévoit que ces mesures doivent être précises et concrètes sans exercer de contrôle d'opportunité ou de proportionnalité par rapport aux capacités d'entreprise, je partage avec Madame Schillinger le souhait de faire confiance aux partenaires sociaux, qui signent un accord ont notamment assure la coordination juridique utile, la commission a donc a émis un avis favorable, a rectifié quater il est nécessaire Monsieur Chassaing, que l'administration exerce un contrôle sur cet accord, la question étant de déterminer sa portée, le contrôle doit être minimum normal ou proportionnelle un contrôle normal des mesures d'accompagnement des salariés qui acceptent la rupture conventionnelle notre commission a transformé ce contrôle normal en contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, votre amendement Jacques collègues revient sur l'apport de la commission sans proposer aucune piste alternative, la commission a donc émis un avis défavorable, enfin le 14 E rectifier terre c'est un amendement proposé par Madame Gruny qui souhaitent donc préciser que le délai de 15 jours, sentant en jours ouvrables la Commission pense ne pensent pas nécessaire d'apporter cette précision : le délai actuel de 15 jours est clair, il s'entend en jours calendaires, c'est donc une demande de retrait sinon un avis défavorable.

42 de Madame Cohen. Et 48 de monsieur votre ceux qui portent tous les 3 sur le contrat de chantier sur le contrat de chantier, de quoi s'agit-il aujourd'hui le contrat de chantier est une disposition qui existe pour le secteur du bâtiment et des travaux publics et qui permet d'embaucher sur une période de 3, 4, 5 ans en fonction de la durée d'un chantier, la durée du chantier étant un peu mobile, parce qu'on ne sait jamais exactement la fin. D et des salariés avec tous les droits du CDI, notamment en matière de formation matière d'ancienneté, il y a tout des droits sortis CDI c'est à notre Avantage aussi, c'est que sur une feuille de pas s'appelle un CDI et, ça, c'est que, comme vous le savez, une différence très importante, notamment lorsqu'on veut emprunter se loger c'est donc je dirais plus et lorsque vous demandez aux salariés s'ils préfèrent un CDD longue durée, on se dit, tout le monde préfère un CDI pour ces raisons évidentes, ceci dit. L'expérience dans le bâtiment, il y a eu, vous demandiez dénombre on a encore pour l'instant que les 5 premiers mois 2017 il y a un certain retard pour le, pour avoir le chiffre c'est c'était 20000 contrats ont été signés dans le bâtiment, donc c'est à la fois par rapport à l'ensemble des emplois dans le bâtiment, pas très important. Mais c'est c'est. Quand même significatif et notamment, c'est important dans les secteurs où la part des chantiers étant très importante les les entreprises hésitent à accepter des chantiers avec l'idée qu'ils doivent faire ensuite un plan social massif, sinon plus, un 2ème chantier donc alors pourquoi on a proposé les on a décidé dans les ordonnances de l'élargir à d'autres secteurs et à quelles conditions et avec quelques garde-fous. On a décidé, parce qu'il y a certains secteurs, vous avez cité la construction navale, c'est tout à fait le cas et on connaît d'ailleurs un chantier qui a été, qui n'a pas pu avoir lieu, pour cette raison là c'est vrai du la ce industrie cinématographique que vous avez cité aussi. ça peut être vrai de certains de, non pas tout informatique ne certains grands projets informatiques alors l'intérêt le le conditions qu'on a mis, c'est que ça ne soit pas défini au niveau de l'entreprise car là effectivement je ne suis pas sûr qu'on pourrait contrôler complètement l'usage, il faut être quand même prudent là-dessus, par contre, au niveau d'une branche, donc il y a quelques branches qui vont être concernés, pas beaucoup, ça va pas concerts. Mais les métiers de bouche. Pas des projets sur 5 ans dans la boulangerie, donc il y a certaines branches qui vont être concernées, qui vont donc négocier des conditions des conditions d'accompagnement de formation de sortie, ça répond un des amendements mais ça va permettre aussi évidemment pour les entreprises qui embauchent des salariés en CDI, si elles ont un 2ème chantier ensuite elles ont qu'un but, c'est de garder les mêmes personnes qui ont développé des compétences et donc c'est vraiment dans

des trajectoires longue durée dans des secteurs qui sont pas la majorité, mais où les chantiers sont longue durée et pourquoi c'est mieux, c'est parce que, aujourd'hui, que font ces secteurs et prennent des CDD à répétition sur ces contrats car il ne s'engage pas de façon massive sur des CDI dans des secteurs qui ou le l'essentiel de l'activité par un grand chantier, ça serait trop prendre trop de risques, résultat, il faut des renouvellements de CDD, 18 mois face et plusieurs personnes successives on l'a vu beaucoup dans ce métier-là et où, finalement, c'est dans le cadre des recours excessif ou dire de la là c'est la Afrique si sur la sécurité, nous ce qu'on souhaite, c'est une flexi-sécurité et donc il faut permettre que ces intérimaires ou CDD et une chance d'être en chantier mais c'est pour ça que ça doit être encadré au niveau de la branche et s'imposer aux aux entreprises et non pas défini par entreprise alors pour toutes ces raisons, je serais défavorable aux amendements 114 142 et 100 48 heures, je pense que nous avons défini les conditions qui permettent de sécuriser le contrat de chantier d'en faire un intérêt à la fois pour le salarié et à la fois pour l'entreprise, grâce au dialogue social dans la branche, en ce qui concerne la l'amendement numéro 49 de suppression de la rupture constructive, je suis évidemment défavorable, j'ai expliqué ce qui était la rupture conventionnelle collective tout à l'heure, mais je voudrais évoquer un sujet qui a été abordée et qu'effectivement un risque, il faut prévenir, c'est le cas où les salaires puisque c'est un accord majoritaire mais en gros, les syndicats, les salariés, l'entreprise serait d'accord pour des départs massifs en clair en près retraite payée par la surenchère je au bout du raisonnement, comment on peut l'éviter, hé bien on l'évite de façon somme c'est que l'homologation

en préretraite et payés par l'assurance chômage, ça ne serait pas possible, autre part, il faut des mesures d'accompagnement de reclassements et de formation et de mobilité, donc on voit bien que c'est pas adapté, troisièmement le les Directs ont d'ores et déjà directives sur ce sujet

à la charge de la collectivité, dans ce cas-là, ça correspond à la fois aux désirs des salariés et que l'entreprise paye intégralement avancer d'un an la retraite il y a peu d'pour entreprises qui auront les moyens de le faire, donc je pense que ça va, ça va limiter ce cas-là, qui n'est pas le cas, souhaité, mais encore une fois, si il y a pas de mesures d'accompagnement de reclassements de mobilité, etc, les directeurs ne pourront pas homologué les accords, donc on prévient comme ça ce risque-là, je voulais donner cette précision alors ensuite en ce qui concerne le l'amendement quand il y en ait parlé, donc je passe à l'amendement numéro de rectifier qu'inquiet Monsieur Chassaing sur la priorité de réembauche en CDI à l'issue d'un contrat chantier je propose effectivement un retrait sinon Roger puisque c'est dans le cadre de la négociation collective, de branche que les conditions doivent être définies donc on peut pas à la fois le soumettre ses conditions à la négociation de branche. Et prévoir et. Et prévoir plus que ce qui n'est déjà prévu, puisque le texte prévoit d'ores et déjà que les modalités de cette priorité de réembauche en s'est dit soit régie et négocié par les branches professionnelles, donc ça serait un peu superfétatoire en ce qui concerne l'amendement numéro 67 de Madame Cohen sur la suppression de la possibilité de conclure des accords RCC dans les TPE. évidemment, je suis défavorable pour des raisons évidentes appartements ou d'la RCC, je ne vois pourquoi ce qui peut être bénéfique à la fois aux salariés et aux entreprises, ne serait pas possible dans les petites entreprises. L'amendement numéro 132 Monsieur Touraine suppression RCC, donc je crois que vous avez compris ce serait un avis défavorable en ce qui concerne l'amendement numéro 165 de Madame Schillinger si on prononce bien comme ça,

les précisions sur le contrôle RCC correction des rares je suis favorable à cet amendement, effectivement plus. Il permet, il permet de sécuriser. Précise le degré de contrôle que l'administration portera je viens d'assister, à quel point il était important, et comme il va, permettent de de bien définir dans les cas qu'on a connu, c'est-à-dire on n'a pas eu besoin puisque il y a pas eu d'accord des syndicats, mais il peut y avoir des cas ou il faut qu'on vérifie que l'accord des syndicats accorder ses salariés hé bien hé bien plein et entier pour ça il faut des critères précis, ça sera le cas grâce à cet amendement,

en fait on je comprends l'intention mais en l'absence de précisions contraire il est considéré de manière usuelle et c'est intervention sont retenus par la cour de concessions que ça s'entend en jours calendaires, donc en fait, c'est déjà de droit commun. Je veux dire, nous n'avons pas besoin de donner une précision sur ce sujet, donc je lui suggérais un retrait ou sinon j'aurais un avis défavorable, enfin pour finir sur l'amendement 191 de monsieur le rapporteur, j'ai un avis favorable car ça permettra là aussi. De préciser et de d'éviter des. Protestation ou des interprétations. D'si facile à faire et. Faut faire valoir l'expression conseil de prud'hommes là qui est claire, nette et précise, donc à chaque fois que le droit est plus précis, c'est mieux pour tout le monde, merci. Madame la ministre, donc je mais au bois, l'amendement 214 avec un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté même voté pour l'amendement 49 avec 2 avis défavorables. Même vote même vote pour le 42 avec 2 avis défavorables. Même vote pour le 48. Alors. Pardon Monsieur Vatrin, explications de vote. Je vais retirer l'amendement 48 40 sommes aperçu qu'il y avait une erreur dans la formulation de notre amendement d'ailleurs mon explication l'avait montré mais je préfère retirer maintenant l'amendement du fait de cette erreur. C'est donc il est retiré l'amendement 2 Khimki acquiesce avec un oeil favorable de la commission, une demande de retrait du gouvernement et ce qui est maintenu, mais ça ça il est maintenu, donc l'avis du gouvernement et défavorable, l'avis de la commission favorable. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté, l'amendement 67 avec 2 invités. Favorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adoptée. Même voté pour l'amendement 130 avec 2 avis défavorables, ce même vote. Amendement 165 avis favorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté, donc le quater Tomba. L'amendement 14 rectifier terre demande de retrait il est retiré, merci et l'amendement de la commission et analyse favorable du gouvernement. Et pour qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté. Nous passons à l'amendement 43 qui le présente. Monsieur voteront. Oui à l'article 34 de l'ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail prévoit dans la continuité de la loi travail qu'en cas de succession d'entreprises dans l'exécution des marchés, les salariés du nouveau prestataire ne peuvent faire invoquer les différences de rémunérations résultant d'avantages obtenus avant le changement du prestataire par les salariés dont les contrats de travail, on était poursuivi, donc je prends un exemple précis récent lorsque la société Cyclocity a perdu le contrat des Vélib avec la mairie de Paris. Les contrats des salariés hanté, repris par la société Smovengo je sais pas si on prononce comme ça, qui a remporté le marché public, mais le problème est là : les salariés Vélib se sont vu proposer de poursuivent leur activité chez Smovengo, mais sans les primes, ainsi le salaire mensuel brut a été diminué 300 400 euros par rapport à ce qu'ils touchaient avant malgré leur ancienneté, donc je crois que c'est exemple monde simplement et concrètement les difficultés rencontrées par les salariés, dans le cas d'un transfert conventionnelle, faisant suite à la perte d'un marché de services et donc, il nous semble que sous prétexte de sécurisation le dispositif prévu par le gouvernement, aboutisse à abaisser le tout simplement le coût du travail ne répond pas à ce problème précis, c'est pourquoi nous demandons l'abrogation. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, l'ordonnance n'a modifié qu'à la marge les dispositions issues de la loi travail mais là seulement supprimer la notion de sites ainsi aucun salarié de l'entreprise, donc qui a remporté le marché ne pourra dorénavant invoqué des différences de traitement n'davantage conservés par des salariés transférés à la suite de l'obtention d'un marché par l'entreprise d'accueil, ce faisant, l'ordonnance recevable les contentieux fondé sur les avantages conservés par les salariés transférés en application de l'accord de branche et étendue vers l'entreprise qui a remporté le marché, quel que soit le lieu de travail des salariés requérant de l'entreprise d'accueil, le but de l'ordonnance et donc de sécuriser les transferts conventionnel dont la raison d'être et le maintien de l'emploi des salariés en dépit de la perte d'un marché par l'entreprise d'origine, c'est un avis donc défavorable. Merci madame la ministre. la ministre. Président, l'avis est défavorable parce que justement vous voulez supprimer le cadre juridique sécuriser cette reprise 7 succès d'une section d'entreprise et qui je pense est l'intérêt de tout le monde qu'on a un cadre juridique sécurisé. Merci. Madame la ministre, donc je mais l'amendement 43 avec 2 avis défavorables de la commission du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté l'amendement 116 Monsieur Touraine. Oui, cet amendement propose d'améliorer l'indemnité allouée aux salariés en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la protection de la grossesse et de la maternité. Porteur. Un petit peu plus long que Monsieur Touraine, je m'en excuse auprès de lui, je voudrais lui rappeler brièvement quand même l'objet de la réforme, un barème obligatoire avec des planchers et des plafonds, a été créé pour fixer l'indemnité accordée à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, en revanche, en cas de licenciement nul le Bahreïn ne s'applique pas le code du travail prévoyant que l'indemnité allouée ne peut être inférieure à 6 mois des salaires sans prévoir de plafond, quelle que soit la nature de la nullité du licenciement, méconnaissance des règles en matière de discrimination de harcèlement, d'accidents de travail de grossesse de maternités par exemple la commission donc pensent que les règles doivent être simples et qu'il ne faut pas créer de nouvelles exceptions parmi les un TMT accordé en cas de licenciement nul donc émis un avis défavorable. Merci madame la ministre. Oui, mais c'est présent, je rappelle que nous avons prévu donc un plancher harmonisée pour tous les cas de figure, mais par contre, dans les cas de discrimination pour différents Cox, la discrimination syndicale, où la situation de santé etc, il n'y a pas de plafond, donc tant dans le cas typiquement la grossesse, la maternité, il n'y a pas de plafond,

défavorable. Donc l'amendement 160 116 pardon je mais au bois avec 2 avis défavorables de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est corrompu. Qui s'abstient, il n'est pas adopté l'amendement 177 Madame Schillinger. Oui, il est proposé que des modèles de lettres-de licenciements soient fixées par arrêté non par décret en Conseil d'État, ces modèles pourront être plus facilement et plus rapidement être ajusté par arrêté en outre le présent amendement supprime la mention des droits et des obligations dans les modèles de lettres en effet cet alinéa peut induire une confusion quant au contenu des modèles de lettres-si ceux-ci ont bien une dizaine le 1er objectif est de notifier le licenciement, il importe donc de ne pas créer de confusion quant à la nature de ce document au regard des informations qui doivent y figurer et celle que ne se qui que facultative pour ces derniers, il appartient à l'employeur de déterminer s'il souhaite les mentionner ce qui lui sera toujours possible de faire. Merci monsieur rapporteur. Oui le le rejet et donc de l'amendement, c'est la possibilité pour un arrêté du ministre du Travail d'établir les modèles utilisés par les employeurs en cas licenciements le recours à un arrêté plutôt qu'un décret est une source de souplesse et de réactivité, la commission a émis un avis défavorable favorable. Nagui favorable, favorable, Madame la Ministre.

vices de forme, ce qui a aussi beaucoup de choses qui sont assez précisé qui est qui a sécurise les partis et y compris les salariés après ça me paraît de bon sens, de fixer, c'est c'est pas des formulaires Cerfa. Un simple Arreter pour les rendre évolutif paraît préférable qu'un décret en Conseil d'État.

Qui s'abstient, s'il est adopté 2 amendements, discussions communes amendement 44, c'est M. Cohen, qui le défend. Pardon, on est à l'amendement 44 ensuite, il y a l'amendement 117 Monsieur Cohen, c'est d'abord l'amendement 44. à la sécurisation des relations de travail prévoit de limiter le périmètre d'appréciation des difficultés économiques au territoire national cette mesure inquiète particulièrement les salariés notamment ceux des grandes entreprises, qu'elles soient françaises ou étrangères avant l'application de l'ordonnance pour déclencher un plan social, une entreprise ou un groupe qui a une implantation internationale doit justifier de sa mauvaise santé au plan international, multinationale ne pouvait pas faire de plan social si ces résultats à l'international, déclaré était bénéficiaire désormais cette même multinationale pour enclencher un plan social, si ces résultats nationaux déclarés sont déficitaires, on imagine les maquillages de comptes possibles, la majorité sénatoriale répondra qu'propose justement d'interdire les licenciements économiques lorsqu'ils sont fondés sur des difficultés artificielle, notamment en matière comptable, comme l'a souligné, notre rapporteur, je cite, les très souvent très difficile pour un juge de détecter les fraudes aux matières de licenciements économiques quand elles interviennent au sein d'un groupe international, un employeur peut en effet pendant plusieurs mois, asséché volontairement le carnet de commandes d'un site, réduire les investissements matériels ou encore diminuer les embaucher formation afin de justifier des licenciements économiques ultérieure, dans le cas des Goodyear Amiens décompte des Continental ou encore des Blanquefort, c'est toujours le même argument qui est donné par les directions des entreprises, la filiale française n'est pas rentable et ce même si le groupe effleurée florissant à l'échelle mondiale, dans le cas des Continental, qui s'étaient battus contre leur licenciement en 2009, la justice avait reconnu que les licenciements étaient illico illégaux en 2013, longtemps après qu'ils aient été prononcés dès lors pour éviter ces dérives, nous proposons de revenir au périmètre international afin de prendre en considération l'ensemble des entités constitue Steve de l'entreprise, je vous remercie. Merci, cher collègue, l'amendement 117 Monsieur Touraine. Oui, je reprends les arguments, je retiens les arguments qui ont été évoqués il y a quelques instants, et par conséquent, je ne vais pas revenir dessus, simplement rappeler que la Cour de cassation de façon constante, a demandé que lorsqu'il y avait des demandes de licenciements dans des filiales françaises 2 groupes appartenant à ou de groupes internationaux toujours demandé que soit examiné l'ensemble des moyens et des des Budgets de l'ensemble de ces établissements là c'est une régression par rapport à la situation antérieure et rien n'empêchera, même si nous sommes vigilants, rien n'empêchera, lorsqu'une entreprise, vous la quittez voudra quitter le terrain tout le territoire national ou voudra procéder à des licenciements, de s'organiser et d'organiser sur l'ensemble du groupe, les moyens de faire apparaître que la filiale française est déficitaire. Merci, monsieur le rapporteur. Le président de la commission. Pense que le choix fait par le gouvernement dans la 3ème ordonnance est un bon compromis entre le périmètre de l'entreprise, le périmètre international et que ce compromis a eu un impact très fort sur l'image de notre pays auprès des investisseurs étrangers donc émis un avis défavorable à l'amendement 44 et 117. Merci madame la ministre. Oui, évidemment je suis défavorable des amendements, je rappelle que, d'abord, la France était le seul pays européen à voir cette clause qui était considéré comme incompréhensible parler non seulement les employeurs mais les partenaires sociaux des autres pays européens, et d'autre part que la vraie protection n'est pas là la vraie protection c'est qu'effectivement la la cause économique une chance immense exploit ce s'évalue maintenant. Au niveau national sauf fraude, or les juges peuvent considérer qu'il y a fraude lorsqu'il y a notamment des remontées de près les prix de transfert ou la remontée d'évidentes et manifestement déconnectée avec la réalité économique d'une filiale en France ou d'une maison mère en France par rapport à sa filiale, le juge apprécie déjà donc cette protection d'ailleurs. Il a de fait pas fonctionner quand même, notamment en ce qui a fonctionné, c'est quand le juge a fait ses appréciations ne ne met pas plus à risques, gérer les les salariés en France et en revanche, elle va permettre une meilleure réciprocité des investissements croisés et donc des créations d'emploi notamment sein de l'Europe. Merci à mon ami. Donc je mais on voit l'amendement 44 avec un double avis défavorable commission gouvernementale qui est pour.

Et retiré. Amendement 118 également retiré l'amendement sort va. Il n'est pas retiré dommage. C'était bien parti. des entreprises qui ont la possibilité de licencier avant cession de l'entreprise, ce qui était parfaitement interdit antérieurement, le repreneur devait reprendre l'ensemble des salariés, cette suppression de l'obligation ou cette nouvelle disposition permettra à des entreprises qui ça, de spéculer sur la valeur de l'entreprise, débarrassant le repreneur d'un certain nombres de contraintes qui pouvait lui être pénible, par conséquent, je demande la suppression de cet.

de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours l'employeur établi et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, l'amendement vise à relever le seuil d'effectifs de 51000 salariés sans le vouloir, notre collègue assouplie de manière radicale les règles du PSE, ce qui n'est sans doute pas dans son intention, je crois qu'il voulait viser le 3 il y a de 3ème alinéa de l'article, qui porte sur le transfert des entité économique autonome et non pas le 1er alinéa, c'est donc une demande de retrait sinon un avis défavorable sur l'amendement, telle que

séduisant, par conséquent je vais retirer cet amendement. Donc amendement est retiré. Merci donc on a 11 amendements discussion commune le 121 Monsieur Touraine toujours. J'ai pas retiré celui-ci 221. je suis désolé de de gâcher votre plaisir. Cet article permet à l'employeur de rectifier le motif de licenciement après la notification de celle-ci aux salariés, ce qui constitue une innovation intéressante du point de vue du droit, en réalité, l'employeur n'est plus tenu d'apporter toutes les précisions nécessaires dans dans la notification de licenciement aux salariés, si bien que le salarié au moment où il reçoit de licenciement, il peut ne pas savoir exactement les raisons pour lesquelles on se prive de ses services, ce qui est ce qui ne lui permet pas de préparer sa défense de façon aussi efficace que possible et c'est un droit du salarié qui lui est encore enlevé. Merci, cher collègue, 46 c'est monsieur Savoldelli, monsieur le Président, Madame la Ministre, nous avons la même argumentation merci donc il est bien défendu. L'amendement 143.

Madame la Ministre, cirque collègues cet encadrement strict des indemnités prud'homales montre une fois de plus que les salariés sont les perdants de cette réforme et que les employeurs tentés par des licenciements hasardeux à bas Bakou seront encouragés par cette condamnation réduite, cet amendement a donc pour objet de supprimer les montant maximum du barème, c'est-à-dire les plafonds d'indemnités prud'homales nous souhaite en effet préserver le pouvoir des juges prud'homaux et leur permettent de prendre en contre d'autres critères de préjudice afin de statuer, comme ils l'ont toujours fait sur l'entier préjudice du salarié abusivement licencié lui octroyant ainsi une réparation adéquate et appropriée par là même on respecte le principe fondamental qui stipule une réparation intégrale de préjudice subis merci. Merci, cher collègue, l'amendement somme

je tiens défendent, c'est très important, bien sûr, nous avons déjà débattu du plafonnement des indemnités prud'homales mais je voudrais revenir sur les arguments du gouvernement le gouvernement et la majorité d'ailleurs ont affirmé à plusieurs reprises que le temps mis par les conseils de prud'hommes pour rendre leur jugement est source d'insécurité pour les salariés, mais je pense qu'il faut se poser la question : pourquoi en est-on arrivé là, si ce n'est parce que l'État n'a pas donné les moyens nécessaires jusqu'à maintenant, son bon fonctionnement et si nous voulons une justice du travail efficace, il faut en tirer les conséquences et lui donner les ressources nécessaires au lieu de cela est toujours sous couvert d'efficacité ou proposer une automatisation des peines et c'est là que nous avons une divergence de fond compris que vous nous dites que la barémisation des indemnités laissera encore un au juge un pouvoir d'appréciation mais je pense que ça ne tient pas la route, puisque le juge ne pourra plus tenir compte de la situation familiale ou de la mobilité géographique du salarié qui aurait été licencié et je rappelle ici de façon abusive, nous pensons pour notre part, et comme cela a été dit par d'autres collègues, que la réparation doit être en fait à la hauteur du préjudice subi, ni plus ni moins, et cela passe par la prise en compte des difficultés réelles qui sont rencontrés par la victime pour retrouver un nouvel emploi et cela ces difficultés varie bien évidemment d'un territoire à un autre, d'une personne à une autre, c'est pourquoi nous demandons la suppression de ces dispositions.

donc, quelques mots sur le plafonnement des indemnités. Des prud'homales, la charge de l'employeur lorsqu'il licencier un salarié sans cause réelle et sérieuse, le plafonnement des indemnités censées rassurer les employeurs qui serait très inquiets face au recours potentiel contre la décision de, de, pour notre part, nous ne croyons pas à cette crainte et nous ne pensons pas que modifier assouplir les règles de licenciement permettront d'améliorer la création d'emplois, d'autant que par la mise en place du plafonnement des indemnités le le juge prud'homal verra son pouvoir d'appréciation extrêmement limité et ça c'est un vrai sujet d'inquiétude, enfin, les salariés ne pourront plus obtenir droit à une réparation intégrale du préjudice comme la prise en compte de la situation spécifique du salarié en cas de licenciement abusif, je pense par exemple à sa situation familiale ou géographique, donc moins de sécuriser les salariés, il s'agit en fait de reconnaître un droit de licencier abusivement l'employeur connaissant à l'avance le prix de sa faute, donc il va évaluer finalement et il va pouvoir choisir de de licencier, donc c'est pour ces raisons que nous demandons la suppression du nouvel article tiret 3 du code du travail et le rétablissement des dispositions antérieures, alors je sais bien que quand une. C'est une loi, c'est un calme mais il faut pas oublier que bien il y a des possibilités donc d'interprétation de contournement et qu'en tout cas ce les éléments que je vous ai donné

Oui je je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, à savoir que c'est un véritable coup ce Crime en même temps qu'un déni de justice, c'est, c'est la première fois, mais moi je suis pas versé dans les affaires de droit mais c'est la première fois que je constate. Qu'on peut décider que quelqu'un qui est victime. D'un dommage particulier n'aura pas droit à une réparation pleine et entière, j'ai peur que ce soit une entorse dans les fondements mêmes de notre droit qui risque d'attirer quelques quelques tentations et, d'autre part, c'est vrai que c'est un pousse au Crime dans la mesure où le chef d'entreprise, l'employeur aura la tentation, compte tenu du prix qu'il saura qu'il a payé de de licencier et de le programmer. Mais un amendement qui propose de fixer à 12 mois le salaire d'indemnisation minimale octroyée par le juge, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail, ou que sa réintégration est impossible. Merci la commission déposé un amendement 180 monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, c'est un amendement précisions sur le Champ d'application de notion de rattrapage. D'accord, le 127 le Touraine. Les licenciements entaché par une faute de l'employeur d'une exceptionnelle gravité notamment par des actes de harcèlement et ou de discrimination sont exclus du barème obligatoire mais les dispositions qui rappelle que cette indemnité due sans préjudice du paiement des salaires lorsque celui-ci est dû, pendant la période couverte par la nullité, le cas échéant de l'indemnité de licenciement légal conventionnel ou contractuelle ont été supprimés, nous proposons de les rétablir, il n'est pas normal que la période pendant laquelle on a considéré que les licenciements étaient venus entacher de nullité, le salarié se voit privée du salaire auquel il aurait eu droit.

l'article la ligne à 17 heures, article 6 n'institut qu'un droit à l'erreur très limité pour l'employeur, il ne dispose que de 15 jours il ne peut que préciser les motifs en aucun cas en ajouter de nouveaux j'ajoute que la lettre de licenciement, précise et, le cas échéant par l'employeur fixé limite du litige en ce qui concerne motif de licenciement, la commission a donc émis un avis défavorable sur l'amendement 46 l'interdiction pour la période de préciser les motifs d'un licenciement pour mémoire je voudrais rappeler que cet article n'institut qu'un droit à l'erreur, donc c'est la même chose que l'amendement précédent et c'est un avis défavorable, l'amendement 143 l'intérêt du barème et justement d'offrir une forme de prévisibilité aux employeurs et salariés, la commission et donc opposés à la suppression des plafonds qui reviendrait à créer une incertitude similaire à celle prévalant avant les ordonnances, je rappelle qu'avant ce barème l'indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avait un plancher de 6 mois de salaire minimum n'est pas de plafond, c'est donc un avis défavorable à l'amendement 122 malgré le travail extrêmement important qui a été fait par les membres du Parti socialiste, pour essayer de nous convaincre que cet amendement était intéressante, la commission a émis un avis défavorable l'amendement 124 c'est la suppression dans le barème prud'homal des planchers lorsque le Conseil constitutionnel a censuré le 5 août 2015 la première version du barème prud'homal dans la loi, croissance et activité, c'était parce que le plafond et non le plancher de l'indemnité devait être en lien Direct avec le préjudice subi par le salarié, par conséquent le risque d'une nouvelle censure par le Conseil constitutionnel n'est pas avéré car l'ordonnance de fixe que des planchers pour les petites entreprises, c'est donc un avis d'favorable à l'amendement 45. la nouvelle rédaction proposée par monsieur Vatrin et ses collègues, les règles du barème prud'homal, c'est donc un avis défavorable de la commission, l'amendement 47, la commission est opposé à cet amendement qui revient sur la création du barème prud'homal avis donc défavorable, l'amendement 125 Monsieur Touraine. à condition de ne pas dépasser les plafonds du barème de l'indemnité sanctionnant un licenciement sans cause réelle et sérieuse et cumulable avec les autres indemnités imposé par l'employeur en cas de non-respect des procédures de consultation de la priorité embauches de l'obligation d'entreprises de moins de 11 salariés de mettre en place un comité social, économique ou, à défaut d'établir un procès-verbal de carence pour prononcer des licenciements économiques, cette autorisation du cumul permet de garantir l'objectif de prévisibilité des procédures de licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est donc un avis défavorable à l'amendement 110 reçoit lui aussi un avis femmes défavorable dans la mesure où plancher actuel de 6 mois pour indemniser un salarié victime d'années Saint-Simon nul et déjà élevé à mes yeux aux j'ai de la commission, étant entendu que cette indemnité n'est pas plafonné, contrairement à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, j'ajoute qu'un plancher systématique de 12 à 12 mois pourrait entraîner de graves difficultés pour les petites entreprises en cas de condamnation leur fermeture, attendons donc a un ou 2 ans pour tirer un 1er bilan de ces nouvelles règles internes indemnitaire et pour l'instant, c'est un avis défavorable quant à l'amendement 127 qu'il a reçu lui aussi un avis défavorable, cet amendement modifie la rédaction de l'article L 12 35 hier et 3 tiré 2 qui vise à rétablir les anciennes dispositions prévues à l'article 12 35 3 tiré un qui était totalement refondue cas de l'orgue de l'ordonnance, donc la commission souhaite revenir au niveau de l'ordonnance : avis défavorable. Merci madame la ministre. Sur les 11 amendements. Ce président alors en ce qui concerne l'amendement numéro 121 Monsieur Touraine. C'est un avis défavorable car d'amendement propose de supprimer les dispositions de l'ordonnance relative à la procédure permettant à l'employeur de préciser les motifs énoncés dans 9 des 10 sur ciment je rappelle que c'est le but, c'est de sécuriser la procédure de licenciement en amont de la procédure contentieuse car trop litiges sont aujourd'hui liées au sentiment que les griefs avait invoqué par la de licenciements sont trop peu expliquées et détaillées donc verser plus on s'en parle et plus on est précis, en amont, mieux c'est avis défavorable, ensuite l'amendement 46 de monsieur Vatrin sur la suppression de la procédure de précision du motif de licenciement, les motifs et sur le motif contaminant pour les mêmes raisons évidemment un avis défavorable l'amendement numéro 143 de Madame taillé pour Lyon sur la suppression des plafonds fixés par le barème. Je crois n'avoir beaucoup parlé au mois de juillet, dans l'heure de la loi d'habilitation, c'est tout, c'est toute l'économie de cette disposition clé ça, être sur un plancher et un plafond, je rappelle que, entre le plancher et le plafond, il n'y a pas de barème étape Aretha donc le juge a une pleine capacité d'appréciation et je rappelle ce qui est très important, c'est que le Conseil constitutionnel a validé le principe d'avoir des barèmes, reconnaissant que lors de la loi Macron il avait, il avait le, le fait que, depuis, avoir des inégalités de traitement pour les salariés de petites et moyennes entreprises, du point de vue l'intérêt du salarié, mais par contre plein principe de barème avec des plafonds avaient été acceptée, considérant que les dommages et intérêts ne sont pas forcément sans limite, parce qu'il y a d'autres considérations, prendre la situation des salariés, l'intérêt général en terme d'emploi, la situation des entreprises, donc nous sommes, je dirais, dans un contexte qu'un principe de barèmes qui est acceptée par conséquent cessionnaire avis défavorable

c'est un avis défavorable, ça été pesé, j'allais dire en fonction aussi des moyennes, mais ce qui se passe pour que ça soit dirais on soit bien dans la logique qu'on souhaitait c'est que on a on passe plus de 1 à 4 pour des motifs similaires des situations similaires et quelque chose qui s'inscrit dans la moyenne, donc je pense que montant prévu sur les plafonds et planchers prévus sont équilibrés amendement numéro 124 Monsieur Touraine sur la suppression de grève civique pour les entreprises de moins de salariés, donc là je pense.

on voit que le principe d'égalité devant la loi est respectée par les dispositions de l'ordonnance, le Conseil d'État nous l'a confirmé, donc je pense que juridiquement nous sommes robuste sur la l'amendement numéro 47 de monsieur vous proposer le retour aux textes antérieurs à l'ordonnance sur la sanction du licenciement causerait sérieuse j'essuie évidemment défavorable que j'avais dit à l'instant, les montants alloués c'est très variable d'une juridique à Sion à l'autre sont que ces écarts puissent s'expliquer par des différences de situation objective

vous voulez rétablir la rédaction précédente 2 du code du travail, en ce qui concerne la sanction du licenciement, ça causerait la sérieuse, je suis évidemment défavorable, je pense que ça fait un peu une caricature de l'attention du gouvernement et bientôt du législateur, je l'espère et je crois que vous avez tout le monde a compris que c'était contraire à l'esprit de la réforme que nous souhaitons mettre en place en ce qui concerne l'amendement numéro 123 de Monsieur

l'indemnité légale de licenciement ne vise pas la dignité légale de licenciement qui effectivement hors Champ mais les indemnités extra-légales notamment contractuelle et conventionnelle, qui sont très très différentes d'une branche à l'autre comme vous le savez, et le juge a toujours souhaité en tenir compte, plus ou moins il en tient compte, ou non, il y a pas compte, comme il le souhaite et là pour le coup, ça serait un peu une entrave à la liberté du juge qui ne nous paraît pas nécessaire en ce qui concerne l'amendement numéro 125 de Monsieur Touraine, vous proposez de supprimer le dernier le le dernier alinéa sur le cumul des indemnités dans la limite du barème, cite, un avis défavorable du gouvernement aussi le barème entend apporter la clarté, la prévisible. C'est, et le fait de.

sur le relèvement des planchers pour les licenciements nuls de 6 à 12 mois de façon générale, j'ai déjà répondu monsieur sur le non-renouvellement des les proches des plafonds qui nous paraissent équilibrées en ce qui concerne l'amendement numéro 181 du rapporteur c'est un amendement rédactionnel qui est utile et j'y suis favorable en ce qui concerne l'amendement 127 de Monsieur Touraine pour que, précisant que les salaires devraient être du même en l'absence de réintégration lorsque le licenciement est nul, je ne suis pas favorable à cet âge où il n'est pas ça c'est nécessaire, nous n'avons pas changé le droit, en l'occurrence et les dispositions relatives au paiement des salaires, même en l'absence de rata Gration n'ont pas été modifiées par les ordonnances l'intention du gouvernement et de rester à droit constant sur cette disposition. Madame la ministre, donc je mais aux voix l'amendement 121 qui a reçu un double avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adoptée, j'imagine que c'est le même vote pour le numéro 46 même vote pour le 143. Même vote pour le 122. Même vote pour le 124 pour le 45 pour le 47 pour le 125 210 donc tous ces amendements ne sont pas adoptées. L'amendement 182, la commission de précision avec un avis favorable du gouvernement, tout le monde est favorable. Est pour. Qui est contre qui s'abstient c'est il est adopté, l'amendement 127 avec un double avis défavorable commission et gouvernements qui est pour. Qui savent qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adoptée, nous poursuivons avec l'amendement française, terre de Madame Bruni. Monsieur le Président, Madame la ministre, en matière de notification de rupture, il convient de tenir compte des dispositions de l'article L 1233 65 du code du travail sur le contrat de sécurisation professionnelle 17 SP dans le cadre du licenciement économique sur ce point, la Cour de cassation a décidé que l'écrit annonçant le motif économique devait être adressée aux salariés, soit dans le document écrit d'information sur le CSP, remis obligatoirement salariés concernés par le projet de licenciement au cours de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser aux salariés, au plus tard à la date d'expiration du délai non des pose le salarié pour prendre parti sur son n'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, c'est-à-dire 21 jours après que le CSP lui était proposé, il convient donc d'adapter l'article L 1235 tiré 7 du code du travail à ces dispositions en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le contrat travailler rompu au terme d'un délai de réflexion de 21 jours dans le cas contraire, c'est la lette de licenciement voyez antérieurement l'acceptation qui vaut rupture du contrat de travail, la commission n'avait dit que cet amendement était satisfait, et en fait je voudrais avoir juste les précisions de la part de Madame la ministre, pour être certain que ce que la Cour de cassation a décidé ne vient pas entacher la loi merci. Monsieur le rapporteur. merci Monsieur Président je rappelle au préalable que le contrat de sécurisation professionnelle est un dispositif d'accompagnement renforcé que doit proposer un employeur qui envisage de procéder à des licenciements économiques dans toute entreprise de moins de 1000 salariés le salarié bénéficie en plus d'une allocation plus élevée que celles accordées par par Pôle emploi en cas dissentiment 75 pourcent du salaire journalier de référence cet amendement présenté par Grigny et selon la commission donc satisfaits par l'article L E 12 33 67 du code du travail, qui dispose que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte, rupture de contrat de travail toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle notre collègue fait référence à une jurisprudence de la Cour de cassation qui porte sur un sujet un peu différent puisque le juge a précisé l'obligation pour l'employeur d'indiquer aux salariés le motif économique due essentiellement et la priorité de réembauche dont il bénéficie, je pense que Madame Elis apporté ensuite les éléments demandés par Madame Bruni et qu'à la suite de tout ça, ben Grigny retirera son amendement. Merci, monsieur le rapporteur, Madame la Ministre. Oui, je souhaite confirmer à amassé un Trisconi que l'Artic L 12 30233 67 du code du travail prévoit déjà que toute je cite toute contestation portant sur la rupture de contrat de travail ou sous le motif se prescrit par 12 mois à à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, ce délai n'est opposable salariés que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle pour qu'il y a déjà des dispositions qui permettent d'adapter la prescription aussi spécificité du contrat, c'est pourquoi je pense que votre amendement est satisfait, je suggère un retrait sinon sur un avis défavorable. Grenier. Oui, je vais, je vais le retirer mais c'est vrai que nous avons besoin en fait d'avoir ces précisions donc je voudrais vous remercier. Merci beaucoup, donc nous passons à l'amendement 128 Monsieur Touraine. Le plancher d'indemnités dues aux salariés dont le licenciement est nul et pour lequel la réintégration ou la poursuite de son contrat de travail est impossible et divisé par 2. Ainsi, le plancher serait de 6 mois de salaire contre 12 auparavant certes au-delà de ce minimum légal la fixation du montant de l'indemnité relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge de fond mais le risque existe d'une généralisation du montant plancher de porter ainsi une atteinte grave au régime de sanctions de la nullité et c'est la raison pour laquelle nous proposons de rétablir le plancher à 12 mois. président a effectivement abaissé de 12 à 6 mois se pencher pour un motif de coordination juridique avec le plancher de 6 mois prévus pour l'indemnité en cas de nullité du licenciement du à un comportement particulièrement grave de l'employeur, dont nous venons de parler, la commission donc souhaite maintenir cette mesure de cohérence et de simplification et elle a émis un avis défavorable. Oui vraiment mise. Rapporteur merci. Donc je mais aux voix l'amendement 128 avec un double avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour.

Le plancher l'anémie étaient versées en cas de non respect de la priorité de réembauche et réduit de 2 mois à un mois encore une division par 2, ça, on pourrait penser qu'il s'agit de acharnement nous demandons le rétablissement du plancher à 2 mois.

Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté l'amendement 50 c'est. Madame. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'article 22 de l'ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail prévoit de confier à la négociation de branche les règles relatives à la durée des contrats à durée déterminée, alors que ce Champ relevé auparavant de la loi d'ordre public le nouvel article L 1242 tiré 8 du code du travail résultant de l'ordonnance numéro 2000 17387 ne mentionne même plus de durée maximale des CDD ainsi les branches ne sont plus contrainte par une durée maximale, alors que la loi fixait auparavant un délai de 18 mois renouvellement inclus le délai légal de 18 mois ne s'applique plus qu'à défaut d'accord de branche étendu de manière supplétive ces dispositions Marc le recul de la loi commune et encourage négociation de régression au détriment des protections dont pouvaient bénéficier les salariés, notamment les plus précaires, les femmes et les jeunes en sachant que les femmes sont plus souvent à temps partiel que les hommes ainsi la proportion de femmes salariées à temps partiel dans les TPE de 2 fois et demie plus importante que celle des hommes à temps partiel

le recours aux contrats courts et d'ailleurs plus fréquent dans les TPE, avec 13,1 pourcent de contrats à durée déterminée, contre 9,5 pourcent des salariés en CDD dans les entreprises de 10 à 19 salariés, il est donc indispensable donc cadré par une norme supérieure et pour ces raisons, nous demandons le retrait de ces dispositions et le rétablissement du droit antérieur. Merci Monsieur le Président, l'ordonnance donne plus de poids, selon la Comission aux accords de branche étendu pour fixer la durée maximale des CDD, leur nombre de renouvellement et les règles du délai de carence dans le respect de l'ordre public social fixé par la loi, je vous demande de faire confiance aux partenaires sociaux de la branche, la commission a donc émis un avis défavorable. Merci, Madame le Ministre. Et Monsieur le Président, Sylvain c'est issu de ce sujet de la gestion de la qualité de l'emploi, incluant les modalités concernant les CDD font partie. Désir de ce qui a été. Sortie des discussions, de concertations avec les partenaires sociaux, pourquoi, parce que l'idée c'est bien de encore une fois de faire confiance au dialogue social dans la branche pour adapter les règles parce que, selon les métiers, il peut y avoir des différences et je rappelle qu'il y a toujours le supplétif de la loi, si les partenaires sociaux ne se mettent pas d'accord, la loi s'applique donc on ne prend pas de risque par rapport au tour des salariés, par contre, prend, je pense, on fait encore une fois confiance au fait qu'ils peuvent aussi améliorer adapter par commun accord, c'est toute la philosophie des ordonnances, donc je forcément un avis défavorable. Merci donc jamais aux voix l'amendement 50 avec un double avis défavorable commission gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté l'amendement 153 Madame Fournier. Madame la Ministre, chers collègues, et il s'agit ici d'un amendement rédactionnel dont l'objectif est de supprimer toute possibilité de relèvement en cas de déchéance prononcée par la commission de discipline des conseillers prud'hommes par cohérence, d'ailleurs, avec les nouvelles sanctions prévues par la loi du 6 août 2015, merci. Merci, monsieur le rapporteur, c'est un avis favorable Monsieur probables. Madame la Ministre. Avis favorable, je pense que c'est une meilleure indexation.

Encore un recours dont la le délai a été réduit par cet amendement, nous rétablissons le délai de recours à 2 ans, quadruple sur du contrat de travail, les délais n'ont cessé d'être réduit pour sécuriser les employeurs, le délai d'un an, nous semble trop court par qui nous amènerait à la situation paradoxale dans laquelle le requérant aurait moins de temps pour monter son dossier que les tribunaux dans le aurait pour l'instruire puisque certaines procédures en région parisienne, dure près de 2 ans lorsqu'un salarié victime d'un licenciement les conséquences psychologiques peuvent être lourds dès son 1er réflexe ne sera pas forcément de mettre en question la légalité de son licenciement. Merci, pardon monsieur rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président, c'est vrai que la loi de sécurisation de l'emploi 2013 a réduit de 5 à 2 ans ce délai de prescription dans la même lignée la 3ème ordonnance à dédoubler ce délai passé Psion, il reste le de 2 ans pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail, mais réduit à un an pour les actions portant sur la rupture du contrat de travail, un délai de réflexion d'un an, et selon la Comission suffisant, je rappelle que la règle de droit commun pour attaquer un administratif, notamment quand il concerne un agent public et de 2 mois, assumant seulement donc la commission a émis un avis défavorable. Merci madame la ministre. ministre. Le président c'est un avis est défavorable, je crois qu'on a le but c'était d'harmoniser tous les délais de recours de droit commun et donc là c'est un an dans l'ordonnance c'est harmonisation mais sans dire qu'on a fait aussi une comparaison internationale que même avec un an le délai psychologique que vous évoquez, que j'entends et le et prise en compte, je rappelle qu'et ce, pour répondre à toute à l'heure, ne faisons pas toujours la France comme l'Allemagne comme modèle en Allemagne, ces 3 semaines, nous, nous considérons que ça n'irait pas du tout, donc on est sur un an, on est quelque chose d'équilibré qui est plutôt qui est plus important que beaucoup de pays européens, mais qui me paraît effectivement nécessaire. Parce que il y a le il y a l'attendent la réaction de l'émotion, après le temps de la réflexion qu'il y a le temps de la contestation, ça donne un recours, je pense, suffisant pour être équilibré là aussi. Merci donc je maison voilà Mandement 131 ans, qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est. Qui s'abstient, il n'est pas adopté l'amendement 51 Monsieur Bertrand. Oui, l'article 30 de l'ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail et instaure une présomption là encore de conformité aux dispositions de leur public pour tous les accords d'entreprise portant sur la mise en place du travail de nuit, concrètement, cela signifie que, quel que soit le motif du recours au travail de nuit l'accord bénéficient d'une présomption de l'égalité, pourtant le sait, des risques de cancer, cancer de la peau, du sein etc augmentent de 19 pourcent en moyenne pour les femmes travaillant de nuit pendant plusieurs années, un des résultats du travail des chercheurs qui ont passé en revue une étude sérieuse 60 T. analyse portant sur 3,9 millions de personnes et plus de 100000 versions chez les travailleurs de nuit de sommeil est en effet très impacté la plupart des études ont montré que le travail de nuit entraîne une réduction du temps de sommeil d'au moins une à 2 heures, mais ce n'est pas seulement la diminution du temps global de sommet qui expliquent ce risque, mais ce qu'on appelle aussi plutôt la des synchronisation ces travailleurs sont exposés en effet à des perturbations majeures de leur horloge biologique, c'est pourquoi, dans un souci de santé qui nous sommes indispensable de rétablir un encadrement du travail de nuit par un accord collectif, mais aussi de lever la présomption de l'égalité des accords d'entreprise, mais en plus, mettant en place ce dispositif. Merci, monsieur le rapporteur. Merci Monsieur président, je comprends les interrogations de de notre collègue, il ne faudrait évidemment pas banaliser le travail de nuit en raison de ses conséquences sur la santé des travailleurs mais cette présomption de l'égalité n'est pas absolue, le juge pourrait être annulé un accord ou écarter son application dans un litige individuel, s'il est manifestement contraire aux dispositions de l'article L. je vous rappelle aussi que cet article prévoit que le recours au travail de nuit est exceptionnel qui doit prendre en compte les impératifs de protection de santé et de sécurité des travailleurs et qui doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique et des services d'utilité sociale, conservons cette présomption d'égalité, nous tirons un bilan dans un an ou 2 de son application, on verra ce qu'on a pour l'instant, la commission a émis un avis défavorable. Monsieur le Président, je souhaite préciser que, évidemment, le code du travail dispose et dispose toujours ça ne change pas, que le recours de travail de nuit doit être est exceptionnelle et doivent être et qu'il est justifié seulement par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale à défaut d'définition légale des tribunaux dans le cas des contentieux engagés sont amenés à délimiter les contours de cette justification et c'est ce qui crée une certaine forme d'insécurité juridique alors, depuis la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le recours à la négociation collective est obligatoire pour la mise en place du travail de nuit l'accord collectif doit comporter des les justifications du recours au travail de nuit, celles-ci doivent correspondre à l'un des 2 cas prévus par le code du travail, la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique, où les services d'Ueli d'utilité sociale, rien ne change, là-dessus, il n'est pas question de changer, vous avez raison, le travail de nuit doit rester exceptionnel lié à ces 2 effets parce qu'on sait qu'il n'est pas sans conséquences, et donc ça ne peut pas être le mode nominal, je dirais, du travail, c'est forcément les conditions exceptionnelles, mais la loi confie également aux partenaires sociaux la responsabilité de prévoir des contreparties au travail de nuit ainsi que les mesures destinées à faciliter pour les salariés travaillant la nuit, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie professionnelle, je crois que la prise en compte d'ailleurs des sujets de santé dans ces contreparties, quelque chose qui est de plus en plus important maintenant que la connaissance sur les effets du travail de nuit. Et et je dirais plus et générale. Alors la loi effectivement on présume la légitimité des partenaires sociaux à incarner collectif dans ce domaine comme dans les autres, c'est toute l'économie des ordonnances et par ailleurs, la charge de la preuve dans le droit en général. Il. Doit incombe à la partie qui considère qu'elle pourrait toujours avoir une partie, même en ayant signé ou n'ayant pas signé qui fait un recours de conditions que on considérant que les conditions, les 2 motifs prévu parce que le travail n'ont pas été respecté mais si l'accord, que si le prêt, qui est aussi le fait et donc je pense que on est dans la société de confiance par la loi dont parle la confiance, elle est dans le dialogue social, encore une fois, ce n'est pas le pouvoir unilatéral de l'employeur, je rappelle que maintenant tous les accords devraient majoritaire, donc c'est quand même d'un exigeant sur le dialogue social qui est forte et que dans le cas de du rôle des partenaires sociaux en la matière nous ne changeons rien sur les conditions exceptionnelles du travail de nuit ne change en rien sur le fait que les partenaires sociaux doivent négocier les contreparties et les conditions

droit social à partir des ordonnances qui est que oui, l'accord a une valeur, les partenaires sociaux font aussi attention à l'intérêt général et à l'intérêt des salariés, je pense que donc nous suivrons sera bien évidemment aussi, mais je n'ai pas l'inquiétude sur ce sujet, quand je ne connais pas d'accord, de nuit, sur lequel il y a, il y a pas des un encadrement très fort par les partenaires sociaux, encore une fois, s'il y avait un dérapage, il y aura un recours et le juge pour l'évaluer. Donc c'est un avis défavorable, alors l'amendement 51 jamais bois. Explications de tous, c'est notre.

il nous dit, indique effectivement il y a des recours possibles contentieux mais en cas litiges individuels, on voit tout de suite, on peut imaginer tout de suite les difficultés d'avoir recours à ce processus. j'entends bien que c'est un dispositif exceptionnel mais bon, on voit aussi, j'ai pas le chiffre en tête, mais qui a des des millions de de travailleuses notamment qui sont concernés, donc en lien avec ce que je disais sur la récurrence des des cancers ce problème me paraît quand même un peu nécessaire d'être traités pneus manière un peu plus sérieux, il me semble, parce que renvoyer au dialogue social, c'est peut-être un peu facile, on est sur un problème de santé publique et dire que dans le cas de l'entreprise, on va pouvoir régler les toutes les questions liées à ce sujet me paraît un peu ambitieux, moi, moi, je veux simplement dire ici aussi que la loi que vous proposez ne règle pas un recul qui a été enregistré dans la précédente loi travail parce que sous couvert de pénurie de médecins du travail rappelle que la loi elle Comrie a acté un recul des visites médicales, qui a été pendant très longtemps prévu tous les 6 mois et je crois qu'on a, on a reculé beaucoup sur ce sujet, donc je pense quand même, ça fait beaucoup d'arguments beaucoup d'choses qui font que, malheureusement, ce qui ressortira c'est que on on ne on banalise le travail de nuit, alors que c'est un problème de santé publique et puisque on propose d'aller vers l'égalité femme et que beaucoup de de de femmes sont victimes du travail de nuit, il me semble que qu'une question qui aurait dû être traité autrement.

Oui, merci Monsieur le Président, l'article 33 de l'ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail prévoit de faciliter le prêt de main-d'Oeuvres des grandes entreprises, vers les petites concrètement pendant une durée d'au d'au d'plus 2 ans, les groupes ou les entreprises d'au moins 5000 salariés pourront mettre à disposition leurs salariés auprès de jeunes entreprises de moins de 8 ans d'existence ou des peines modo plus de ceux dont plus de 150 salariés, cette opération sera considéré comme dépourvu de but lucratif, y compris lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur au salaire versés aux salariés, aux cotisations sociales et aux frais professionnels, une telle disposition permettra pour les grandes entreprises d'externaliser leur Main-d'oeuvre dans les petites entreprises qui deviendrait de fait leurs sous-traitants, sans qu'elles assument la totalité de la prise en charge des salaires, il y a un fort risque de notre point de vue d'accroître le pouvoir des donneurs d'ordres sur les sous-traitants, c'est pourquoi nous demandons l'abrogation de cette disposition.

1397 du 22 novembre 2017 a introduit un nouveau dispositif de prêt de main-d'oeuvre à but non que lucratif destiné à sécuriser la mise à disposition des salariés souvent hautement qualifiés apportant leurs compétences à des jeunes entreprises ou des PME afin d'assurer que les structures bénéficiant aujourd'hui du mécénat de compétences qui prend souvent la forme d'un prêt de main d'homme puisse bien s'inscrire la accueil, les salariés, accueilli par elle pour des projets d'intérêt général ou d'utilité sociale dans ce nouveau cadre juridique, cet amendement disent à étant expressément la définition des entreprises utilisent utilisatrice figurant à l'article L. 82 41 tiré 3 du code du travail à ces personnes morales dont la liste est fixé dans le code général des impôts ainsi des structures associatives ou des fondations, par exemple, pourront accueillir dans les conditions prévues par le code du travail des salariés de grandes entreprises, sans encourir aucun risque juridique ou fiscal, par ailleurs, l'amendement précise possibilité de facturation des charges qu'on est cependant aux salariés prêtés par son employeur à l'entreprise d'accueil en confirmant la possibilité des prêts à titre gratuit avec une facturation de charges nul qui pourront bénéficier à des entreprises ou associations disposant des de moyens très limités pour s'attacher l'apport de compétences nouvelles. je voudrais Monsieur Vatrin dissiper un malentendu, contrairement à ce qui est écrit dans l'objet d'amendements, l'entreprise prêteuse devra assumer la totalité de la rémunération des salariés mis à disposition, qui concerne évidemment leur rémunération d'origine, ce n'est que dans la facturation du pré-calculé par la grande entreprise qu'elle pourra prévoir un niveau inférieur à son coût réel afin de donner un coup de pouce à l'entreprise d'accueil justement concrètement un ingénieur chevronné, employé dans un grand groupe, pourra conserver son salaire lorsqu'il est mise à disposition d'une Start-Up, tandis que l'entreprise d'accueil ne remboursera par exemple que la moitié du coût très réelle du prêt, donc c'est un avis défavorable donné par la Commission à l'amendement pour ce qui est de l'amendement de Madame Schillinger, il s'agit de l'élargissement des bénéficiaires du prêt de manoeuvre à but non lucratif, aux associations, cette élargissement du dispositif apparu utile à la Commission, car si on ne mentionne pas explicitement les associations pourraient être exclus du dispositif, l'amendement précise également que la facturation du prêt de la structure prêteuse la structure d'accueil peut-être nul, afin de ne pas remettre en cause l'action de mécénat de compétences qui existe aujourd'hui, c'est donc un avis favorable. Merci mon ami. Oui, ce président les 2 amendements portent sur le sujet du mécénat de compétences, quelle est l'idée, l'idée c'est que les grandes entreprises qui veulent aider le leur écosystème de start-ups de PME autour d'elle ou bien dans l'. 4 de leurs mécènes, faire du mécénat de compétences il y a une forte demande des salariés, souvent de pouvoir aller aider quelques mois sur un projet parce que il y a des compétences dans un groupe qui n'existe pas dans une association, nous donne une petite entreprise de pouvoir aider pour un projet industriel produit marketing, en sachant que ces compétences-là ne serait pas accessible financièrement à l'association ou la petite entreprise et qu'il n'y en a qui est le besoin n'est pas forcément permanent, j'ai eu l'exemple. Vécu d'une. Grande association de l'aide alimentaire ou par exemple des sujets de logistique sont extrêmement complexes et où finalement le message compétence et parmi une grande entreprise de des les jeux des ingénieurs logisticien quelques mois le temps de monter un système qui a permis à la gestion de changer d'échelle dans la banque alimentaire, pareil pour les Start-Up, il y a souvent besoin de recherche et développement de marketing au départ n'ont pas les moyens, donc c'est un formidable moyen de à la fois de motivation souvent pour les salariés, pour les grands groupes, c'est donc de céder à un prêt de au sens du mécénat de compétences qui va être père mi-aujourd'hui qui n'était pas sécuriser juridiquement qui souhaitait parfois sur cette sécurité juridiquement, donc je pense que c'est une bonne chose, c'est d'idée quand même que les entreprises de taille moyenne ou grande peuvent aider des petites entreprises ou des associations a démarré à se développer, je. Parce que c'est aussi une solidarité de compétence qui est intéressante, donc, pour ces raisons-là, évidemment je serai défavorable à l'amendement numéro 52 de Madame Cohen est favorable à la demande en 161 Nam Schlinger. Merci madame la ministre, donc je mais voire amendement 52 avec un double avis défavorable, commissions et gouvernements qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté l'amendement 161 rectifier avec un double avis favorable comme ils ont gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté. Mais voit maintenant l'article 6. Qui est pour. Qui est quand même. Qui s'abstient, il est adopté article additionnel après l'article 6 l'amendement 53 Monsieur Guey. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le fait que la question des licenciements dits boursiers est une vieille histoire et que cela fait déjà quelques années que l'opinion publique à l'occasion de se scandaliser de la manière dont certaines directions d'entreprises se sépare d'une partie de leurs salariés, différent du licenciement pour motif personnel qui tient à la personne même du salarié ou pour motif économique, caractérisée par des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, même s'il y a, il y aurait des choses à dire le seul Issam Simone boursier est inacceptable, or ce dernier présente la particularité de peser sur les salariés qui, elles, sont victimes alors même que les entreprises qui les employait jusqu'alors ne connaissent aucune difficulté particulière ni prévisibles aujourd'hui, les entreprises peuvent licencier alors qu'elles sont prospères, elles peuvent même licencié dans le seul but d'accroître la rémunération des actionnaires, c'est en 99 que l'affaire Michelin a mis en évidence ces situations, chacun se souviendra par exemple que cette année-là, la direction annonçait simultanément, donc des bénéfices semestriels en augmentation de 20 pourcent une augmentation des dividendes et 7500 suppressions d'emplois, suivi dès le lendemain par une progression de 12 pourcent du cours de l'action, plus récemment, en 2010 Alstom qui avait annoncé vers Gül 22 2 milliards de bénéfices, a décidé de supprimer 4000 postes, on sait où cela nous a mené aujourd'hui, avec les risques de démantèlement de l'entreprise, chaque semaine, chaque jour des entreprises bénéficiaires décide de licencier afin de conserver les marges de profit nécessaires à une importante redistribution des aux actionnaires désormais avec les ruptures promotionnel collective Carrefour, la Société Générale, Peugeot et les autres pourront sans sourciller licencié pour accroître leurs dividendes notre amendement vise justement refusé cela et interdire que les entreprises championnes des dividendes versés aux actionnaires, licencient leurs salariés sans état d'âme. rapporteur. Ce président notre commission a eu déjà repoussée de très nombreuses fois cet amendement ou dits boursiers, c'est un avis défavorable qu'elle a émis cette fois-ci encore. La ministre madame la ministre, s'il vous plaît. Il y a eu aussi ce débat est donc je le même avis que le rapporteur. Donc, mes chers collègues. L'amendement 53, donc avis défavorable de la commission avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui et quand. Qui s'abstient, il n'est pas adopté l'amendement 54 Madame pruneaux. Merci monsieur le président c'est amendement vient en en complément de celui que vient de de présenter mon collègue Fabien Guez Fabien Guez donc je présente prévoit le remboursement des aides publiques lorsque le licenciement pour motif économique aura été jugé sans cause réelle et sérieuse, notamment en cas de licenciement économique boursier l'entreprise se verra condamné à rembourser le montant des exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié au titre de l'ensemble des c'est là des salariés initialement concernées par le licenciement ou la suppression d'emplois, par ailleurs, l'entreprise prendra le cas échéant le bénéfice ou l'opportunité de bénéficier du crédit impôt recherche ou du crédit impôt comptabilité, le fameux CICE enfin, le juge pourra ordonner le remboursement de tout ou partie du montant dont aurait bénéficié l'entreprise au titre du CIR et du CIC, je vous remercie. Si l'avis de la commission sont porteurs. Oui c'est un avis défavorable Monsieur Président, on a déjà repoussé plusieurs fois également, je voudrais, puisqu'on demande des interventions j'interviens, je rappelle qu'en cas, licenciement économique, sans cause réelle et sérieuse, le juge peut ordonner le versement des indemnités, en application d'un barème l'amendement pose aussi un problème majeur, il ne prévoit pas sur combien d'années le remboursement des réductions de cotisations patronales peut porter un an, 2 ans, 3 ans ou plus, donc pour toutes ces raisons, la Commission avait émis un avis défavorable. C'est madame la ministre. Oui je tout en ayant un avis défavorable je comprends l'intention, je pense que c'est pas en ayant une mesure universel qui s'applique à tous les cas, il y a licenciements économiques et licenciements économiques contexte contexte par contre je pense qu'à chaque fois qu'il y a des engagements spécifiques vis-à-vis d'une entreprise je pense notamment à certains dans l'actualité, il est clair que quand il y a un engagement vis-à-vis de l'état d'une entreprise sur un certain nombre de choses, s'il y a licenciements qui peuvent intervenir, ce qui a des nouveaux effets économiques qui arrive, il faut à ce moment-là qu'est le respect complet des engagements donc je le mettrais sur un autre terrain,

donc on ne peut pas avoir une mesure qui Universal qui gérait sanctionneraient de tous les cas de figure, qui ne correspondent pas du tout la même situation, je pense que par compte les engagements contractuels qui sont faits et c'est d'autres gouvernements si employes il y a un certain nombre d'entreprises qui ont pris des engagements contractuels ce contact changer peut y avoir des raisons licenciés mais c'est pas d'un pas respecter un certain nombre d'engagements, donc je pense que c'est plutôt dans ce terrain-là que ça se joue, donc je suis défavorable à l'amendement, mais je comprends l'intention et je pense que sur un autre terrain, nous continuerons à agir. La ministre genèse au voile amendement 54 avec un double avis défavorable la commission du gouvernement qui est pour.

Merci monsieur le président, avec cet amendement, nous vous proposons d'une part, d'encadrer le recours des entreprises au contrat de travail à durée déterminée afin que ces contrats cesse d'être utilisés comme des variables d'ajustement, nous vous proposons d'autre part, de limiter le nombre de personnes en contrat à durée déterminée à 10 de l'effectif total dans les entreprises d'au moins 11 salariés, ces 2 mesures contraignantes visant à lutter efficacement contre la précarisation du marché du travail qui pèse sur les salariés en 1er lieu sur les femmes, comme nous avons eu l'occasion de le préciser, à plusieurs reprises le total des CDD, intérimaires, des CDD, des intérimaires et des temps partiels subis représente 4 millions de personnes, la proportion des emplois précaires, traduit aussi la spécialisation de la France dans des productions à Bakou salariaux au détriment de l'exigence de montée en gamme de notre industrie, nous proposons donc avec cet amendement, de limiter le nombre de personnes en CDD dans l'entreprise, en fixant un plafond à 10 pourcent de l'effectif global dans les entreprises de plus de 10 salariés. Merci, monsieur le rapporteur. d'avoir ce débat au printemps prochain, lors de l'examen du projet de loi sur l'assurance chômage, puisque le gouvernement pourrait à ce moment-là, proposé de pénaliser les entreprises qui utilisent beaucoup de contrats courts, peut-être à travers un système de bonus-malus pour l'instant, c'est une demande à par des commissions de retrait, sinon ce serait un avis défavorable, on attend dans ce débat. Madame la Ministre. Vous êtes président, j'ai déjà répondu à un débat similaire tout-à-l'à heure contenu que la question de la de lutter contre la précarité dans les règles de l'assurance chômage est déjà une question sur lequel j'ai interpellé les partenaires sociaux qui sont en train de discuter et que nous aurons là l'occasion de discuter printemps dans un débat législatif, je propose le retrait, sinon j'aurais un avis défavorable. Il est maintenu, il est maintenu. Donc le jeu mais où l'amendement 55 avec un double avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté l'amendement 57 Monsieur Bertrand. Oui, je crois qu'avant de le défendre, tout le monde a bien compris qu'on est sur toute une série d'amendements bon alternatif qui propose d'aller plus loin que la réglementation actuelle donc poser des, des, des, des sujets d'avenir dites sur les licenciements boursiers que finalement peu toujours rester en justice, on peut toujours qu'il y a pas de cas pareil André simplement le cas de d'une commune à proximité de mon lieu de résidence s'appelle Hénin-Beaumont et où il y a eu des centaines de salariés victimes de licenciements boursiers, je pense que vous connaissez aujourd'hui l'étiquette politique de cette ville ne pas légiférer sur ces questions, renvoyé à plus tard y à d'autres débats, à un moment donné on le paye d'une autre manière et sur le plan politique, alors ici on est sur la diminution du temps de travail, et encore un autre sujet de société, et je pense que nous entendons bien que il y a un débat sur le le sujet je crois que chacun ici, reconnaît les mutations dans le travail et la nécessité de repenser le travail et l'idée que les progrès technologiques, notamment l'émergence de l'interdit gens artificiel bouleverse le monde du travail simplement ici comme sur les autres sujets licenciements boursiers, la limitation des contrats précaires, pensons qu'il faut agir et qu'il faut au moins qu'on ait ce débat sérieusement ici dans leur hémicycle une bonne fois pour toutes, sinon, vous aurez toujours nos amendements sur de nombreux textes alors ce que nous proposons n'est pas une idée nouvelle, on sait que les 35 heures ont permis par exemple de la création de 350000 emplois, on sait que les progrès technologiques vont faire que ce sera difficile de trouver une place à chacun dans la nouvelle société de travail, on est à 39 heures et demi temps effectif de travail il y a des marges de manoeuvre pour s'interroger sur une réduction réelle du temps de travail possibilité d'aller vers par étapes vers les 32 heures nous paraît être une bonne solution, donc nous voulons par cet amendement anticiper la mutation du marché du travail et donner à nos concitoyens à plus de temps pour s'engager différemment au service de la société. Merci, cher collègue, l'avis de la commission. C'est. C'est une un avis défavorable je reviendrai pas sur les 35 heures, en particulier sur les conséquences au niveau des hôpitaux par exemple, je voudrais juste dire que pour l'instant la proposition telle qu'elle est faite dépasse le cadre du projet de loi de ratification il correspond pas à l'analyse que la Commission peut avoir sur les enjeux économiques auxquels nos peut-être notre pays est confronté, elle a donc émis un avis défavorable. à la ministre. Monsieur le président, je crois que nous avons ouvert dans la loi d'habilitation sur qui a indiqué que nous pourrions modifier le temps de travail, l'ensemble des salariés en France, je crois que c'est un petit peu hors sujet de la loi de ratification pour les mêmes raisons, après on pourra débattent sur le fond mais.

Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté l'amendement 58 de M. Cohen. points particulièrement en avant pour vanter ses mérites, ici même dans notre haute assemblée, c'était la mise en place d'un plancher de 24 heures minimal hebdomadaire, l'objectif était bien évidemment d'en finir avec les mini-contrat de quelques heures qui ne font qu'entraîner de la précarité, nous avions bien évidemment soutenu cette mesure qui allait pour nous dans le sens d'une amélioration des conditions de travail, notamment des femmes qui, on le sait, sont majoritairement concerné malheureusement très vite et nous l'avions dénoncé cette mesure positive a été suivi de très nombreuses dérogations dans les entreprises, ce qui a rendu caduque cette belle ambition, c'est pourquoi nous proposons en travers de cet amendement de majorité à un taux de 25 pourcent les heures de travail comprises entre 15 heures hebdomadaires et 24 heures hebdomadaires pour une durée de travail inférieure ou égale à 15 heures par semaine, ou lorsque la durée quotidienne du travail est inférieur à 2 heures, nous proposons que ses heures de travail soit rémunéré à un taux majoré de 50 pourcent ces majors à ces majorations ont à la fois pour but de compenser, de faibles salaires, du fait du petit nombre d'heures effectuées et à la fois dissuasif pour les entreprises, trop de femmes travaillent à temps partiel de façon subie, il est temps pour nous de faire de mettre fin à ces discriminations, genre qui ont des conséquences au quotidien sur les salaires et les retraites, voici Madame la ministre, une nouvelle fois. L'occasion de faire évoluer les choses, alors parfois on nous dit que c'est pas le bon véhicule bon vecteur etc plutôt mais au bout d'un moment il faut agir et nous ou pense que c'est pas mal sur ses ordonnances, qui concerne les conditions de travail. rouvrir le débat sur le temps partiel dans ce texte ne ne semble pas utile pour l'instant, donc je veux dire aussi que l'idée de majorer aussi fortement le coût du travail pourrait être très néfaste pour certaines entreprises, donc elle a émis un avis défavorable. Madame la Ministre. Dans le cas des débats autour de la loi travail qui a pas prévu la loi sur la souvent du dialogue social, on n'a pas prévu de traiter ces sujets-là, on a eu gère les 2, les 2 mouvements, on vous proposait de majorer les paiement des heures effectuées en deçà de 24 heures par semaine, d'autres ont proposé de relever et 24 heures ou de supprimer les 24 heures tout entend mais ce qui est certain, c'est que c'était pas dans le Champ de ce que je tiens à rester strictement dans le Champ de la loi d'habitation, donc je prolonge pas le débat là-dessus parce que c'était pas dans le Champ de la loi. Merci Cohen. Explications de vote. Oui, parce que je, j'entends les les arguments mais là tout au au cours de de cet article avec mon groupe nous avons fait un certain nombre de propositions pour combattre la précarisation de la flexibilité du travail, on nous dit que c'est pas le bon vecteur sur les 24 heures c'est pas seulement s'attaquer au temps partiels subis monsieur le rapporteur, mais c'est le fait qu'il y a une attaque aujourd'hui et qui concerne notamment les femmes, sur le fait qu'il y a eu plein dérogation ainsi 24 heures et du coup ça fait des petits boulots de, de, de quelques heures, alors je veux bien que ça ne soit pas le moment, le lieu, etc, mais j'attire l'attention du gouvernement et de d'autres Haute assemblée parce que à un moment donné, il faut effectivement ensemble, trouver des solutions qui remédie un problème durement vécue par une partie de la population qui est non négligeables faut autant on trouve souvent des solutions et notamment au niveau des grands groupes etc on arrive à débloquer de l'argent pour soi-disant créer de l'emploi et on voit bien que ça marche pas, autant là, je pense qu'il faut avoir la même détermination et je souhaite être entre du j'ai entendu Madame la ministre hier que c'était une une préoccupation globale cette égalité professionnelle et voilà je, je trouve que c'est important, mais ce que nous dénonçons aussi au niveau des des petits boulots de quelques heures, ça fait aussi partie de l'accroissement des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes, et je souhaiterais donc que ça fasse aussi l'objet de la réflexion que vous allez mener et que nous avons envie de mener avec vous pour aboutir parce que on a envie d'aboutir pour améliorer les conditions de travail des femmes notamment. Merci, cher collègue Monsieur Cannet pour explications de vote. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, je ne voudrais pas laisser croire que dans cet hémicycle, tout le monde considère qu'il faille mettre des contraintes supplémentaires pour les entreprises et considérer que le temps de travail soit constamment subi et pas choisi, il faut aussi penser à tous ceux qui ont envie de choisir un temps de travail qui soit inférieure à la durée légale du travail et les discours tels qu'on les entend la tendent à considérer que l'ensemble de des salariés seraient exploités, ce n'est pas du tout la réalité dans les entreprises sur le terrain et donc je ne veux pas laisser dire c'est ce message au sein de notre hémicycle en même temps que depuis un certain nombre d'amendement j'observe Monsieur le Président que alors que nous considérons tout ce qu'il y a trop de normes et de contraintes dans notre pays on ne cesse de proposer des normes et des contraintes supplémentaires qui vont faire quoi qu'ils vont faire ce qu'on a observé ces dernières années, c'est-à-dire le chômage qui augmente, alors qu'il faut tout faire pour que l'emploi soit au coeur de nos premiers. Merci, cher collègue Monsieur Chassaing pour explication de vote. Oui, très rapidement, très rapidement Monsieur Président donc Madame Cohen effectivement dans ses propos, essayer de trouver du travail pour que ce soit un salaire décent pour les femmes, je suis d'accord mais si vous voulez, il faut faire attention lorsqu'on met des contraintes parce que moi j'ai été président d'une association dans le secteur rural qui a embauché des des femmes pour faire donc

encore et le nombre de personnes suffisant pour pouvoir travailler plus de 24 heures et donc ça a été un handicap, donc il faut bras effectivement dans le dialogue qui aura pour cela, il faudra aussi prendre en compte ces problèmes parce que si on met une contrainte de 24 heures et bien au départ, on n'aura peut-être pas les heures et on prend pas embaucher des personnes. Merci, cher collègue, donc je mais aux voix l'amendement 58.

Madame la ministre, mes chers collègues, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire a annoncé présenté en mars. Un projet de loi pour transformer l'entreprise et leur permettre d'innover, se transformer, grandir et créer des emplois. Alors que nous sommes constructifs avec le groupe nous avons sur les communistes constructif, on le voit, on apporte un certain nombre de propositions, nous sommes minoritaires mais nous continuons à les mettent sur la table et à faire grandir le débat dans ce pays, j'ai entendu tout à l'heure monsieur le rapporteur milliards ça fait très longtemps qu'on entend cela, oui, mais comme ça continue, on propose et on continu, ramené le débat. Nous avons donc une proposition de mesures au ministre pour transformer l'entreprise c'est cet amendement qui propose d'encadrer les écarts de rémunération au sein d'une même entreprise sur un rapport alarmant de avec il y a débat là aussi s'apprête de à 10 à 30 nous nous proposons de avec l'encadrement des salaires a été mis en place dans les entreprises publiques, avec un plafond de rémunération de 450000 euros. En place dans les entreprises publiques, nous proposons donc d'aller plus loin, en encadrant les salaires des entreprises publiques mais aussi privées de avec. J'ai bien écouté ce que propose notre collègue alors il dit que monsieur Bruno Le Maire a proposé un projet de loi concernant les entreprises, pour le mois de mars, nous sommes en janvier, il dit ensuite qu'il fait des propositions au ministre, pas des propositions qui doivent donc rentrer dans cette loi, puisque cet homme seul le n'était ne prévoyaient pas ce genre de proposition, donc c'est nul et on avenue pour ce soir, on en reparlera avec Bruno Le Maire en mars. Donc c'est un avis défavorable. Ma mise. Même sa ration que le rapporteur, c'est juste que ça ne sera pas mars mais ça sera au printemps par contre avec un esprit un petit peu l'escalier parce qu'il y a le même mot rémunération je voudrais rebondir sur ce que disait Madame Cohen tout à l'heure, ce que je vais demander, c'est parce que il y a des professions il y a des branches qui ont négocié et celles qui sont plus utilisatrices du temps Monaco 4 heures qu'on ait une analyse d'abord femme et puis aussi des contreparties qu'elles sont faites donc dans le débat qu'on aura dans la réflexion qu'on aura sur l'égalité salariale hommes-femmes se faire faire un examen plus particulier, des moyens, des branches qui ont où il y a beaucoup de travail à temps très partiel, moins de 24 heures pour qu'on est en tout cas une analyse complète de la situation, je ne sais pas si on sera d'accord sur les solutions, mais en tout cas je voudrais, je pense que c'est un sujet, il faut qu'on regarde et quel type de contrepartie ont été négociés.

Merci, cher collègue, donc l'amendement 64 c'est madame Bruno. Merci monsieur le président, autre exemple et autres futures propositions de de notre groupe, le, le taux de chômage des jeunes actifs c'est établi à 22,6 pourcent à la fin du 1er semestre 2017 selon les récents chiffres du ministère du Travail si la plus part des indicateurs économiques sont au Vert, le chômage des jeunes reste particulièrement marquée en France, les jeunes constituent en fait une véritable variable d'ajustement en cas de crise ou de récession et il se pourrait que la situation ne s'améliore pas vraiment dans les mois à venir, cet amendement, ce que nous proposons une solution innovante, c'est-à-dire on souhaiterait réserver 10 pourcent des nouvelles embauches aux jeunes de moins de 25 ans, c'est une des propositions, je vous remercie. Oui, donc l'amendement propose l'obligation pour les entreprises employant plus de 20 salariés de consacrer au moins 10 pourcent de leurs embauches des jeunes âgés de moins de 25 ans cet amendement dépasse, il faut encore le cadre de la loi d'habilitation certains je voudrais dire quand même que certaines entreprises réservent déjà plus de 10 pourcent de leurs embauches à des jeunes, alors que l'amendement vise uniquement le seuil de 10 pourcent en outre une approche purement mathématique n'est sans doute pas adapté à la complexité du sujet du chômage des jeunes, la vraie question est plutôt celle de leur formation et de leur adaptation besoin d'entreprise donc là pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis, une demande de retrait ou un avis défavorable. Merci dans la ministre.

les les ordonnances que nous avons examiné, nous avons vu que on revenait sur la quasi intégralité du code du travail telle que nous le connaissons mais par contre, n'avons pas trouvé de dispositions répondant à la question du développement du numérique au travail et notamment des plateformes type Hubert en France leur ça engager des procédures et les travailleurs des plateformes s'organisent pour faire reconnaître le lien de subordination qui les lie alors employeurs par cette amendement, nous proposons de mieux les protéger en instaurant une présomption de salariat fondée à la fois sur le lien de subordination juridique et sur la relation de dépendance économique, en effet, ces travailleurs sont aujourd'hui doublement privés de protection n'étant pas salarié n'ont pas droit aux dispositions protectrices du code du travail n'étant pas réellement indépendant non plus il ne bénéficient pas de la protection économique coffre donc cet état-là, c'est une situation à laquelle il convient de mettre un terme, cet amendement, nous en donne, nous semble-t-il l'occasion. C'est un amendement donc qui vise à présenter des des critères pour identifier une relation salariale afin de supprimer le statut de faux travailleurs indépendants, c'est un moment extrêmement intéressant il vaut le coup qu'on en discute et qu'on en reparle, par la suite, il dépasse cependant la le projet de loi de ratification est le projet d'habilitation, par ailleurs, donc c'est une demande de retrait pour en parler plus tard mais enfin c'est ça, ça valait coup d'en parler. Sinon, un, qu'il Madame la Ministre. L'avis du gouvernement sur l'amendement 60. il y a des discussions et on y reviendra dans le cas de l'assurance chômage ou souhaite que les travailleurs indépendants puissent avoir un filet de sécurité, et parmi les travailleurs indépendants, il y a des micro-entrepreneurs et il y a travers des plateformes, donc il y a des sujets aussi récemment de la prise en compte d'accidents voilà donc, donc on est sur un sujet qui est clairement des travailleurs indépendants mais dont l'activité il y ayant un lien peut amener certaines obligations pour les plateformes numériques qui leur donne du non pas un emploi mais une activité, donc nous n'aura l'occasion d'y revenir, là aussi dans la prochaine loi décidément, quelle belle voix en prospectif. M. Cohen presque excessive. Comme vous pouvez le le constater : on a là une dynamique au niveau du groupe puisqu'on anticipe les lois et on fait des propositions pour permettre une réflexion déjà sur ses bancs de notre assemblée, et y compris au gouvernement, donc fait très fort, mais pour les raisons qui nous ont été dites, on retire notre amendement, on y reviendra lors de dans prochain examen. Merci, cher collègue, l'amendement 7 quater au Monsieur Rapidement sur le président de la ministre, cet amendement inséré un article additionnel proposant un rapport examinant le recours effectif au télétravail dans les entreprises françaises, évaluant les besoins d'encadrement juridique de ces nouvelles pratiques. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur. en commission la démonstration qu'il avait dit rapport qui avait été demandé comment il est qu'aucun de ces rapports demandés n'a été fait depuis donc c'était pas la peine de demander des rapports supplémentaires puisqu'il a déjà un retard considérable en plus de ça, l'amendement d'autres collègues, est satisfait car les partenaires sociaux ont remis le 27 mai 2017 au gouvernement un rapport sur le télétravail en application l'un de l'article 57 de la loi travail c'est d'ailleurs ce rapport qui a alimenté la réflexion du gouvernement pour réformer le télétravail dans sa 3ème ordonnance donc une demande de retrait sinon un avis défavorable.

Qui est pour. Ce qui est encore entre. Qui s'abstient, il est adopté aussi sur l'article 6 bis qui est pour l'article 6 bis. Qui est contre. Donc il est adopté. Alors je vais suspende la séance à elle sera reprise à 21 heures 30 pour la suite de l'examen de ce texte mais j'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission d'information sur Alstom et la stratégie industrielle du pays a été publié cette candidature sera ratifié si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement, la séance est suspendue, elle sera donc reprise à 21